La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique. De la précédente séance a été distribué. Hé bien. Il n'y a pas d'observation, je n'en vois pas le procès-verbal est adoptée sous les réserves d'usage. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en Direct sur Public Sénat sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat. J'appelle chacun de vous, mes chers collègues, a observé au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect qu'il s'agit du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. Et si l'on pouvait s'écouter dans un relais. Silence. Ce serait magnifique. Merci. La parole est au président Guillaume Gontard, pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Vous avez la parole, cher collègue. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre. J'avais prévu de vous interpeller avec véhémence pour dénoncer les manoeuvres auxquelles se livrent votre gouvernement et vos alliés pour empêcher un vote en séance plénière de l'Assemblée nationale, un vote ne serait-ce que symbolique sur le report de l'âge légal de la retraite. Mais au regard des événements consternants ah devenue ce matin à l'Assemblée. C'est avec une profonde gravité que je m'adresse à vous. Madame, la Première ministre. Les droits des oppositions politiques sont le fondement même de la démocratie. C'est à l'aune de ses droits qu'on juge la qualité d'une démocratie, notre pays à tous les échelons national ou locaux fait déjà pâle figure avec une hypertrophie des pouvoirs exécutif et des assemblées réduite à leur seule fonction tribunitienne. Pour tous nos partenaires européens, régime parlementaire rompu à la négociation et à une certaine culture du compromis notre régime politique est une incongruité pour ne pas dire une aberration. Dernière preuve en date de culture politique très différente. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez remet son mandat en jeu après avoir perdu une élection municipale. Rien de tel chez nous où le gouvernement avance en écrasant toute contestation devant lui. Ce matin c'est bien plus que la bataille de retraite qui est joué à l'Assemblée nationale en torpillant une initiative parlementaire de l'opposition en bafouant le droit d'amendement, en transformant le corset de l'article 40 ans véritable étau vous créez un précédent délétère qui menacent de réduire à néant le droit d'expression déjà famélique des parlementaires madame, la Première ministre, vous êtes une démocrate, vous l'avez clamé ici même en juillet 2022. Comment pouvez-vous tolérer la dérive autoritaire dans laquelle le président vous enferme. Merci. La parole est à madame la Première ministre. Si monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le président Gontard. Je suis souvent surprise d'entendre les mêmes qui se disent défenseurs du Parlement. Être les premiers à en refuser les règles. Monsieur le président Gontard Revenons-en aux faits. L'examen de la réforme des retraites a eu lieu avec 175 heures de débat parlementaire. Elle a été votée par deux fois par le Sénat et le Conseil constitutionnel s'est prononcé très clairement sur la conformité de l'essentiel du texte à notre constitution et sur le rejet de de demande de référendum d'initiative partagée qui visait à l'abroger. La proposition de loi dont vous parlez qui fait actuellement l'objet d'un examen par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale aggraverait considérablement les charges publiques et réduirait les recettes cela contrevient de façon évidente à l'article 40 de notre constitution. Ce texte, vous le savez Monsieur le Président est anti-constitutionnelle et personne n'est dupe de la manoeuvre qui se joue. Monsieur le Président Gothard vous appeler au respect du Parlement au débat je vous je vous renvoie à ses principes. Ce matin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté et à supprimer l'article de la proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites. C'est un vote clair et démocratique, mais immédiatement après la NUPES a répondu par l'obstruction avec le dépôt de 3000 sous-amendement pour empêcher un vote final en commission. La réalité c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES. Elle n'a qu'une réponse l'obstruction. De mon côté je crois en notre constitution et je respecte le travail du Parlement. je souhaite que l'examen de la proposition de loi puisse aller à son terme dans de bonnes conditions et que le contrôle de la recevabilité des amendements puisse exercer normalement dans la sérénité. En somme, je ne souhaite qu'une chose, le respect de nos règles et du débat parlementaire, je vous remercie. Merci monsieur le président Gontard 14 secondes. Madame, la Première ministre d'abord l'obstruction c'est vous toutes les règles tordre les règles, ce n'est pas appliqué les règles madame, la Première ministre, vous pouvez entrer dans l'histoire en ouvrant une page nouvelle de notre république parlementaire vous seriez entrerait hélas comme une faut soyeuse de la démocratie française. La parole est maintenant Madame, Colette Mélot pour le groupe les indépendants République et Territoires, vous avez la parole, cher collègue. Je ne serai pas là demain. Ce sont les derniers mots de Lindsay, 13 ans, adressé par message à l'une de ses camarades de classe. Le 12 mai dernier, Lindsay a décidé de mettre fin à ses jours. Parce que la vie lui était devenue insupportable. 13 ans c'est normalement l'âge de l'insouciance et de la joie de vivre mais pour elle, c'était l'enfer. Parce qu'un groupe d'élèves la harceler tous collèges et sur les réseaux sociaux avec une violence inouïe. L'Insee vient ainsi compléter une liste déjà beaucoup trop longue. Chaque année près d'un million d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire et une vingtaine d'entre eux commet l'irréparable. Madame la Ministre, il faut que cela cesse. Avec ma collègue Sabine Vanek qui vit ce drame dans son département. Nous avons remis notre rapport sénatorial sur ce sujet à monsieur. Monsieur Pap Ndiaye Ministre de l'Éducation nationale. Ce rapport comprend 35 préconisations autour de 3 priorités prévenir détecter les cas et les traiter systématiquement et sans délai. Madame la Ministre, la situation est urgente. Dès qu'un cas de harcèlement, Paris s'est immédiatement que tous les acteurs concernés doivent agir sans minimiser. Les situations le cyber harcèlement. Fait. Son son Oeuvres très rapidement en démultipliant les conséquences graves. L'enfant n'ayant. Plus de répit, même dans la sphère privée. Le programme phare a le mérite d'exister mais il est malheureusement encore loin d'être appliquée dans tous les établissements. Malgré tous les efforts déployés, force est de constater que tout n'est pas mis en oeuvre pour sauver les enfants victimes de harcèlement. Dans le cas de l'Insee, la situation était parfaitement connu dans l'établissement, conclut lesquels aide cette jeune fille a-t-elle reçu. A-t-on vraiment tiré les leçons des drames précédents. Madame la ministre, quelles mesures concrètes, comptez-vous mettre à 9000 immédiatement. Merci. La parole est à Madame. Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, vous avez la parole madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Colette Colette Mélot permettez-moi tout d'abord d'adresser tout mon soutien et toutes mes pensées à la famille de Lindsay. Nous avons fait et vous le savez de la lutte contre le harcèlement une priorité et je sais Madame la sénatrice que nous partageons ce combat et que vous êtes impliqué sur ce sujet depuis longtemps. Vous le savez nous concentrons tous nos efforts pour lutter contre ce fléau délictuel nisation du harcèlement généralisation du plan Farr dans toutes les écoles primaires, les collèges et dès la rentrée 2023 et dans tous les lycées, formation de très grande ampleur pour tous les personnels à la prévention à la détection et à la prise en charge du harcèlement diffusion large des numéros verts 36 18 et 36 19. Et le ministre a annoncé très récemment une procédure spécifique, décret qui viendra en juillet pour déplacer l'élève harceleur, comme l'avait proposé, madame la sénatrice Marie Mercier et pourtant oui, nous sommes de nouveau face à un drame depuis le le suicide de de à l'Automne dernier. La mère de Lindsay avait interpellé la direction de l'établissement parce que l'Insee étaient victimes de violences et de moqueries de la part d'une autre élève de son collège. Cette élève avait fait l'objet d'une exclusion de 3 jours puis en raison d'une récidive cet élève avait été exclu définitivement fin février de ce collège. Ensuite, il semblait que la saison la la la la situation s'était apaisée mais le cyber harcèlement que vous évoquez a continué à l'abri des regards et du contrôle des adultes et des personnels enseignants. C'est un sujet fondamental sur lequel nous devons continuer à travailler, largement souligné dans votre rapport sur le le harcèlement et ce n'est que 3 jours avant ce geste fatal que l'équipe du collège a de nouveau été alertés pour la situation de l'Insee. Mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui des poursuites pénales sont engagées, 4 adolescents et un adulte ont été mis en examen. Du côté de l'Éducation nationale, le ministre a missionné l'Inspection générale pour mener une enquête administrative. Sachez, madame la sénatrice, que l'éducation nationale et ses personnels mettent tout en oeuvre pour éviter ces drames, restons tous solidaires et mobilisés contre ce fléau. Je veux dire. Si Madame la Ministre. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mes chers collègues. C'est à vous madame, la Première ministre que je veux m'adresser et à travers vous au président de la République pour. Soutenir ici dans cet hémicycle. Une cause juste la cause d'un petit peuple oublié un peuple qui a fait l'objet il y a plus d'un siècle d'un génocide et un peuple qui est aujourd'hui aux prises avec une tentative d'épuration ethnique, culturelle et religieuse comme vous le savez depuis près de six mois l'Azerbaïdjan bloquent le corridor de Latchine. Qui relie ce petit territoire à l'Arménie et il fait donc il transforme le Haut-Karabakh en prison à ciel ouvert dès le mois de février, le 22 février, la Cour de justice internationale. A d'Azerbaïdjan de lever le blocus parce que le blocus mettent en danger la vie de 120.000 Arméniens. Dont 30.000 enfants et c'est dans ces conditions. Dans ce contexte que l'Arménie défaite par la guerre des 44 jours. Le sabre sous la gorge. Sa souveraineté désormais mises en jeu menacer son intégrité territoriale aussi. Pourrait envisager d'abandonner le Haut-Karabakh. Dans ces conditions de questions et à ces 2 questions, je voudrais aussi associé. Dans un geste transpartisan mon collègue Gilbert Luc de Vina qui préside le groupe d'amitié franco-arménien. Première question, la France a. Toujours fait du principe d'autres d'autodétermination des peuples est un principe cardinal pour le Haut-Karabakh, comme pour toute sa politique étrangère est toujours le cas. 2ème question l'épuration ethnique n'a jamais été aussi éminente question. Qu'allez-vous faire pour la prévenir pour l'empêcher. La parole est à madame la Première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bruno Retailleau. La France hein avec ses partenaires est pleinement engagée en faveur d'un règlement durable du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous suivons la situation avec la plus grande attention et, je sais votre mobilisation sur ce sujet, monsieur le président. La Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est rendu dans la région fin avril pour appeler les parties à reprendre les discussions, qui était alors bloqués. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union européenne. Les négociations de paix reprennent. C'est un signal encourageant et nous saluons le rôle actif des États-Unis avec qui nous nous coordonnons étroitement. Monsieur le Président, Retailleau. Notre pays est engagé au plus haut niveau pour la paix dans la région. Demain en marge du sommet de la communauté politique européenne de qui. China au le président de la République sera aux côtés du chancelier Scholz et de Charles Michel pour une réunion avec le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais. Il existe aujourd'hui une voix pour la paix. Elle passe par la reconnaissance mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des 2 pays. Elle passe par la délimitation de la frontière commune. Et nous saluons à cet égard les déclarations du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Dans ce conflit, la France n'oublie pas les enjeux humanitaires et les conséquences du blocage persiste persistant du corridor de Latchine. Nous n'avons eu de cesse de rappeler la nécessité de mettre en oeuvre la décision de la Cour internationale de justice du 22 février. Plus particulièrement. Monsieur le Président, Retailleau. Vous avez raison d'évoquer les droits et garanties des populations du Haut-Karabakh qui doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Vous pouvez compter sur le plein engagement de la France pour continuer à trouver des solutions durables et à la paix dans la région. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Retailleau 17 secondes. Madame, la Première ministre je sais l'engagement de la France. Je sais, je reconnais l'engagement du président de la République, mais aujourd'hui, nous devons faire plus, on doit faire plus parce qu'on est à la veille d'une tragédie, on doit faire plus parce que on le doit aux Arméniens à ce peuple frère avec lequel nous partageons tant de notre histoire des Liens des Liens d'affection autant que des Liens de civilisation les Charles Aznavour les compositions d'Alain de Michel Legrand. Les films d'Henri Verneuil dont le prénom était à chaudes et puis aussi l'héroïsme de Manouchian qui bientôt sans doute entrera dans la encore que le dans le côté on. C'est la raison pour laquelle nous devons faire encore beaucoup plus. Merci. Nous avons des devoirs et cela nous oblige madame, la Première. Monsieur il y a des questions. Plus importante. Peut être plus difficile. La parole est maintenant madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste. Vous avez la parole, cher collègue. Merci monsieur le président. Voilà une question difficile, en effet. Vous avez, Monsieur le Ministre Atal. Vous avez présenté hier votre plan de lutte contre la fraude sociale. Je souhaite d'abord vous remercier de convenir que la fraude sociale est une réalité est une fraude aux finances. Publiques a traiter comme tel, je fais ce rappel d'autant plus volontiers que j'ai été traitée de menteuse dans cet hémicycle et support du Rassemblement national par un ministre votre majorité quand j'avais évoqué ce sujet il y a quelques années. 4 ans plus tard, de graves dysfonctionnements demeure les fraudes sont évalués à 6 à 8 milliards. Froget de basse, la Cour des comptes relève le taux important de fraude documentaire et demandent la sécurisation d'immatriculation des bénéficiaires. Faute de sécurisation, nous construisons vous construisez sur du sable vous présenter des mesures ponctuelles utile mais vous abandonner la voie de la biométrie voter 2 fois ici au Sénat pour un système de fusion entre la carte nationale d'identité et la carte vitale. Il y aurait entend-on des voix divergentes au sein du gouvernement pour cet outil dont la mise en chantier prendra des années. Pouvez-vous nous donner Monsieur le Ministre, le calendrier de la mise en place de cette mesure est justifiée. Votre choix quand on connaît le temps qu'il faut aujourd'hui en France pour avoir une carte nationale d'identité. Merci cher quoi. La parole est à monsieur Gabriel. Attal Ministre délégué chargé des Comptes publics, vous avez la parole. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Nathalie Goulet. La lutte contre la fraude sociale, comme la lutte contre la fraude fiscale est fondamental. Et quand on parle de lutter contre la fraude sociale, on parle tout simplement de garder le contrôle sur notre modèle social. En reprenant le contrôle de ce qu'on donne et à qui on le donne et je voudrais commencer ma réponse en vous remerciant. Vous avez travaillé depuis de nombreuses années sur ce sujet, vous avez commis un rapport très important en 2019 avec ma collègue Carole Granjean qui était député à l'époque vous avez participé au groupe de travail que j'ai mis en place pour l'élaboration de ce plan et plusieurs mesures de mon plan viennent directement de propositions que vous aviez émises j'en cite une à partir du 1er juillet prochain. Nous ne verserons plus d'allocations sociales sur des comptes bancaires C'est vous qui aviez fait cette proposition et nous l'avons reprise vous m'interrogez sur la carte Vitale biométrique. C'est une proposition effectivement qui a été émise à plusieurs reprises ici même nous avons confiée à l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances, une mission sur le sujet, le rapport a été remis à quelques jours, il est à votre disposition, que dit ce rapport. ça coûterait très cher, 250 millions d'euros par an. De il y a de vrais freins juridiques et la CNIL s'oppose à cette mesure. Trois, il y a des freins pratique les syndicats de médecins dans le rapport disent eux-mêmes qui s'y opposent et par ailleurs il y a des fins pratiques aujourd'hui si vous êtes cloué au lit, que vous envoyez votre proche chercher vos médicaments à la pharmacie. Si vous donnez donnez si vous devez donner vos empreintes pour avoir vos médicaments. Convenez que c'est assez compliqué. La mission IGAS IGF recommande une autre voie de sécurisation de la carte vitale en faisant migrer la carte vitale. Sur la carte d'identité et c'est cette voie que nous avons décidé de poursuive ça permettra de lutter davantage contre la fraude à l'identité pour l'accès aux soins dans notre pays par exemple à travers du tourisme médical illégal. Nous venons de lancer avec Gérald Darmanin et François Braun, une mission de préfiguration pour déterminer le calendrier et les modalités. L'objectif c'est d'aller vite mais évidemment qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accès aux soins et aux droits pour les Français, on sait qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour renouveler ses titres d'identité évidemment tel chantier une telle bascule ne peut s'envisager. Donc on n'est pas revenu à la normale même si la Première ministre a annoncé des moyens très importants pour qu'on puisse revenir à des délais normaux. Donc la mission de préfiguration sera lancée d'ici à l'été. remises. Merci Madame Goulet. Oui monsieur Ministre vous savez qu'il y a des mesures urgentes à faire, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a absolument pas de lien par exemple entre le titre de séjour en France et et les droits sociaux. Vous avez quelqu'un dont le titre de séjour expire et dont la carte vitale continuent à fonctionner. Vous avez aussi dans le rapport de la Cour des comptes du 24 mai. Un chiffre un peu étonnant de 58 millions de cartes Vitale actives, ce qui fait un surnombre de deux millions six alors que, là, l'administration a refusé de fournir à la Cour des comptes. Le nombre de cartes Vitale actives par année de naissance qui permettrait évidemment de contrôler l'exactitude de ces cartes vous avez également 44.000 Near frauduleux. Vous avez un fichier âgé de rêve pour les étrangers. Remplacé par l'administration numérique des étrangers en France qui ne fonctionne pas dans la cour dit que c'est toujours pas pas opérationnel. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de dysfonctionnements majeurs. Il faut absolument les régler sinon votre plan ne sert à rien. Merci. La parole est maintenant monsieur. Pierre Ouzoulias. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme tous les ans, presque 900.000 candidats ont soumis non sans angoisse, leurs à la procédure Parcoursup comme tous les ans depuis 2018. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les modalités, les critères et finalement l'intelligibilité des conditions d'examen des dossiers par certains établissements, il est admis par exemple que certaines filières réalise une première sélection des dossiers par le seul l'usage d'un algorithme. En outre, comme l'a révélé la Cour des comptes 20%, des commissions d'évaluation intègrent dans leurs critères celui du lycée d'origine. Certaines d'entre elles pourraient même pondérer les notes du contrôle continu par le rang de classement de celui-ci ce qui pénalise les élèves issus des établissements des communes populaires. Notre groupe s'est opposé à cette sélection qui est imposé par le manque de place et le sous-investissement chronique dans l'université nous estimions à l'inverse que la France a l'impérieux devoir de former plus d'ingénieurs plus de techniciens et plus de diplômés de l'université pour affronter les défis climatiques technologiques et sociaux, mais dans l'immédiat. Considérons avec la Commission européenne, le Conseil constitutionnel. La Cour des comptes, le défenseur des droits, le comité d'éthique de Parcoursup et la commission de la culture du Sénat qu'il est impérieux de présenter de façon explicite au candidat les procédures d'examen de leur dossier. Certains établissements ont usé et abusé d'une dérogation législatif discutable pour s'affranchir de l'obligation faite à tous les agents publics de rende compte de son administration. Comment pouvons-nous reprocher aux Gafam via TikTok de nous cacher leurs algorithmes et accepter l'opacité de ce de Parcoursup. Merci monsieur le président. Merci cher collègue. La parole est à madame Sylvie Retailleau Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Ouzoulias. Alors d'abord je voudrais vous dire combien je partage avec vous cette ardente et je dis bien ardente obligation de la transparence, en particulier quand il s'agit de l'avenir de l'avenir de nos jeunes, non pas parce que nos enseignants profiterait de l'opacité pour pouvoir faire de la sélection discriminante mais parce que la transparence était fait la transparence pardon. Et effectivement le levier un levier pour accompagner en particulier une meilleure orientation pour nos jeunes, mais aussi un levier pour pour rendre les résultats de Parcoursup plus prévisibles et donc diminuer le stress pour les étudiants, les élèves et leurs familles. Alors depuis 5 ans, que faisons-nous. Eh bien depuis 5 ans l'amélioration continue de Parcoursup accompagne cette meilleure de ces critères que vous appelez les critères d'analyse de nos formations là où il n'y avait rien. Nous avons expliqué les attendus. Et oui, nous avons rendu obligatoire l'affichage des critères. Pour cette session 2023, nous avons été à l'écoute, puisque nous avons refondu complètement la manière dont sont présentés ces critères pour apporter effectivement une information plus précise plus transparente au candidat les formations de Parcoursup, incluant les classes préparatoires devront produire aussi en fin d'année un rapport sur les critères utilisés et ce rapport sera rendu public sur la plateforme. Approfondir la transparence, c'est évident. Hé mais c'est aussi préserver le secret des délibérations collégiales des enseignants. Ce n'est pas un réflexe corporatiste ou une volonté de sauvegarde de l'opacité. C'est la conviction que la délibération des enseignants que l'on connaît parce que je voudrais insister sur le caractère humain de Parcoursup, qui a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2020 et la garantie d'un regard humain derrière Parcoursup. Il y a des commissions d'examen, il y a des enseignants qui travaillent et je voudrais profiter de cette occasion pour et insisté sur le travail à tout niveau de nos collègues je je finirai par dire que je sais que demain s'ouvre la période pour nos étudiants leur famille de de des résultats des voeux et je voudrais leur dire que l'on pense à eux que je pense à eux et que tout est fait pour les la compagnie. Madame la ministre. Merci. Essayer de penser à eux. Mais si possible dans les 2 minutes. Allez monsieur Ouzoulias s'une poignée de secondes poignée. Merci, monsieur le Président Madame. La Ministre c'est un discours que j'entends depuis 2018. Il faudrait que maintenant les choses changent. L'université était un service public il faut que votre ministère se donne les moyens d'examiner établissement établissements les conditions dans lesquelles est réalisé cette sélection. Merci Monsieur le Président. Merci. La parole est maintenant à monsieur Bernard buis pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole, cher collègue. Merci. Si monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre délégué chargé des Comptes publics. vous avez annoncé un vaste plan de lutte contre la fraude sociale fraude multiforme, évalué à 11 milliards d'euros qui rassemble aussi bien et les cotisations sociales éludées. La fraude aux prestations de santé ou aux allocations sociales. La fusion de la carte vitale avec la nouvelle carte nationale d'identité. Mesure phare de votre nouveau plan soulève plusieurs interrogations, tant sur sa mise en oeuvre technique, que sur la protection des données. Déjà adopté par plusieurs pays européens dont la Suède, le Portugal ou la Belgique. Cette carte d'identité, une fée électronique Hybrid permettrait pourtant de renforcer les contrôles afin de résorber les fraudes aux prestations sociales. Vous avancez également que dans 70% des cas, la fraude aux prestations de santé est à l'initiative d'un professionnel, par le biais de surfacturation ou de facturation d'actes fictifs l'an dernier, l'assurance maladie aurait ainsi détecté 300 millions d'euros de fraude vous chiffrez également les arrêts maladie dits de complaisance à 30 millions d'euros entre 2017 et 2022. Par conséquent, Monsieur le Ministre, quels sont les moyens que vous comptez. Pour détecter et lutter contre ces prescriptions abusives. Merci pour vous répondre. La parole est à monsieur Gabriel Attal Ministre délégué chargé des Comptes publics, vous avez la parole. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Bernard, lui. Oui vous avez raison, la lutte contre la fraude sociale nécessite des moyens. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé un renforcement des effectifs de contrôle de l'ordre de 20% sur les 5 prochaines années et un investissement massif dans les systèmes d'information. Un milliard d'euros pour moderniser les systèmes d'information des caisses de Sécurité sociale sur les 5 années qui viennent et il y a du chemin à parcourir. J'étais d'ailleurs c'est une recommandation qui m'avait été faite d'aller. En Belgique pour rencontrer la Banque Carrefour, de la sécurité sociale, on voit à quel point leur système de données sont plus performants. J'étais hier à la Caisse nationale d'allocations familiales. On m'a présenté un dossier tout à fait édifiant. Dans le département du Val-de-Marne 437 dossiers de non conformités identifiées. Il s'agissait venant de Roumanie, de personnes qui avaient fait des fausses déclarations de de résidence des fausses déclarations de salariés en France 8 millions d'euros de préjudice. Sur le seul département du Val de Marne via le numérique, on doit renforcer renforcer nos outils de détection et de sanctions. D'où l'investissement que j'ai annoncé sur la question des de la fraude aux prescriptions de santé que vous avez. C'est une réalité dans notre pays. Il ne faut pas stigmatiser évidemment l'écrasante majorité la quasi-totalité des professionnels de santé font les choses dans les règles et donnent de leur temps pour les autres et pour leurs patients mais il y a des fraudes. L'an dernier nous avons déconventionner 5 centres de santé notamment dentaires et en ophtalmo qui surfacturé à l'assurance maladie, un certain nombre d'actes qui en réalité n'avait pas été réalisés auprès de patients et donc j'ai annoncé dans le plan un dispositif. Nous allons faire en sorte que désormais compte des Français des patients sortent d'un centre de santé, ils reçoivent automatiquement par SMS. La liste des actes qui ont été. Fifine facturés à l'assurance maladie par le Centre de santé ils se rendent compte qu'il y a des actes qui ne leur ont pas été réalisées pour le signaler avec un bouton de signalement. Ce qui permettra à l'assurance maladie d'orienter ses contrôles vers les centres de santé ou les professionnels pour lesquels il y a le plus de suspicion de fraude. Voilà une mesure parmi d'autres, vous avez raison comme vous, je considère qu'il faut lutter implacablement contre ces fraudes. C'est ce que nous faisons avec mes collègues du gouvernement, évidemment François Braun Jean-Christophe. Combe singulièrement sur les prestations sociales et l'assurance maladie et je sais pouvoir compter et je votre soutien. Merci Monsieur le Ministre pour ses moyens annoncés qui je l'espère et nous l'espérons tous permettront de lutter contre cette fraude sociale qui gangrène notre pays. Merci. La par les maintenant Monsieur Bernard Jomier. Pour le groupe socialiste. L'écologiste et républicain. Merci monsieur le président avant de poser ma question je voudrais saluer madame, la Première ministre pour ses propos concernant Pétain et le Rassemblement national. Certes, Certes, la politique ne se résume pas à des positions morales mais celle-ci, eu égard à votre fonction. Et en particulier à votre histoire personnelle mérite le respect. Ma question sera simple. Un protocole thérapeutique a été mis en oeuvre jusqu'au 31, de 102.021 dans notre pays et puis y'portant sur 30.000 personnes et en violation flagrante de la loi protégeant les personnes soumises à une recherche médicale. C'est un fait inédit et c'est un fait grave sans précédent. Alors Monsieur le Ministre. Pourquoi une telle inertie des pouvoirs publics face à ce scandale. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que se déclenchent enfin une action et on l'a vu ce matin. Pourquoi. N'avez-vous pas pris les mesures. Pour mettre fin à ce scandale et que comptez-vous faire maintenant. Nous parlons ici d'une. Étude. Qui a été présenté en preprint c'est-à-dire qu'il n'est pas encore acceptée par des revues scientifiques. Heureusement, devrais-je dire, qui porte sur 30.000 patients qui ont été traités à l'institut hospitalo-universitaire Marseille Méditerranée pour dire les mots en dehors de tout cadre d'expérimentations cliniques en dehors de tout cadre d'utilisation des médicaments puisqu'ils étaient utilisés or. And AMM autorisation de de mise sur le marché. Alors concernant cet, cet institut en plus médicaments je je tiens à le préciser, qui avait déjà fait la preuve de leur inefficacité dans le cadre du traitement de la Covid 19. Par rapport à cette situation une enquête IGAS ESR nous a rendu ses conclusions en septembre 2022 à ma collègue, Sylvie Retailleau et moi-même nous avons immédiatement saisi le procureur de la République de Marseille par le biais de 2 articles 40 devant la constatation dans cette enquête de pratique aussi bien managériales que de suivi des études cliniques. Inappropriées voire déviantes. Nous avons dans les suites convoquer l'ensemble des administrateurs de cet IHU en leur. Imposant la mise en place d'un plan de redressement sur la base des conclusions de cette enquête IGAS GES Comme vous je déplore ce nouvel. Épisode inadmissible de cette affaire sachant que la justice étant est en train de suivre son cours comme vous avez pu le le constater avec moi dès ce matin. où cette proposition de publication qui pour moi s'apparente à de la provocation, nous serons amenés et d'étude est en cours avec le service juridique à prendre avec ma collègue, Sylvie Retailleau pour l'enseignement supérieur, la recherche et moi-même toutes les mesures nécessaires, envers l'ensemble des signataires de cet article, je vous remercie. Merci Monsieur Jomier. Monsieur le mini et je pense que vous-même avait conscience de la faiblesse de votre réponse. Il y a 2 ans. Les alertes étaient déjà nombreuses. Les rapports de l'ANSM. Le rapport de l'IGAS et bien avant. En 2015, l'INSERM quitter le conseil d'administration de l'IHU Méditerranée. Café, l'université d'Aix-Marseille pour mettre fin à ces dérives. Rien. Qu'avez-vous fait messieurs les ministres, monsieur Véran. Vous étiez ministre de la Santé, vous n'avez pas répondu à la question écrite que j'ai déposé concernant les dérives de l'IHU madame Frédérique Vidal, ministre de la recherche n'a pas répondu non plus à mes questions. Hé bien si l'ensemble des institutions de notre pays et les ministres se sont tus et ont fait preuve de faiblesse. C'est peut-être parce que le chef de l'État et à couvrir de sachets l'heureux immunité le patron de l'IHU et c'est un dysfonctionnement grave de nos institutions. Merci cher Merci cher collègue. La parole est maintenant Monsieur Bernard filles à l'air pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, cher collègue. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et une fois n'est pas coutume dans cet hémicycle. Je voudrais parler d'amour. L'amour en général passe par l'amour de la langue qui n'est ni nationaliste ni conservateur mais qui exigent des preuves et des épreuves on ne fait pas n'importe quoi avec la langue ces mots de Jacques Derrida sont repris par le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. Dans le rapport au Parlement sur la langue française. Et pourtant. Le 10 mai 2023 à l'université Lyon II l'énoncé d'un examen de licence en droit était rédigé dans un langage inclusif excessif par son intégrisme. Toulouse avec un Z à la place de tous. Als pour il ou elle mais aussi professionnels appel à été reconnu que Aussi incompréhensible. Pourtant, la langue de la République est le français essentielle à notre lien social pour Michelin même l'identité de la France, c'est sa langue d'ailleurs à l'article 2 de la Constitution, il était écrit la langue de la République est le français. Tous les citoyens ont ainsi le droit démocratique garanti par la loi de recevoir une information et de s'exprimer dans leur langue. La loi Toubon affirme. Le droit aux Français pour que l'ensemble de la société puissent se comprendre et échanger. Et plus loin d'ailleurs dans l'enseignement et la recherche. C'est la langue de l'enseignement des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires. Il s'agit de redonner à ce cadre légal toute sa dimension politique et d'agir pour maintenir son efficacité. Ces mots sont dans le rapport au Parlement. La circulaire du 6 mai 2021 adressé aux personnels de l'Éducation nationale énonce les mêmes principes pour les actes administratifs et les pratiques d'enseignement. Madame la Ministre à l'université dans le respect absolu de la liberté académique à laquelle nous veillons tous. Que pouvez-vous faire pour que la liberté de pensée d'innover, de créer se fasse avec le vocabulaire des actionnaires officiel de l'Académie française qui n'est pas figée,

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur fiel air merci beaucoup. D'abord pour votre question je. Excusez-moi. D'abord je voudrais me permettent de compléter. Juste pour rappeler 2 éléments importants sur le cadre normatif, vous en avez rappelé. Dans lequel nous nous plaçons effectivement le 1er c'est la circulaire de 2017 du Premier Ministre de l'époque Édouard Philippe sur les règles de féminisation qui s'applique aux actes de nature juridique et aux textes administratifs et il le dit clairement dans un souci de clarté et d'intelligibilité immédiat de ces documents. Autant d'impératifs auxquels je suis auquel nous sommes également attachés donc en espèces. Elle ne s'applique pas aux sujets d'examen effectivement. Car dans l'enseignement supérieur, vous l'avez dit les enseignants-chercheurs sont en fait entièrement libre. Quant au sujet de leur cours mais aussi de leurs sujets d'examen et leur formulation. L'université, pas plus que le ministère effectivement vous l'avez dit sur la liberté académique n'exerce directement de contrôle ni sur les sujets ni sur le contenu pédagogique des enseignements, sauf en cas de propos diffamatoires injurieux ou discriminatoire. Donc juste pour appeler dans le cas de Lyon, sur lequel vous m'interrogez effectivement les preuves en droit de la famille proposer un choix entre 2 sujets qui permettait l'un comme l'autre d'aborder une épreuve du droit de la famille. Toutes 2 traitée dans le cadre des enseignements dispensés mais si l'un des deux sujets proposé a été rédigé dans une forme d'écriture dite inclusive et je n'en dirai pas plus que ce que vous avez décrit l'autre était effectivement parfaitement classique. Cela étant, si votre question est encouragé vous l'usage de l'écriture dite inclusive dans les sujets d'examen ou contrôle ou tout document sous forme utilisant des points médians ou des mots comme vous l'avez prononcé ma, ma réponse est clairement non et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il se trouve que je suis comme vous et je crois que beaucoup d'entre nous ici affiché à notre belle langue. Il se trouve que je suis aussi très attentif aux questions de représentation. C'est pourquoi notre langue est suffisamment riche pour s'exprimer sans véhiculer de stéréotypes de genre et c'est pourquoi nous développons les guides pour pouvoir aider et pouvoir ne pas tomber dans cette caricature par rapport aux examens, je vous remercie. Allez, allez, on se calme. Orateur ou réponse des deux minutes c'est deux minutes c'est pas deux minutes 25 2 minutes 30. Monsieur le rapporteur général Jean-François Husson à la parole pour le groupe. Les républicains. Madame la Ministre, 2022. Année record en matière de saisie de drogue mais 2022 forcé de le reconnaître. C'est aussi une montée inexorable de la violence liée au trafic de drogue. C'est aujourd'hui un phénomène qui gangrène nos territoires des grandes villes en passant par les villes petites et moyennes. Mais même aussi les territoires ruraux qui subissent aujourd'hui une spirale de règlements de comptes avec utilisation d'armes à feu. Hé bien sûr, fusillade. Le Creusot qui arpentera. Mais aussi. Orléans Chambéry. Valence à mort et dans mon département de Meurthe-et-Moselle ville rue. 5 blessés dont 3 blessés graves. Madame la Ministre, comment l'État répond-il aux appels à l'aide des populations et des élus locaux. Face à ces populations qui d'ailleurs sont souvent sous sous l'emprise d'une forme de terreur. Quels moyens déployés en termes de surveillance de force de protection et de sécurité et dans une zone police comme cette de ville rue quel plan d'action concret, comptez-vous mettre en oeuvre. Merci monsieur le rapporteur général. La parole est à Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales la ruralité. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur général. On partage le constat je vous demande de bien vouloir excuser Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Herrmann est en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Les villes que vous avez cité Villerupt dans votre département. On fait l'objet d'une fusillade. J'ai été moi-même ici. En échange. Avec vous-même ou un de vos collègues, il y a 15 jours sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur s'est mis en capacité de se mobiliser immédiatement à tout acte de violence, il y a des trafics de stupéfiants, que cela soit dans les des grandes villes ou dans les villes de taille moyenne, un effort significatif a été fait sur les renforts policiers avec des ouvertures de postes importante lors du mouvement général 2023 plus 11 postes ouverts pour la CSP de Longwy dont dépend la commune de Villerupt et plus 44 postes ouverts sur le département du Meurthe et Moselle, Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus global avec notamment une augmentation de 8500 postes pour la police nationale et la gendarmerie nationale sur 5 ans grâce à la Lopmi. Par ailleurs, une concertation permanente avec les élus locaux ont été mises en place, je vous l'avez dit, elle a eu lieu le 26 mai, le préfet reçu des élus de Meurthe-et-Moselle afin d'échanger sur les différents axes d'amélioration possibles pour la sécurité du territoire, plusieurs propositions ont été mises sur la table et vont faire l'objet de nouveaux échanges avec les élus lors d'une réunion place Beauvau le 5 juin. L'ensemble des préfets. Je je je le rappelle, sont à la disposition des élus pour adapter les dispositifs de sécurité aux anges et notamment pour garantir la mise en oeuvre des instances locales. De sécurité. Mais pour mettre en oeuvre les financements de la vidéoprotection. Par exemple, je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur général. Francis. Madame la Ministre. Finalement. J'ai assisté à la réunion du du 26 mai. Mais vous savez ce que vous venez de dire, ça fait plus d'une décennie. Qu'avec des gouvernements successifs. Ces éléments sont donnés mais finalement les effectifs de police ne sont jamais à la hauteur aujourd'hui à Villerupt Longwy 70 personnel là où il en faudrait 95 78 personnel là où il en faudrait 95 annonces du ministre

c'est de prendre en compte la gravité de la situation. Faut-il attendre des événements encore plus grave pour que aux côtés des collectivités territoriales, l'État sache mobiliser. Nous comptons sur l'état. Là. Parole est maintenant madame Florence Béatrice compta pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Chers collègues. Merci monsieur le président. Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui partout en France, les enseignants manifestent le refus du pacte que votre gouvernement propose car le compte n'y est pas, loin de là et loin notamment de la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 10%, tous les enseignants en septembre prochain. L'éducation nationale vit une véritable crise d'évocation, le nombre d'inscrits au concours en 2023 est en nette baisse par rapport à 2021 et les démissions ainsi que les ruptures conventionnelles ont été multipliés par 5. La dégradation des conditions de travail et du pouvoir d'achat en sont les principales causes. L'enjeu de cette revalorisation aurait aurait donc dû concerner la partie socle c'est-à-dire inconditionnel. Mais en réalité, elle est loin de rattraper les baisses de pouvoir d'achat de 15 à 25% de ces vins de de de ces 20 dernières années ni de rivaliser avec nos voisins européens. Alors qu'un enseignant débuté sa carrière à 2,2 SMIC. Dans les années 90, il est aujourd'hui à 1,2 SMIC. La rémunération des enseignants est inférieure de 15% à ceux de l'OCDE et je ne parle pas de nos voisins allemands. C'est donc cette enveloppe socle qu'il faut avoir le courage d'augmenter fortement et qu'il faut traduire par un relèvement des points d'indice et non par des primes. Quant à la part d'augmentation en échange de missions supplémentaires, elle n'est en aucun cas et de revalorisation salariale. C'est une provocation alors même que les enseignants français travaillent davantage que leurs homologues européens et avec davantage d'élèves ça contribue draps à dégrader encore les conditions d'enseignement, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus. Allez-vous Madame la Ministre entendre les enseignants et assurer à tous les personnels, une augmentation salariale sans contrepartie qui rattrape les pertes de pouvoir d'achat et qui traduisent la considération de la nation. Merci pour vous répondre. La parole est à Madame. Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Béatrice blattes Je vous rappelle que le pacte enseignant est l'un des deux volets que le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre pour revaloriser le le métier d'enseignant ainsi que sa rémunération pour rendre ce métier plus attractif. Nous sommes face à un enjeu crucial de mise à niveau des rémunérations et de recrutement des professeurs pour les prochaines années sur la revalorisation inconditionnelle qui va bénéficier donc à tous les enseignants ainsi que monsieur le président de la République s'était engagé à compter de la rentrée prochaine tous les nouveaux professeurs titulaires débuteront à plus de 2000 euros nets par mois. Par ailleurs, l'ensemble des professeurs connaîtront une augmentation de mensuel de leur rémunération nette de 95 allant allant jusqu'à plus de 200 euros se sont ainsi 850.000 professeurs et personnels d'éducation et d'orientation qui vont bénéficier de cette augmentation. Cette revalorisation de tous. Représente 2 tiers de l'enveloppe globale et inédite de 3 de 3 milliards d'euros inscrite budget du ministère à cette augmentation inconditionnel s'ajoutera uniquement pour les professeurs volontaires, j'insiste sur ce point, une rémunération supplémentaire en contrepartie de missions complémentaires chaque mission sera indemnisé 2250 euros brut par an, un professeur pouvons choisir plusieurs missions ainsi par exemple la professeur qui choisira trois missions sera rémunéré en plus de sa rémunération de base à hauteur de 3750 euros brut par an pour le cas des lycées professionnels pour lesquels j'ai engagé une réforme d'ampleur. La rémunération des professeurs volontaires pour ce pacte sera un forfait annuel de 7500 euros brut. L'objectif est donc clair, il ne s'agit nullement d'imposer à toutes un quelconque travailler plus pour gagner plus mais bien pour toute émission complémentaires de rendre un service public de l'éducation plus efficaces pour nos élèves et de valoriser l'engagement des enseignants. Je vous remercie. secondes. Madame la Ministre, vous n'avez pas pris la mesure de la situation, nos enseignants méritent une juste revalorisation salariale votre réforme n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle va au contraire des organiser notre système scolaire et dégradé les conditions de travail. Merci.

Le 11 mai, a rendu une décision par laquelle il annule le règlement de l'Institut des langues de l'université de Grenoble parce que il fut écrit en écriture inclusive, utilisant à la foire. Le point médian et le langage de genre. Le tribunal explique clairement que ce règlement est illisible et qu'en tout cas il n'est pas écrit en français et il n'est pas conforme à la Constitution. Quelques jours après. Dans une interview au Figaro. Madame la Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est quand même en charge de former nos élites. Explique que finalement au titre des libertés académiques on peut accepter l'écriture inclusive. Alors madame, la Première ministre mais qui faut-il croire. Le président de la République. Qui à Villers-Cotterêts. Le temple de l'écriture et de la langue française avait affirmé que c'était un véritable trésor qu'il fallait le protéger. Ou faut-il croire vos ministres qui s'explique à l'envi que finalement on peut accepter l'écriture inclusive qui détruit la langue française. Pour vous répondre. Pour vous répondre. La parole est à madame Sylvie Retailleau Ministre de l'enseignement supérieur et la recherche. Si Monsieur le Président. Merci. Mais ça vous messieurs les sénateurs. Ont monsieur le sénateur blanc alors merci déjà de me donner l'occasion de repréciser. Je sais, excusez-moi, mais il y en a. Merci monsieur le sénateur. de me donner le, l'occasion de préciser, non comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pour l'utilisation de l'écriture inclusive. Je crois que vous avez et c'est pour ça que je ça ça me donne l'occasion quand on explique, de l'écriture à ce Clusif avec des points médians ou bien, comme ça a été. Redit tout à l'heure des exemples qui sont proches, non respect de la langue française. Mais quand on dit cher toutes et tous ceux que j'appelais l'expression et c'est d'inclure l'ensemble c'est très différent de la clique inclusif et cela me donne l'occasion et je vous en remercie de le réexpliquer tout d'abord Monsieur le Sénateur, je vous sais très attaché aux libertés académiques dont on parle aussi ici par rapport au sujet de Lyon puisque effectivement le cas de Grenoble tombe sous la coupe de la circulaire. Et donc le as le tribunal administratif a rendu, vous le savez, vous l'avez rappelé, dans le cadre de vos travaux avec le sénateur Gattolin sur les ingérences étrangères. On ne peut pas être pour la liberté académique, l'autonomie des universités et fut. Si j'ai continûment le ministère pour qui la paire viennent à tout bout de Champ pour régir le contenu de ce que proposent les enseignants et les enseignants-chercheurs. Je voudrais juste rappeler pourquoi cette liberté académique est importante, ce qui nous empêche pas de donner effectivement des consignes claires en nous appuyant sur les circulaires qui existent pour pouvoir respecter la langue française comme on se doit de la respecter et avoir des sujets des examens et en enseignement au niveau d'une langue intelligible claire, ce qui est important, je vous rejoins là-dessus pour l'enseignement de tous nos étudiants je vous remercie. Merci monsieur Blanc. Oui merci. Le moins qu'on puisse dire. Madame la Ministre c'est que votre réponse est quelque peu ambigu en tout cas elle n'est pas clair. Et d'abord vous ne répondez pas aux dispositifs fois au jugement du tribunal de Grenoble sur l'inintelligible IT et surtout sur le problème constitutionnel et puis vous ne répondait pas à l'Académie française qui en matière d'écluses de d'écriture inclusive parle d'un péril mortifère. Elle parle d'une aberration alors et Camus disait et tout le malheur des hommes provient du fait qu'ils ne tiennent pas un langage clair. Eh bien moi j'invite aujourd'hui le gouvernement à tenir un langage clair, l'écriture inclusive, c'est oui ou c'est non. Si c'est non décidée enfin que tout texte de quelque nature qu'il soit écrit en un clic, en écriture inclusive est nul de plein droit

La Première ministre a présenté. Voilà 10 jours. Le les pistes du gouvernement concernant la transition écologique. Et elle a annoncé qu'un plan d'action seraient proposées à la fin juin. Bien entendu, monsieur le président. Nous sommes tous attachés à la transition écologique et en particulier pour aller vers une énergie de plus en plus décarboné. Mais il nous semble important de tenir compte à la fois des réalités économiques à la fois des réalités territoriales des réalités sociales. Ainsi. Nous sommes particulièrement inquiets concernant le projet d'interdiction d'installation de chaudières à gaz. Parce qu'il est transparent. Il transparaît dans les propos que cela pourrait survenir. Or aujourd'hui. Plus d'un logement sur quatre. Ah comme mode de de d'énergie le gaz. Il est donc important de tenir compte de cela et je souhaitais connaître les intentions réelles du gouvernement. À cet égard. Pour vous répondre. La parole est à madame Agnès. Pannier-Runacher Ministre de la Transition énergétique. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les députés, Monsieur le mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Canivez. Le président de la République nous a fixé un objectif clair en matière de transition énergétique. Être le 1er pays. Industriel à sortir des énergies fossiles et c'est une condition, si nous voulons atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Ce défi est immense, vous le savez, nous ne pouvons le réussir que grâce à la mobilisation de chacun d'entre nous. C'est pourquoi le gouvernement travaille sous l'égide de la Première ministre a des feuilles de route secteur par secteur pour décarboner et notamment évidemment sur le secteur du bâtiment et du logement. Et vous le savez dans le bâtiment 47% des émissions de CO2. Si on regarde l'usage du bâtiment, ce sont ces liées au chauffage au gaz. Alors on le sait, réduire les énergies fossiles dans ces logements c'est réduire la facture c'est réduire notre dépendance à des énergies importées. Et donc augmenter notre souveraineté et c'est agir contre le dérèglement climatique. Ce mouvement, il n'est pas nouveau puisque les dispositifs ma prime Rénov'permettent aujourd'hui déjà d'accompagner les Français qui souhaitent changer de chaudière et avoir une chaudière non fossiles et nous avons également pris une mesure importante qui est de ne pas permettre l'installation de chauffage au gaz dans les bâtiments neufs. Nous allons continuer à travailler. C'est tout l'objet de la concertation que je vais lancer avec mes collègues Christophe Béchu et Olivier Klein, pour faire en sorte de trouver par anticipation et en nous projetant dans la durée les meilleures solutions permettant à la fois de construire les filières alternatives. au chauffage à gaz et vous savez que nous avons des positions non négligeables sur les pompes à chaleur par exemple mais également de faire en sorte que les Français où qu'il soit sur le territoire et quel que soit leur type de de logements puisse être accompagnées dans l'évolution de leur mode de chauffage et au final pour tenir nos trajectoire de baisse de gaz et émission de de à effet de serre. Je sais que vous y êtes particulièrement attaché, nous lancerons donc prochainement cette concertation et vous pouvez compter sur nous pour le faire de manière pragmatique éduquer mais pour ne pas perdre de vue l'ambition climatique que nous quoi. Si Madame la Ministre Monsieur K navette et lui seul monsieur. Merci Monsieur le Président je comprends et je partage cette ambition d'économie décarboné. Madame la ministre. Mais je dois rentre le gouvernement attentif au fait que nous ne pouvons nous contenter d'une seule source d'énergie. Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait un mix énergétique qui permettent d'assurer la réelle souveraineté de notre pays en s'est aperçu cet hiver que de se reposer sur la seule situation de l'électricité pour tous les usages nous amenait à quelques déconvenues et donc il importe que dès à présent nous prenions bien cela en compte et sur les territoires ruraux en particulier, on sait bien que nous avons des foyers qui ont des moyens très limités et on sait que la production de gaz renouvelable peut apporter à la fois des solutions économiques à notre pays, mais aussi des solutions intelligentes pour. L'énergie de nos territoires. Donc soyons attentifs à cela. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Cristina plus chez pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, l'actualité de mon département l'heure me conduit à évoquer l'exclusion des enfants porteurs de handicap a prise en charge complexe en l'occurrence certains cas d'autisme. OK. La République ne garantit pas un droit descend à l'éducation. D'ailleurs le 17 avril. La France a été condamnée par le comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Pourtant. De nombreux Budgets ont été mis sur la table depuis des années le virage de l'inclusion a été engagée et tant mieux mais je crois Madame la Ministre qu'on soit passé d'une extrême à l'autre. Inclure qu'la prise en charge et compliqué. Ce n'est pas laisser ses enfants à domicile pendant plusieurs années avec un saupoudrage d'intervenants ponctuels à temps très partiel générant la rupture professionnelle d'un parent et sa précarité économique. Inclure ce n'est pas hypertrophiée les moyens alloués à la comitologie et à la concertation au dépens de la création effective de places en structure d'éducation adaptée. Inclure c'est comprendre que le milieu dit protégé a toute sa place parmi les propositions comme lieu d'expertise au bénéfice des enfants dont la prise en charge et la plus complexe. Alors Madame la Ministre qu'avez-vous prévu pour résorber le problème de l'embouteillage dans les instituts médico- éducatifs pour la rentrée prochaine. Quelle solution digne allez vous proposer à ses parents désespérés qui en sont même à se mettre en grève de la faim. Et qu'elle voit de financement allez vous mettre en oeuvre pour sortir des éternels effets d'annonce et fléché enfin les Budgets vers la création de places supplémentaires. Madame la Ministre, ces enfants ne sont pas des enfants de la Republika à temps partiel, ils ont comme les autres. Le droit à une éducation à temps complet.

Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pucher je vous remercie de votre question, elle va me permettre de faire un point. Effectivement, j'ai rencontré aujourd'hui le maire de pause. Dans votre département et et il a des préoccupations très légitime de papa mais là aussi portée il porte aussi le sujet plus globale de famille et qui sont comme lui dans des impasses. Aujourd'hui, l'école inclusive ces 430.000 enfants inclus dans l'école de la République. Mais les IME s'est mis le 140ème sur notre territoire national pour 71.000 places. Les places à l'IME n'ont jamais été supprimée n'ont jamais été diminué et ont toujours continuer à évoluer. Il faut savoir que sur ces 71.000 places nié me. Il y a de façon anormale 10.000 places occupées par des adultes. Sous-amendement Creton qui restent dans 16ème. Notre première mission doit être avec les départements, chaque département de travailler efficacement et concrètement à faire en sorte de trouver des solutions différentes pour ces adultes afin de redonner de la capacité à 16ème de pouvoir accueillir des enfants car la place des enfants, c'est dans des établissements pour enfants. Deuxièmement, il y a des territoires dans notre pays qui sont en manque de solutions et ça nous les avons bien identifié. Il y a une vingtaine de départements, environ et nous allons travailler prioritairement à proposer des nouvelles solutions des nouvelles places ou solution dans ces départements et enfin il y a des handicaps particuliers et complexe, comme vous le disiez, qui nécessite aussi. De porter des solutions nouvelles. La conférence nationale du handicap a donné l'occasion au président de la République de s'engager sur 50 nouvelles 50.000 pardon pour la France entière et c'est dans ce contexte là que nous allons déployer ceux-là c'est un effort majeur de millions d'euros de plus sur nos Budgets et que nous déploierons sur les 5 prochaines années. Merci madame Flucher. Augmentons avec plus de souplesse. Les capacités d'écueils soit structure par structure ou. Ou même en, en, en permettant des des projets innovants parce que c'est vrai que ces enfants qui sont tellement vulnérables. Ils méritent une attention toute particulière de la nation. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques Lozach. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques en effet la Coupe du monde de football féminin va se dérouler du 20 juillet au 20 août prochain. Or à ce jour, aucun accord n'a été trouvé avec les diffuseurs éventuelle pour sa retransmission TV en France, l'appel d'offres concernés n'a toujours pas abouti. Cette réalité devient préoccupante appréciation confirmée par le président de la FIFA, organisatrice de l'événement, je cite, si les offres continue et ne pas être équitable, nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans les 5 grands pays européens. Je précise que les revenus ainsi générés sont redistribués intégralement pour le développement du sport féminin et que les chaînes françaises s'étaient engagées à davantage favoriser le sport féminin, l'enjeu la Coupe du monde 2023 est capital et la non-. Retransmission de match de notre équipe nationale. L'une des meilleures. Elle fait partie du top 5 mondial serait d'autant plus incompréhensible que la dernière édition fut organisée en France en 2019 et avait remporté un succès dépassant toutes les prévisions. Ainsi le match de quart de finale, avait-il que avait-il connu le score d'audience le plus élevé de toute l'année 2019 pour TF1 et 4 ans plus tard, cette équipe serait laissé à l'abandon par tous les diffuseurs potentiels. Avec la loi du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport. Le Parlement a voté la possibilité de créer une société commerciale visant à gérer plus efficacement des droits audiovisuels du sport professionnel. Pour l'heure seul le football est. Il serait Il serait paradoxal que, parallèlement à cette démarche. La dimension féminine de cette activité exclu des bénéfices financiers escomptés lors d'un grand événement international. Il y va symboliquement de la promotion de l'affirmation et du financement du sport féminin, l'enjeu et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Les obstacles à l'émancipation de la femme par le sport pouvez nous indiquer si à ce stade, il y a lieu de rester optimiste quant à ses retransmissions. En un mot, la France sera-t-elle. Privée de Coupe du monde féminine, enfin le décret de décembre 2004. Listant les 21 événements d'importance majeure doit-il être élargie à l'ensemble des matchs des équipes de France de football et de rugby masculine et féminine et si oui dans quel délai. Merci. Pour vous répondre. La parole est à monsieur. Olivier Véran Ministre délégué chargé du renouveau démocratique porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs sénatrice. Vous l'avez dit, en 2019 nous étions 12 millions de téléspectateurs pour encourager l'équipe de France féminine de football face au Brésil. 12 millions, ça crée beaucoup de vocations et on a besoin de montrer ces images de sportive de de haute compétition pour donner envie aussi à notre jeunesse de faire du sport, qu'elle soit féminine ou masculine. Il y aura dans 50 jours le début de la Coupe du monde féminine de football à nouveau c'est du côté je crois de l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour ne pas dire de de bêtises et nous voulons évidemment que les Françaises et Français puisse regarder la France, nous l'espérons en finale le 20 août prochain de cette Coupe du monde. À l'initiative de la France mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne de l'Angleterre, autant de pays européens. Passionné de football, comme chacun sait, la ministre des Sports dont j'excuse l'absence parce qu'elle est actuellement, donc pour un événement D. J moins 100 de la Coupe du monde de rugby cette fois-ci, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a rédigé un communiqué commun avec ses homologues européens à destination de la FIFA des annonceurs pour dire sa volonté qu'un accord puisse être trouvé de manière à ce que la Coupe du monde féminine de football puissent bien être diffusés dans notre pays, ainsi que dans l'ensemble des pays européens. Passionné de football. Elle l'a dit ce matin qu'une solution sera trouvée pour se faire par ailleurs, monsieur le sénateur. J'insiste avec vous sur la nécessité de diffuser du sport féminin aujourd'hui c'est que 5% du sport diffusé sur la télévision qui concerne le sport féminin. Or le sport féminin est un sport de qualité d'excellence et qui fait rêver. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. La parole est maintenant madame Florence Lasserre arabe pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les fermetures temporaires, des services d'urgences et de maternité se multiplient en raison des difficultés de recrutement médical ainsi en l'espace d'un mois, le service des urgences du centre hospitalier de Sainte-Foy la Grande a été fermé à quatre reprises, ce qui correspond à une durée de 17 jours au total, les services d'urgence d'Arcachon et la maternité de Langon ne sont pas plus épargné ces fermetures temporaires ne se limite pas au département de la Gironde et touche l'ensemble du territoire. Ces arrêts sont beaucoup plus prégnant sur les territoires ruraux. En cause, le manque de Mersin, de médecins accrue par la mise en oeuvre de la loi risque qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires. Or on constate déjà 14.000 décès supplémentaires par an dans les zones rurales par rapport aux villes par ailleurs de 2012 à 2019, on observe une augmentation de 7% de la mortalité infantile ainsi en l'espace d'une décennie. La France est passée du 2ème au 25ème rang européen. Cette dégradation alarmante de notre système de santé est inacceptable. Votre gouvernement culpabilise les médecins en laissant penser qu'ils sont responsables de la situation. Ce matin j'ai appris que la chef de service d'une de ces structures. En poste depuis de depuis de depuis plus de 30 ans vient de faire une tentative de suicide. Ce que vivent les médecins est inhumain. Ils ne sont pas là pour pallier les insuffisances du système, c'est votre responsabilité, nous connaissons des difficultés de recrutement et de fidélisation des praticiens hospitaliers en raison d'un manque d'attractivité. Le constat est sans appel. Aujourd'hui 30% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants. C'est du jamais vu. Monsieur le ministre, il faut remettre de l'attractivité pour la médecine hospitalière. Nous avons le devoir collectif de renverser cette situation. Quelles solutions pérennes proposez-vous pour pallier les difficultés de recrutement médical et éviter la multiplication des fermetures temporaires de services d'urgence et des maternités. Merci. Si pour vous répondre. La parole est à monsieur François Braun Ministre de la Santé et de la prévention. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice la. Effectivement, les difficultés de notre système de santé sont à qu'et dans les services avec plus forte pénibilité, en particulier la pénibilité des gardes de nuit. Donc vous faites bien de de signifier les services d'urgence et les maternités de maternité cumulant en plus la difficulté d'avoir 3 spécialités pour pouvoir assurer un fonctionnement en maternité et les gynécos obstétriciens, anesthésistes réanimateurs et pédiatre. Ces difficultés sont sont connus ces difficultés ne sont pas nouvelles et je ne peux pas vous laisser dire que l'intérim en tout cas la la justifier, lutte contre les dérives de l'intérim médical qui était en train d'assécher complètement nos hôpitaux soit responsable de la situation actuelle, nous avons au contraire passer ces difficultés pendant le, le mois d'avril et le mois de mai et maintenant nous avons la visibilité de ce qui se passe réellement sur notre territoire comme je m'y étais engagé, nous trouvons des solutions certes alternative sur l'ensemble des territoires pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans le cadre des parcours de soins. Je vous rejoins lorsque vous dites que ces difficultés ne sont pas nouvelles et sont anciennes, elles sont en particulier, dû à des difficultés du nombre de personnel médical je ne rappellerai pas. Le numerus clausus parce que fort heureusement le gouvernement précédent a levé cette barrière du numerus clausus qui quoi qu'on en dise nous permet aujourd'hui d'avoir 15% de médecins en plus qui vont sortir de nos facultés dans quelques années la solution elle est globalement sur 3 principes un principe d'éthique, c'est comme ça qu'on reconstruit notre système et c'est ça la lutte contre les dérives de l'intérim et d'autres luttes financière un principe d'équipe à l'échelle de l'équipe de chaque service que l'on peut reconstruire et un principe de. Territoire la responsabilité territoriale a été mis en place au niveau des hôpitaux, pendant ces travaux contre les dérives de l'intérim. Elle a fonctionné, elle fonctionne encore pour assurer la meilleure réponse à nos concitoyens et je profite des dernières secondes pour préciser qu'en ce qui concerne l'aide médicale urgente, c'est-à-dire les urgences vitales qui est un sujet que je connais bien, celle-ci reste garanties sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Merci madame la Sarah. 10 secondes. Monsieur le Ministre, vous ne répondez pas à ma question. Le président de la République promet aux Français le désengorgement des urgences d'ici fin 2024. Mais tant que les personnels soignants ne sont pas rémunérés à hauteur de leur engagement de responsabilité le désengorgement des urgences restera une belle promesse. Merci. La par les maintenant madame Lana Teto Annie pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président Madame. La Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question sera. Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Monsieur le ministe. Depuis quelques mois je suis continuellement interpellé par nos compatriotes polynésiens sur les délais d'obtention d'un passeport. Dans un territoire comme le mien. Ainsi, pour tous ceux situés hors zone européenne détenir un passeport à jour est une condition essentielle pour se déplacer. Mais l'obtenir relève aujourd'hui du parcours du combattant. Nous on est sait les difficultés rencontrées évoqué à l'échelon national. Mais pour nos citoyens ultramarins située si loin du centre dédié à l'élaboration des passeports. Ma question est la suivante. Quelles mesure combien d'aller-t-il d'adopter d'adapter pour des délais plus raisonnables dans l'obtention et l'acheminement de passeport en outre-mer. Merci. Pour vous répondre. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales de la ruralité. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Lana. Tetuanui. Je vous demande de bien vouloir excuser Monsieur le Ministre de l'intérieur des outre-mer qui d'ailleurs étant d'outre-mer pour vous dire et vous le savez que le les délais de délivrance des passeports et des cartes d'identité a augmenté énormément avec l'augmentation du nombre de demandes, on est passé de 9 millions en 2021 à 12 millions en 2022 à 15 millions actuellement. Donc nous mettons des moyens très importants, nous avons encore renforcer ses moyens pour raccourcir ces délais, à la demande de madame, la Première ministre il y a exactement un mois. Mais. Les délais en Polynésie sont particulièrement. Satisfaisants, ils sont.

à 50 jours, on est à 70 jours, il y a 2 mois. Donc les délais moyens baissent mais les délais en Polynésie. Vous avez 18 dispositifs de recueil et on est en train d'en mettre un 19ème donc que les délais soient trop longs et même un mois vous vous trouviez que ce soit trop long, je suis d'accord avec vous, nous y travaillons, nous portons l'objectif de les baisser très significativement d'ici l'été. je vous demande d'entendre que. Ben les collectivités locales et, et le préfet en Polynésie fait un travail remarquable qui fait que le délai est très bas. Merci. Madame. Je suis sûr que vous allez dire votre ravissement allez-y Madame la fenêtre. Madame la ministre, je vous remercie. Mais je vais être gentille aujourd'hui je vous pardonnerez je vous excuserez mais par la méconnaissance mais. De ce qui se passe dans nos collectivités. Ultramarines. Si je m'exprime aujourd'hui c'est parce que il y a un problème. Si tout allait bien. Je me tairai mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Parce que là où je vous interpelle aujourd'hui à l'approche des grandes vacances scolaires, pour tous ceux et toutes celles qui veulent rentrer dans nos cours l'activité. Il y aura la rentrée universitaire au mois de septembre. Pour tous nos étudiants qui vient de Rouen poursuivent les études ici. En France en fait quoi. On dit plus métropole Andy hexagone aujourd'hui d'après l'Assemblée nationale. Mais on fait quoi. Les services de l'État, les services du commissaire précisément en Polynésie française, quand les arbres. Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils disent à la sénatrice PS cuisine excusez nous madame Martine actrice. Il y a trop de, de monde on n'y peut rien, ils font attendre, mais c'est à environ d'entendre ça en 2023.

je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h 30 pour le débat sur le bilan de l'application des lois, la séance est suspendue.

La séance est reprise. La parole est d'abord à Madame, Amel Gacquerre, pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci monsieur le président je souhaiterais rectifier en un vote lors du scrutin numéro de 192, de la séance du 30 mai 2023 sur l'ensemble du projet de loi visant, donner à la douane, les moyens de faire face aux nouvelles menaces Madame Doineau a été considérée comme ne prenant pas part au vote, alors qu'elles souhaitaient voter pour. Je vous remercie. Merci, cher collègue, acte et donner de votre mise au point, elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la CMP chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle le débat sur le bilan de l'application des lois. La parole est à madame Pascale Gruny. Président de la délégation du bureau en charge du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chaque disposition législative qui demeurent inappliquées est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens. Ce ne sont pas là les mots du Sénat mais de la Première ministre dans une circulaire du 27 décembre 2022 relatives à l'application des lois. Les mots sont forts et rappelle l'importance de notre débat d'aujourd'hui, mais qu'en est-il des actes. Le bilan que je vous présente aujourd'hui. Analyse la mise en application des lois adoptées lors de la session parlementaire 2021 2022, c'est-à-dire entre le premier octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Sur cette période 64 lois ont été adoptées. 18, loi été d'application directe et 46 loi nécessité un total de 649 mesures d'application. Par rapport à la session 2022 1021, le taux global d'application des lois s'améliore pour s'établir à 65% contre 57% l'année dernière. Par ailleurs, le délai moyen de prise des textes d'application diminue, passant de 6 mois et neuf jours l'année dernière à cinq mois et 20 jours, respectant ainsi la limite de six mois que s'est fixé le gouvernement, par une circulaire de février 2008, objectif réaffirmé dans la circulaire de décembre 2022. Enfin le taux de remises de rapports du gouvernement, Parlement progresse. Il est de 36% contre 21% l'année dernière. Mais le diable se niche dans les détails hein et ces amélioration globale cache des réalités très disparates. Certes le taux global d'application progresse mais il reste très variable selon les lois et selon l'origine du texte. Une loi emblématique de la session comme la loi 3DS n'avait ainsi un taux d'applications que de 52% au 31 mars 2023. Plus d'un an après sa promulgation. Et surtout les loi d'origine parlementaire ont bien. Un plus faible taux d'applications que les autres. Ce taux s'établit à 56% contre 65% toutes lois confondues. Cet écart de près de 10 points et d'autant plus frappant que les lois d'initiative parlementaire. Contiennent en général un nombre bien plus limité de mesures réglementaires. La loi, d'origine sénatoriale, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique dite loi Rennes hein du 15 novembre 2021 n'affichait au 31 mars 2023 quintaux d'application de 33%. Elle ne nécessiter pourtant que 6 mesures d'application. Je souhaiterais ici attirer tout particulièrement l'attention sur l'application des mesures ici d'amendements sénatoriaux. Le Sénat, soucieux de ne pas alimenter une inflation législative déjà chronique et pourvoyeur raisonner de nouvelles mesures réglementaires d'application par voie d'amendement par rapport au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Mais alors que le taux global de prise de textes d'application s'établit à 65%. Il chute à 57% pour les mesures issues d'un amendement sénatorial, contre une moyenne de 67% pour celle issue d'un amendement du gouvernement et de 70% pour celles issue d'un amendement de l'Assemblée nationale. Ce dernier chiffre peut en partie s'expliquer par l'existence d'amendements présentés par des députés, mais en réalité suggérée par le gouvernement. Cependant, une nouvelle fois, c'est bien la question du respect effectif de la volonté du législateur lorsque celui-ci siège au Palais du Luxembourg, qui se trouve posée. S'agissant de la remise des rapports du gouvernement au Parlement, si le taux global de rendu s'améliore. Aucun des 21 rapport demandé au détour d'un amendement d'origine sénatoriale n'a été transmis là encore cette déficience est d'autant plus dommageable que suivant une doctrine constante les commissions font pourtant preuve de parcimonie dans leur demande de rapport. La réserve du Sénat comme l'année dernière, continue à ne pas être récompensé. Je terminerai cette présentation générale en abordant la question de l'application des lois adoptées avec après engagement de la procédure accélérée. Le gouvernement recourt toujours massivement à cette procédure. Puisqu'elle s'est appliquée à 45 des 64 loi adoptée sur la session 2021 2022. Pourtant, et c'est un paradoxe, le délai moyen de prise des textes d'application n'en est pas pour autant plus rapide. Ce délai moyen s'établit à 6 mois et 8 jours contre un des les moyens toutes lois confondues de 5 mois et 20 jours même si l'écart n'est pas exorbitant, le constat s'impose donc d'une célérité imposer au Parlement à laquelle le gouvernement quant à lui ne s'astreint pas pleinement jusqu'à dépasser le délai de six mois prévu depuis 2008 et réaffirmé en 2022. S'agissant de la procédure accélérée. Je note au passage que la secrétaire générale du gouvernement dans son audition au Sénat de juillet 2022. Assuré que le gouvernement avait bien entendu les messages les plus récents sur le souhait notamment du président du Sénat, que cette procédure ne soit pas systématiquement solliciter elle indiquait qu'une procédure intermédiaire pourrait être imaginé une procédure certes accéléré mais tout en respectant les délais de 4 à 6 semaines prévues à l'article 42 de la Constitution, précisant qu'il s'agit d'une piste qui devra être regardée. Où en est-on aujourd'hui de cette réflexion et, que proposez-vous. Avant de revenir à des questions de fond sur l'application de certaines lois. J'aimerais, monsieur le Ministre aborder des questions de méthodologie comme vous le savez les méthodes retenues par vos services et celle retenue par le Sénat ne sont pas exactement les mêmes. Outre la prise en compte propre au Sénat des mesures différées nous recensons les arrêter et les décrets prévus pour l'application des lois. Vous ne retenez quant à vous, que les mesures appelant un décret d'application. Cette année, l'écart est particulièrement important, ce sont 68% pour notre taux hors mesures différé et 74% pour le vôtre. L'explication n'est que le taux de parution des arrêtés que les services du gouvernement, je le rappelle n'inclut pas dans leur bilan est particulièrement faible, à 42% contre 72% pour les décrets. Cette année encore, nous regrettons cette absence de suivi des arrêtés par le secrétariat général du gouvernement pour l'application d'une loi. Peu importe que la disposition adoptée renvoie à un décret ou un arrêté la non adoption de l'un ou de l'autre a pour effet dans les 2 cas d'empêcher la volonté du législateur de se traduire pleinement dans le droit. L'année dernière Madame Landais avait envisagé que le secrétariat général du gouvernement soit au moins le relais d'une demande de suivi un peu plus précis des arrêtés et sur des schémas plus harmonisée avec éventuellement des clauses de revoyure. Alors que le gouvernement a tenu par une circulaire actualisé a rappelé avec force à ses services, l'importance du suivi de l'application des lois. Où en est-on là aussi de ce projet. Monsieur le Ministre, je souhaite pour terminer vous poser quelques questions précises en ma qualité de membre de la commission des affaires sociales, ainsi que de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments. La première concerne l'application de l'article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Cet article a inscrit dans le code de la sécurité sociale, la possibilité de prise en compte de critères d'implantation des lieux de production sur le sol français pour la fixation du prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Au cours de la navette, le gouvernement avait fait valoir qu'un décret précisant les conditions d'application de cette disposition serait de nature à retarder sa mise en oeuvre. Toutefois faute de décret. Celle-ci a été soumise à l'élaboration d'une doctrine propres par le gouvernement et le comité économique des produits de santé, le CEBS, mais celle-ci a pris beaucoup de retard et a défini un Champ d'application plus restreint que ce que le législateur a voulu ma 2ème question concernait elle aussi les mesures de nature à lutter contre ce phénomène de pénurie de médicaments. L'article 61 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, a introduit dans le code de la santé publique. La notion de préparations hospitalières spécial mais le décret en Conseil d'État indispensables à son application n'a toujours pas été pris alors que ces préparations. Ces préparations constitue un moyen fort utile de lutte contre les pénuries de médicaments indispensables, comme ce fut le cas au plus fort de la pandémie. Enfin j'appelle par avance votre attention sur l'article 37 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Cet article prévoit d'ajouter une 4ème année au 3ème cycle en mai de général afin notamment que les internes puisse réaliser un stage de pratique ambulatoire en priorité dans les déserts médicaux, un sujet très attendu surtout n'était nos territoires. Ce faisant, il remplace une précédente disposition qui n'avait pas trouvé à s'appliquer faute de mesures d'application. Vous comprendrez donc que je ne souhaite pas que l'histoire se répète. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos réponses. Merci. Merci madame la présidente. La parole est maintenant monsieur Franck Riester Ministre chargé des relations avec le Parlement pour cinq minutes. Monsieur le président, madame le président de la délégation du bureau. Mesdames, et messieurs les présidents de commission mesdames et messieurs les sénateurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité du travail présenté par Madame le président Gruny et les contributions des commissions permanentes sur la base de nombreux échanges avec le secrétariat général du gouvernement dont je souhaite souligner l'engagement permanent pour piloter l'application des lois. La Première ministre a rappelé dans la circulaire du 27 décembre 2022. Les principes et les modalités de cet exercice en soulignant qu'il s'agissait d'une triple exigence de démocratie. De sécurité juridique et de responsabilité politique. L'adoption d'une nouvelle circulaire près de 15 ans après la précédente témoigne de la volonté du gouvernement d'assurer une application des lois qui soient tout à la fois rapide et conforme à l'intention du législateur. Au 31 mars 2023 hors mesures différer le taux d'application des lois, publié entre octobre 2021 et le 30 septembre 2022 était de 74%, soit une augmentation de 14 points par rapport à l'année dernière. Cet effort ne s'est pas relâchée 40 n'en compte des derniers textes adoptés depuis fin mars, ce taux atteint désormais 78%. J'ajoute que pour l'ensemble des lois adoptées au cours de la XVe législature, le taux d'application et de 92%. Comme vous l'avez indiqué madame le président ce taux d'un n'inclut pas les arrêtés qui relèvent d'une compétence ministérielle et qui sont en vérité trop nombreux pour faire l'objet d'un suivi centralisé. Le secrétariat général du gouvernement appelle toutefois régulièrement l'attention des ministères sur ce point et je prends l'engagement d'évoquer cette question lors du prochain comité interministériel sur l'application des lois. En outre, près de deux tiers des décrets d'application ont été pris dans le délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi, conformément à l'objectif rappelé par la circulaire de la Première ministre. On ne saurait toutefois se satisfaire totalement de ce résultat. Comme vous l'avez souligné dans votre rapport, l'application de certaines lois, y compris ancienne reste en deçà des attentes. Les ministères concernés Travail continuellement à minorer leurs taux d'application. La progression de la loi climat résilience d'août 2021 ans témoigne. De 12 131 mars 2022, le taux d'application de la loi s'élève désormais à 78%. Vous pointez par ailleurs à juste titre l'écart de 9 entre le taux d'application des lois d'origine gouvernementale et celui des lois d'initiative parlementaire. Il ne faut toutefois pas y voir le signe d'une mauvaise volonté de la part du gouvernement mais principalement la conséquence d'une moindre anticipation des textes d'application des lois d'origine parlementaire. Lors du dernier comité interministériel sur l'application des lois. J'ai demandé au directeur de cabinet de tous les ministres de réduire cet écart car cela est tout à fait essentiel au respect de l'initiative parlementaire. Quant à la remise des rapports, les taux de transmission par progresser. Ainsi 71% des rapports d'application des lois ont été remis à ce jour. Il est certainement possible de progresser encore sur ce point. Quant aux autres rapports ponctuels demander le taux de remise et de 43%. Madame le président. Je partage votre mécontentement sur l'absence de remise des rapports demandés par le Sénat et m'engage dès demain matin à écrire au ministre concerné. Enfin, s'agissant du recours aux ordonnances auquel le Sénat prête la plus grande attention. Celui-ci s'est considérablement réduit sur la période récente. Ainsi, alors que 353 ordonnance avait été prise au cours de la XVe législature, seulement 23 ont été publiés depuis le début de cette législature et 34 habilitations ont été demandés par le gouvernement. Enfin pour vous apporter des précisions sur certains points Madame le président Madame, le président concernant la procédure accélérée, son engagement sur les projets de loi est une tendance de long terme qui vise surtout à permettre la convocation d'une CMP dès la fin de la première lecture. Dans la pratique, son impact sur les délais prévus à l'article 45 de la Constitution et modéré et le gouvernement s'efforce de le limiter au mieux. S'agissant des dispositions relatives aux médicaments. Le décret sur les préparations hospitalières spéciale est en cours de concertation en vue d'une publication au second semestre 2023. Quant au comité économique des produits de santé il prend bien en compte la localisation de la production dans la fixation du prix en vue de sécuriser l'approvisionnement selon l'amélioration du service médical rendu. Voici les éléments dont je souhaitais vous faire part en introduction de ce débat et je vous en remercie. Merci, monsieur le Ministre, nous allons maintenant procéder au débat interactif, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, maximum, y compris d'éventuelles réplique le gouvernement dispose d'une durée et. Yves allant dans ce débat. La parole est d'abord aux représentants des commissions à commencer par Madame. Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. au regard de l'actualité, si vous me permettez je vais consacrer mon propos au secteur de l'énergie. La loi du 24 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ces ces faits atteint 20 mois après sa promulgation, un taux d'application de 58% qui apparaît assez modeste au regard des ambitions affichées par le gouvernement de nombreuses dispositions sont encore manquantes dans les domaines du logement, comme par exemple la définition des classes de logement de l'agriculture, comme par exemple l'expérimentation du menu végétarien. Dans le domaine de la forêt comme par exemple l'adaptation de la gestion forestière et la prévention du risque incendie ou de l'énergie avec l'utilisation de Mathiot bio de matériaux pardon biosourcés tandis que la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie est une priorité partagée sur ces bancs d'où provient ce retard heureusement Monsieur le Ministre, que nous avons légiférer dans l'urgence les débats en matière de politique énergétique révèle l'absence de vision à long terme et en revanche la nécessité d'une véritable programmation. C'est la raison pour laquelle la loi Énergie Climat modifié par la loi climat résilience a prévu qu'une loi quinquennale détermine les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale. C'est un point majeur du compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, cette loi devait être prise avant le 1er juillet prochain et prévaloir sur tous les documents programmatiques réglementaire dont la TPE et la stratégie nationale bas-carbone. C'est une obligation légale inscrite au Code de l'énergie. Certes, la Première ministre a annoncé une loi sur le sujet. Toutefois celle cette loi sera présenté après la présentation de la PPE et la stratégie nationale bas-carbone bas-carbone. Ce qui est contraire aux objectifs à la volonté du législateur. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions sur la loi énergétique. Monsieur le Ministre. Et mobilisé pour la mise en oeuvre de cette loi énergie-climat, je vous rappelle d'ailleurs dans les échanges que nous avons eu. Ensemble que les projets de loi. ENR et nucléaires ont été adoptés prioritairement pour se caler dans la. Trajectoire énergétique actuelle. Mais pour autant, la volonté d'avoir une vision ensuite global et c'est donc. Une confirmation que je dois vous faire aujourd'hui c'est que un projet de loi de programmation énergie climat. Sera bien présenté à l'Automne comme l'a indiqué la Première ministre le 26 avril dernier lors de la présentation de la feuille de route du gouvernement cette loi doit remettre notre pays sur la bonne trajectoire énergétique en s'appuyant sur les textes précédemment voté un grand chantier de concertation a été lancée le 23 mai par la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avec les parlementaires avec les élus locaux, les professionnels des secteurs concernés avec les partenaires sociaux et la société civile. Il doit aboutir à la fin du mois de juillet. Ce chantier est structuré autour de groupes de travail piloté par des élus et rassemblant les différentes parties prenantes autour de plusieurs thèmes de travail sur les objectifs de la programmation sur les moyens pour les atteindre et la déclinaison déclinaison territoriale et opérationnel de cette stratégie. L'ambition du gouvernement et de proposer une loi de programmation qui soient. Concrète et la plus consensuelle possible vu l'importance du sujet. Ce qui implique d'associer les différents acteurs à son élaboration. La mise en oeuvre des choix énergétiques exige en effet de la stabilité et donc du consensus sur les orientations retenues. La programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone seront adoptées par décret dans l'année suivant l'adoption de la loi de programmation afin que ces 2 documents soient bien définies sur la base des objectifs fixés par le Parlement. Merci la parole est maintenant monsieur Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Merci président, Monsieur le Ministre. En ce qui concerne notre commission le bilan de l'application des lois est plutôt positif, car l'essentiel des lois d'ONU-Sida suivant l'application est désormais totalement applicable néanmoins néanmoins. Si l'ensemble des décrets prévu par la loi. Relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ont bien été pris la mise en oeuvre de l'un de ces décrets pose un véritable problème. Il s'agit du décret 787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Plus de 20 mois, 20 mois après la promulgation de cette loi et malgré la publication du décret. Cette commission qui doit être composée d'un collège de parlementaires et d'un collège de personnalités qualifiées n'a toujours pas été mise en place, c'est un sujet que notre commission suit attentivement. Il s'agit quand même d'une modeste enveloppe de 13 milliards et les co-rapporteurs ont même écrit. à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a de cela de mois pour lui demander quelles sont les perspectives de la mise en place de cette commission et quelles sont les circonstances qui la bloque encore aucun, aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour, vous allez sûrement me donner des précisions, je vous remercie. C'est sûr. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le Président. Bon vous m'interrogez sur le retard pris pour la mise en place de la commission de l'aide publique au développement. Il s'explique par un sujet de gouvernance concernant la présidence comme vous le savez de la commission. La loi du 4 août 2021 a en effet placé la commission d'évaluation de l'aide publique au développement auprès de la Cour des comptes afin qu'elle bénéficie de l'indépendance et de l'expertise de la cour en matière d'évaluation des politiques publiques. Elle n'a toutefois pas prévu la présidence de la commission par son 1er président comme il est pourtant d'usage pour les autres institutions adossée à la juridiction financière comme le Conseil des prélèvements obligatoires. Si un décret a bien été pris le 6 mai 2022 sur les modalités de fonctionnement de la commission. La question de sa présidence a fait l'objet de nouvelles discussions lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, comme vous le savez, le gouvernement ayant proposé de préciser ce point par un amendement adopté par le Sénat. Cette disposition n'a toutefois pas été conservé par l'Assemblée nationale dans le texte promulgué. Après cette nouvelle période de discussion au Parlement et après concertation et la Cour des comptes. Les travaux ont pu reprendre au printemps sur la base de la gouvernance initialement prévue. Les 8 personnalités qualifiées ont été identifiés seront prochainement désignés par un décret de la Première ministre. Par ailleurs, de députés, de sénateurs devront être désignés pour composer le collège des parlementaires. Je peux également vous indiquer que la Cour des comptes a déjà lancé des travaux de préfiguration pour permettre une mise en place de cette instance dès l'ensemble des nominations effectuées. président Cambon. Je. Merci de ce rappel. Je souhaite effectivement que cette commission soit mise en place très rapidement, comme je l'ai indiqué, il s'agit d'un véritable contrôle parlementaire. Délégation modeste de sénateurs de députés doivent participer à cette commission, mais c'est quand même essentiel. Commission d'évaluation, 13 milliards de crédits chaque année. Je compte sur la diligence du gouvernement pour pour que les différentes consultations entre la Cour des comptes. Le Parlement, l'Assemblée nationale, Sénat bien sûr mais de ce dispositif en route. Je pense que ce sera. Au bénéfice d'un meilleur contrôle parlementaire. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Madame Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Lors de ma communication. Sur l'application des lois. J'ai indiqué que les 9 loi examiné par la commission des affaires sociales. Un total de 191 mesures réglementaires d'application. Alors, 116 mesures ont été prises au 31 mars. Soit un taux de 61%. Mais je focaliserait mon propos sur le retard d'application dont souffrent la loi du 7 février 2022 relatives à la protection des enfants puisque la semaine passée, nous avons entendu la secrétaire d'État Charlotte Caubel sur ce sujet en effet seulement 37% des mesures réglementaires attendus ont été prises. nous entendons les raisons avancées, l'ampleur des mesures à prendre. L'entrée en vigueur de la loi en toute fin de législature et les délais de consultation des différentes instances et la secrétaire d'État pointé les défaillances de l'étude d'impact de cette loi mais au Sénat nous ne refus trompe pas en effet que les études d'impact des projets de loi peuvent être tout à fait elliptique. Toutefois, ces raisons ne justifient pas certaines situations absurdes je pense un décret encadrant l'hébergement hôtelier des enfants protégés pendant le délai transitoire avant une interruption complète et le décret intervient alors que la période transitoire, il a déjà écoulé aux 2 tiers en commission, nous avons noté que le taux d'application de la loi devrait être porté à 75% disent si l'été puisque. 9 sur les 15 mesures encore attendues sont bien avancées, mais pour vous ne pouvez-vous nous dire ce qu'il en ait des six dispositions restantes pour lesquels il n'est pas prévu de décrets à court terme. Monsieur le ministre. énoncé la secrétaire d'État chargé de l'enfance, madame Charlotte Caubel s'est engagé devant votre commission la semaine dernière a publié 75% des décrets d'application. Au mois de juin. Le délai de publication des textes s'explique notamment par le chant décentralisé de cette politique qui implique un temps de concertation technique avec les services départementaux, les acteurs associatifs et un temps de concertation, comme vous le savez. Politique avec l'association des départements de France. Par ailleurs, ces textes nécessite la consultation obligatoire de plusieurs instances comme le Conseil national d'évaluation des normes et le Conseil national de la protection de l'enfance. Concernant l'ordonnance dont le délai d'habilitation a expiré. Celle-ci portait sur l'extension et adaptation de certaines dispositions de la loi en mer. Après réexamen de par les services cette habilitation n'a finalement pas été mise en oeuvre. Cette situation ne soulève toutefois pas de difficultés de fond car il n'y a pas de problématique particulièrement signalé en matière de hein dans les territoires concernés. Au-delà de ces cas d'espèce, je ne peux toutefois que regretter avec vous que des demandes d'habilitation ne soit pas utilisé dans le délai imparti. Enfin je peux vous indiquer que le sujet du rapport demandé sur l'inscription à l'assurance maladie de certains actes effectués par les infirmières puéricultrices dans les services de la PMI fera l'objet de discussions lors des Assises de la pédiatrie pour identifier les suites données à cette question. Merci madame la présidente de Roche. Monsieur le Ministre, sur les rapports. Nous on a une jurisprudence très clair, nous ne demandons jamais parce qu'ils ne sont jamais rendues donc c'est déjà on simplifie la tâche du gouvernement. Ils sont très exceptionnellement rendu. On a une mission d'information que l'on a créé de suivi de l'application des lois sur la protection de l'enfance à Bernard Bonne donc on on a eu cette audition très bien avec le ministre mais on, on suivra aussi ce dossier de façon très proche. Merci madame. Présidente. La parole est maintenant Madame Marta de Cidrac vice-, présidente de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il me revient d'intervenir cet après-midi au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dans le bilan d'application des lois que nous avons dressé au début du mois de mai, nous avons déploré le taux d'application trop faible de certains textes. C'est notamment le cas de la loi du 15 novembre 2021, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dit Warren issus des travaux menés pour notre commission par Patrick Chaize Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte fin mars après près de 18 mois après les promus la promulgation du texte seulement de mesures sur les 6 prévus avaient été prises par le gouvernement de décrets doivent notamment préciser les modalités de mise en oeuvre de l'éco-conditionnalité de l'Avantage fiscal attribué au centres de données en matière d'électricité alors que la France fait face à une crise énergétique et une crise d'eau sans précédent qui vont s'aggraver dans les années à venir en raison du réchauffement climatique. Aucun secteur ne peut être exonérée des efforts à mener pour la préservation de nos ressources énergétiques et naturelles. Nous appelons donc à la publication rapide de ces décrets qui inciteront les centres de données à rationnel il et leur consommation d'énergie et d'eau. J'en viens mon second point qui concerne l'application encore incomplète de la loi d'orientation des mobilités qui a pourtant été publié il y a plus de trois ans pour ne donner qu'un exemple. Le cadre réglementaire de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport public urbain par autobus de la RATP demeure inachevé. L'un des décrets prévu au terme de l'article 158 de la loi est relatif à la portabilité de certains droits des salariés en cas de changement d'employeur est encore attendu alors que nous approchons un grand pas de l'échéance de l'ouverture à la concurrence fixée au 1er janvier 2025 la finalisation de son cadre réglementaire doit constituer une priorité tant pour le bon déroulement du processus que pour donner de la visibilité aux salariés. Quant aux conditions qui s'appliqueront en cas de changement d'employeur, comme vous pouvez le constater. Monsieur le Ministre, nous sommes toujours dans l'attente, mais peut être nous rassurez-vous par votre réponse je vous remercie. Monsieur le Ministre. Vous ne voulez pas. Rassurée madame de Cidrac. Pardon, monsieur le président, madame la sénatrice. Concernant l'ouverture de la concurrence du réseau de bus de la RATP. L'article 158 de la loi d'orientation des mobilités est venu préciser le cadre social applicable à cette ouverture à la concurrence afin de protéger les salariés transférés de garantir la continuité du service public. Le cadre social de l'ouverture à la concurrence pour le réseau de bus de la RATP repose sur 4 décrets dont un reste à prendre, ainsi que sur deux arrêtés d'application de ces décrets. Le décret relatif à la portabilité du régime spécial de la retraite de la RATP a fait l'objet de première réunion technique en fin d'année 2022. Entre la RATP la caisse de retraite des personnels de la RATP et les services ministériels. Compte tenu de la réforme des retraites. Les travaux reprendront après la publication des décrets mettant en oeuvre la réforme pour les régimes spéciaux. Ensuite, je tiens à vous informer que la l'homme et la la mise en application de la l'homme et de 95%. S'agissant de la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, du 15 novembre 2021. Il s'agit de fixer par décret les modalités de mise en oeuvre de l'écho qu'on danse conditionnalité de l'Avantage fiscal attribué au centre de données en matière d'électricité spécifiquement comme vous l'évoquiez les indicateurs chiffrés que doivent respecter les sans donner de données dans leur consommation. Les travaux interministériels sont en cours et une première version du décret a été élaboré toutefois une analyse de la base légale est actuellement menée pour éviter un risque de contentieux sur les indicateurs techniques envisagées au regard de la doctrine fiscale. L'élaboration des mesures d'application pourra se poursuivre. Une fois ce sujet. Merci Merci la parole est maintenant à monsieur Claude Raynal, président de la commission des finances. Merci monsieur le président, madame la vice-président de monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour ce qui concerne la commission des finances. Nous constatons un taux de mise en application équivalent à celui de la session précédente donc sans progrès mais non plus sans détérioration avec toutefois un point positif. Davantage de mesures ont été publiés avant le délai de 6 mois. Mais certaines dispositions ne sont pas mises en oeuvre. Je voudrais dire donc vous interroger, Monsieur le Ministre, les 3 points suivants. L'article 9 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022. Prévoyez des mesures devant s'appliquer aux aéronefs et aérodromes concernant les tarifs d'assises sur l'électricité. Les recettes provenant de la taxe sur le transport aérien ou la taxe sur les nuisances sonores aériennes ces mesures appelé cinq arrêtés d'application. Pourquoi ces arrêtés n'ont-ils pas été pris alors même que le Parlement a été invité à les adopter en session extraordinaire. Le seront-ils. Et quand. 2ème. Sujet, l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 a introduit un nouvel article 14 18. Au sein du code général des impôts relatif pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe annuelle sur les logements vacants aux obligations déclaratives des propriétaires de locaux d'habitation. Selon des modalités fixées par décret. Avant même la parution du décret, administration fiscale, a lancé l'ouverture de la procédure de déclaration en ligne dès le 23 janvier 2023, celle-ci devant être accomplies avant le 30 juin. Pouvez-vous nous confirmer que le décret d'application a finalement été pris courant avril est-il pas étrange publier ce décret après avoir mis en place la procédure. Enfin les articles 130 131 134 de la loi du 22 mai 2019 relatives à la croissance et à la transformation des entreprises je loi pacte. Prévoyez des textes réglementaires doivent en tirer les conséquences de la privatisation d'aéroports de Paris. Au regard du fait que la privatisation d'ADP semble repoussé à une date indéterminée ne vous a repéré-t-il pas pertinent d'abroger se mesure qui n'ont plus vocation à à s'appliquer. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le Président rénale. La loi de finances rectificative 2022 comprend en effet plusieurs dispositions relatives aux aéronefs et aérodromes qui appelle des mesures d'application pour le tarif réduit d'accises sur l'électricité, pour la fourniture d'électricité aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes. Une demande de dérogation de la directive 2003 96 CE a été adressée en avril 2022 à la Commission européenne. Celle-ci a demandé des compléments d'information qui lui ont été adressées au cours de l'été, la demande est en cours de traitement par la commission. Pour les règles applicables aux exploitants d'aérodromes en terme de leur gestion. Un arrêté a été pris le 27 décembre 2022. Concernant les déclarations de coût des exploitants d'aérodromes. S'agissant du solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes à rembourser les arrêtés sont en cours de rédaction. Enfin pour l'exonération de tarifs de l'aviation civile de la taxe sur les transports aériens de passagers pour les vols au départ de l'aéroport de Bâle-, Mulhouse, un projet d'arrêté a été soumis à consultation le 24 mai dernier. Il sera très prochainement publier pour une entrée en vigueur. Du nouveau tarif le 1er juillet. En ce qui concerne l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 portant suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'administration a en effet ouvert dès le 23 janvier 2023. La procédure de déclaration en ligne avant la publication du décret, appelé par l'article 14 18 du code des impôts. Compte tenu du niveau de précision de la loi et dans un souci de célérité concernant cette mesure très attendue. La publication du décret, le 30 avril 2023. Par ailleurs, avant la date limite de l'obligation déclarative fixé le 30 juin 2023 et sans incidence sur la légalité du service de déclaration en ligne. Enfin concernant les dispositions de la loi pacte du 22 mai 2019 relatives à la privatisation d'ADP, les conditions de marché de sont plus réunies pour envisager la privatisation du groupe ADP. Compte tenu des incertitudes qui entourent la reprise du trafic aérien, il est aujourd'hui impossible d'établir un calendrier prévisionnel pour une éventuelle cession qui est reporté mais pas abandonner. Dans ces conditions l'abrogation des mesures de la loi pacte dont l'entrée en vigueur est conditionné à cette privatisation n'est pas requis. Merci la parole est maintenant Madame, Catherine Di Folco vice-, présidente de la commission des lois. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, je souhaite évoquer 2 exemples précis qui illustrent pour les textes examinés par la commission des lois, les difficultés d'application qui peuvent naître. Malgré la prise effective de mesures par le pouvoir réglementaire. Le 1er concerne l'article 229 de la loi 3DS qui prévoit les conditions dans lesquelles les chambres régionales des comptes participe à l'évaluation des politiques publiques territoriales. le décret du 2 décembre 22 pris pour son application prévoit que la chambre régionale des comptes, peu de sa propre initiative procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. Or cette capacité d'auto-saisine me semble excédé très largement l'intention du législateur. L'analyse des travaux parlementaires montre ainsi que l'intention du législateur n'était pas de créer une faculté d'auto- saisine aux Chambres régionales des comptes, mais de créer une compétence nouvelle d'évaluation des politiques publiques territoriales à la saisine exclusive des collectivités territoriales en la matière le pouvoir réglementaire a donc outrepassé l'intention du législateur. Le ministre de la cohésion des territoires, a opposé une fin de non-recevoir la question écrite de notre collègue Françoise Gatel, rapporteur de ce texte tendant à ce que le décret soit modifié pour respecter le souhait du législateur. Alors restez-vous vous aussi dans le déni. Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement. Le second exemple, et l'article 3 de la loi relative aux lanceurs d'alerte pour lequel le pouvoir réglementaire n'a cette fois pas été au rendez-vous de l'ambition fixée par le législateur. Cet article prévoit un système de réception et de traitement unique au sein des groupes de société loin de traduire cette volonté de simplification. Le décret du 3 octobre 2022 instaure un système. Perdant-perdant ou c'est de manière assez inexplicable au lanceurs d'alerte lui-même de retirer son signalement pour le redéposez auprès de la filiale la plus appropriée pour le traité. La Commission européenne avait pourtant ouvert la porte à une véritable procédure commune afin d'allergie, d'alléger les charges administratives pesant sur les entreprises et de simplifier le système, le Parlement l'avait entendu et malheureusement, le gouvernement a préféré faire la sourde oreille. Comment expliquez-vous pareille situation. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la présidente Di Folco. L'article 229 de la loi 3DS prévoit en effet que les chambres régionales des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques locales, le décret pris pour l'application de cette disposition prévoit que la chambre régionale des comptes, peu de sa propre initiative procéder à l'évaluation d'une politique publique. Relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. La rédaction de la loi 3DS est une reprise à l'identique de l'article du code des juridictions financières relatifs à la Cour des comptes qui dispose qu'elle contribue à l'évaluation des politiques publiques sur le fondement de cette disposition législative de principe la Cour pour réaliser de sa propre initiative, une évaluation de politique publique. Par conséquent l'article de la loi 3DS permet dans les conditions prévues par voie réglementaire aux Chambres régionales des comptes de procéder de leur propre initiative à l'évaluation d'une politique publique sur son ressort territorial. Le gouvernement considère ainsi que le décret pris est conforme aux termes de la loi. S'agissant de l'article 3 de la loi du 21 mars 2022 sur la protection des lanceurs d'alerte. Le décret du 3 octobre 2 2022 pris pour son application distingue les phases de réception et de traitement des signalements. Si dans un groupe de sociétés. Le principe est celui d'un traitement au niveau de l'entité concernée par la violation. La réception des signalements peut en revanche être mutualisés et se faire au sein de n'importe laquelle des entités notamment la société mère ou encore être géré en externe par un tiers. Le décret pris épuise l'ensemble des opportunités offertes par la directive 2019 1937 dites lanceurs d'alerte qui ne permet pas en particulier. De prévoir une externalisation une mutualisation spécifique des procédures de traitement des signalements dans les groupes de société. Merci la parole est maintenant monsieur Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. je souhaite revenir sur une nouvelle fois sur le recours aux ordonnances pour transport pour transposer les directives européennes ou prendre des mesures d'application des règlements comme vous le savez, le règlement du Sénat de la commission des Affaires européennes d'une mission de veille afin d'identifier les sur-transpositions et de s'assurer que le gouvernement les justifie tant elles peuvent nuire à la compétitivité de l'économie française. Or, lorsque le gouvernement choisit de recourir aux ordonnances pour transposer transposer les règles européennes en droit national. Ils révèlent rarement au Parlement ses intentions précises en particulier lorsque le texte européen comporte des options facultatives, ou lorsque l'habilitation qu'il demande au Parlement pour prendre l'ordonnance va au-delà des exigences de mise en conformité avec les textes européens. Un exemple récent permet de mesurer l'ampleur de la difficulté. La transposition de la directive dite CSR des sur les déclarations de performance extra-financière des entreprises. Le gouvernement a en effet sollicité une habilitation dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture dite Dadu. Or la directive n'avait pas encore été adopté, le délai d'habilitation sollicité était donc très long l'élaboration du projet d'ordonnance n'avait même pas été lancée, ce qui ne permettait pas au Parlement de se prononcer en ayant connaissance des orientations du gouvernement, ce dernier ne les avait d'ailleurs pas encore défini. Au surplus, le périmètre de l'habilitation était particulièrement large excédés sans conteste celui de la directive, comme vous le savez, le Sénat a rejeté cette demande d'habilitation dans un premier temps, avant finalement d'accepter en commission mixte paritaire, une version fortement resserré du Champ d'habilitation. Au vu de la directive adoptée dans l'intervalle, Monsieur le Ministre, le gouvernement peut-il nous assurer que pareille mésaventure ne se reproduira pas et qu'il intégrera dorénavant les mesures de transposition dans le projet de loi lui-même. Merci monsieur le le président. Monsieur le Président Rapin. En terme de vecteur le recours aux armes aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution représente de 7% des mesures de transposition de textes européens. Le gouvernement veille à y recourir pour des mesures de transposition essentiellement technique. La ligne retenue et de privilégier un projet de loi ou une proposition de loi dédié pour les directives les plus sensibles politiquement. Le recours aux habilitations est encadré par le secrétariat général du gouvernement et le SGA eux dans le cadre des réunions relatives aux travaux de transposition comme vous le savez et de préparation des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne femme têtue. J'ajoute que la nouvelle méthode voulue par la Première ministre prévoit un recours très modéré aux habilitations. Il est par ailleurs régulièrement demandé au service d'être en capacité de présenter au rapporteur les projets d'ordonnance envisagé lors de l'examen des demandes d'habilitation afin d'éclairer au mieux leur décision sur cette demande. C'est ce qui a été fait pour le dernier projet de loi Dadu notamment par la chancellerie. J'ajoute enfin que les efforts conjugués en faveur de l'adaptation rapide du droit national au texte européen permet à la France de présenter actuellement un déficit de transposition particulièrement faible de seulement 0 3 %. Je vous remercie. Merci la parole maintenant monsieur Laurent Lafon, président de la commission de la culture de l'éducation et de la communication. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. S'agissant de la commission de la culture de l'éducation et de la communication. Vous me permettrez dès à présent d'ajouter le sport à cet intitulé, le bilan de l'application des lois au 31 mars dernier et contrastée si l'applicabilité de certains textes s'avère satisfaisante. Je pense notamment à la loi de programmation de la recherche. Les mesures réglementaires attendus sur d'autres peinent manifestement à voir le jour. Il en va ainsi, Monsieur le Ministre de des décrets prévu par la loi créant la fonction de directeur d'école, le ministre de l'Éducation a récemment pris soin de préciser que. Leur publication avait été je cite retardé afin d'articuler leur disposition avec les nouvelles missions proposées aux professeurs des écoles dès la rentrée prochaine. Pouvez-vous donc nous confirmez Monsieur le Ministre que l'horizon de publication de ces mesures demeure bel et bien compatible avec la prochaine rentrée scolaire. Il en va de même pour les mesures réglementaires prévues par la loi pour une école de la confiance. Je souhaiterais à cet égard m'assurer en particulier de l'intention du gouvernement de publier le décret prévu à l'article 30 du texte et prévoyant notamment l'élaboration des conventions de coopération entre établissements médico-sociaux établissement scolaire pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. La prise en charge du handicap à l'école est un sujet sur lequel sur lequel pardon. La commission a beaucoup travaillé ces derniers mois et que cette mesure pourrait il compte contribuer à faire avancer significativement. S'agissant enfin de la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale des enfants sur les plateformes en ligne. L'absence de publication de la seule mesure réglementaire du texte rend malheureusement celle-ci inopérant. Alors que s'annonce l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Je souhaiterais savoir si la mise en oeuvre de cette loi est encore d'actualité ou définitivement abandonné. Merci monsieur le ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le Président la font. Concernant la loi que vous évoquez du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école de mesures ont été appliquées sur les 6 mesures attendues. Les textes récents à prendre sont en cours de finalisation. Ils ont été examinés au comité social d'administration du ministère de l'Éducation nationale du 16 mai et débattu en Conseil supérieur de l'éducation lors de sa séance du 17 mai. Le Conseil d'État devrait en être saisie dès cette semaine. S'agissant de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, elle présente actuellement un taux d'application de 90% avec 18 mesures appliquées sur un total de 20 mesures actives. La publication des décrets d'application manquant relatif au handicap va intervenir à la suite du conseil national du handicap, avant la fin donc de l'année 2023. Concernant la loi du 19 octobre 2020 encadrant l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, l'étude de l'Observatoire de la parentalité de l'éducation numérique publié fin février 2023 a permis de mieux appréhender les enjeux liés à cette exploitation et les besoin de régulation sur la base de ces résultats. Le décret sera pris très rapidement. Merci, monsieur le Ministre. Après la parole au président de Commission nous passons à la parole aux représentants des groupes et nous commençons par monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe RDSE. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous anime aujourd'hui est un incontournable de la vie parlementaire et de l'évaluation du Sénat mais il prend cette année une toute autre saveur, celle de la valeur de la loi, projets et propositions de loi, celle de la valeur du cheminement parlementaire réglementaire, celle de la valeur de la démocratie représentative de ses élus. Chers collègues, vous me permettez de saluer le travail réalisé par la présidente se passera le. Il dit beaucoup sur l'état de l'institution parlementaire et insiste clairement sur des leviers d'action qui chers collègues nous concerne également trop de lois en procédure accélérée trop vite des lois pantagruélique mal digéré des communications hein pressé les travers sont connues. Je salue un parallèle l'intention qui préside à la circulaire du 27 décembre 2022 pour qui veiller à une rapide et complète application des lois répond à une exigence de démocratie de sécurité juridique et de responsabilité politique. Toutefois, mes chers collègues comme l'énoncé si justement Pierre Manent France à la conception d'une démocratie purement formel et périodiques si je puis dire, ne correspond pas former ses mains à une réalité vivante. C'est bien celle-ci que je suis attaché, les conditions d'application de la loi font beaucoup pour notre vitalité démocratique tout d'abord, nous devons prendre conscience que n'essaie pas seulement le temps de publication des décrets qui pose problème. Mais bien que le concitoyen comme nos collectivités en besoin. Information conjugués. Est connu pour anticiper leur action. a l'Uruguay a insisté sur la loi climat et résilience, la loi 3DS et qui pour certains Antarctique un suspens sont des frais pour l'action locale c'est ce qui se place pour la qui piquait station Dusan par exemple 2ème point qui intéresse égal mais mes collègues députés, celui de l'encadrement plus strict des réseaux d'influence au moment de la rédaction. Ces steacks leur consultation peut être utile mais dans des conditions plus réglementé limitée dans le temps en toute transparence et sans préjudice pour la durée et la qualité de rédaction de textes réglementaires, mon dernier point, s'adresse à tous nos collègues au gouvernement. Mes chers collègues, nous pouvons anticiper dès le début de la discussion parlementaire quelques difficultés des textes la méthode le porte l'expérimentation et le porte-plusieurs cadres d'expérimentation nos mains. Local trop dilué dans les processus d'évaluation parlementaire la méthode répond pourtant un bel objectif celui de renouveler notre démocratie et de s'éloigner du populisme, celui de trouver des solutions acceptables. Je remercie Monsieur, Monsieur Merci monsieur le président, monsieur le sénateur Jean-Yves Roux vous évoquez tout d'abord les difficultés rencontrées par les destinataires de nouvelles normes pour les appliquer, prenant comme exemple les dispositions relatives aux Anne si je partage. Votre souci de stabilité de lisibilité du droit permettez-moi de souligner que sur ce sujet. La Première ministre a pris des engagements devant le congrès des maires et que le Ministre de la Transition écologique de l'aide des territoires Christophe Béchu a réagi dès l'été dernier face aux difficultés remonté par les collectivités territoriales en suspendant les textes d'application pour revoir le cadre applicable. Ce travail se poursuit au niveau législatif et réglementaire sur la base de la proposition de loi du Sénat qui sera examiné par l'Assemblée nationale le 21 juin prochain. Vous avez également évoqué je vous cite les réseaux d'influence lors de la rédaction des textes d'application. Sur le sénateur s'il est essentiel de prévenir tout conflit d'intérêt et a fortiori de sanctionner toute dérive en la matière. Les administrations des échanges réguliers avec les parties prenantes que soit chargée de réglementer, de contrôler et le cas échéance de sanctionner on reprocherait à bon droit aux administrations d'être déconnecté de la réalité. Quotidienne et du terrain. En l'absence de telles relations. Par ailleurs, préalablement à leur adoption. Les mesures réglementaires sont soumises de manière presque systématique à la consultation obligatoire d'organismes consultatifs. Quant au recours à l'expérimentation avant une éventuelle généralisation je souscris à vos propos sur l'intérêt de cette démarche dans laquelle le gouvernement s'est résolument engagé. Je suis très notamment à titre d'exemple, le droit de dérogation du préfet expérimentée en 2018 et 2019 sur la base du décret du 29 décembre 2017 puis généralisé en 2020 et qui a fait l'objet d'un bilan positif par les gains en 2022. On peut également mentionner le dispositif France expérimentation. Piloté par la direction interministériel de la transformation publique qui permet de lever les blocages juridiques entravant la réalisation de projets innovants grâce à la mise en place de dérogation à titre Enfin, j'ajouterais que la Première ministre a insisté, le 17 mai 2023 auprès des cadres dirigeants de l'État sur la pertinence d'expérimenter de prendre son risque et a invité chacun à se saisir de toutes ses capacités de dérogation et d'adaptation. Merci, je, je vois bien la passion dans ce débat mais si chacun pouvait rester dans les 2 minutes. Vous n'imaginez pas le ravissement que ce serait. La par les maintenant Monsieur André Reichardt pour les républicains. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, je souhaite intervenir au sujet de la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne dont j'ai été le rapporteur, cette loi illustre selon nous des dysfonctionnements dont on souhaiterait qu'il ne se reproduise plus. À l'avenir, j'explique, j'avais à l'époque critiqué la méthode employée, le texte était visiblement une fausse, proposition de loi ça existe. Rédigé par la direction centrale des ministères concernés, déposée par les députés, les députés du groupe majoritaire discuté au Parlement sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Le tout dans un domaine qui n'était pas sans compétence sans conséquence pour nos libertés publiques puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de retirer en une heure des contenus à caractère terroriste en ligne vous souvenez à l'époque de la loi du 24 juin 2020, dite loi Avia, qui avait été censuré. Le gouvernement souhaitait aller vite dans cette affaire là PPL. Adapter la législation française au regard du règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne compte tenu de ces enjeux. Le Sénat, nous avions accepté de jouer le jeu et d'adopter le texte en urgence pendant la session extraordinaire de juillet. Six juillet en commission 12 juillet en séance 19 juillet en commission mixte paritaire. 26 juillet, donc vraiment rapide. La loi a été promulguée le 16 août, après une décision de conformité du Conseil constitutionnel que s'est-il passé depuis rien rien faute de décret d'application. Cette loi n'est pas applicable dans l'attente de ce décret aucune disposition aucune injonction de retrait national n'a pu être émise par l'Office central de lutte contre la criminalité ton disque aucune injonction de retrait qui affronte transfrontalière venus d'une autorité européenne ne peut être traité. Finalement, après tout cela. Seule la nomination d'un suppléant de la personnalité qualifiée nommée au sein de l'Arcom est intervenue ce qui est un bilan bien maigre, vous en conviendrez monsieur le Ministre. Quand ce décret sera-t-il publié j'ajouterais franchement, peut-on éviter de tels dysfonctionnements à l'avenir merci. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, je vous évoquez l'application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, telle que modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne à laquelle vous aviez pris une part importante en tant que rapporteur. L'article. De la loi de 2001, 4 ainsi modifié prévoit un décret pour préciser les modalités d'échange d'informations dans le cadre des injonctions de retrait de contenus à caractère terroriste comme vous l'évoquiez entre d'une part l'autorité administrative et l'Arcom et d'autre part entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désigné pour la mise en oeuvre du règlement UE 2021 784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021. Le projet de décret a été présenté en section de l'intérieur du Conseil d'État le 16 mai 2023. Il est désormais en cours de signature et sa publication est prévue avant l'échéance du 7 juin 2023. Dans les jours qui viennent. Date à laquelle la France devra remettre un rapport de mise en oeuvre du règlement européen précités. Merci la parole maintenant monsieur Alain Marc pour le groupe les indépendants. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous ici une fois la loi votée le rôle du législateur n'est pas terminée. Comme chaque année à cette période, nous examinons le bilan de l'application des lois cet exercice traditionnel, c'est inscrit dans notre mission de contrôle de l'action du gouvernement en effet la bonne exécution des lois requiert une attention constante de notre part. J'aborderai trois problématiques spécifiques, la première se rapporte recours trop fréquent à la procédure accélérée. Si si elle aussi était inscrite dans la Constitution. Son utilisation répétée voor excessive porte atteinte au principe de la double lecture et oblige le Parlement à débattre dans des délais très restreint. Or la commission des lois constaté que parmi les 20 loi promulguée qu'elle avait été examiné au fond 17 avait été adopté après engagement de la procédure accélérée. Monsieur le Ministre, le recours à la procédure accélérée doit demeurer une exception. Quant à la 2ème problématique, elle concerne le respect délais pour la publication des rapports au Parlement sur l'a déjà été dit, le taux de publication global n'est que de 36%, ce chiffre n'est pas satisfaisant. Enfin la 3ème problématique porte sur l'inflation législative. Nous déplorons le fait que ce phénomène perdure. Si pour la commission des lois, le coefficient multiplicateur des dispositions législatives similaire à celui de l'année dernière. En revanche, nous constatons que le nombre d'articles comptabilisés au niveau du dépôt est en augmentation de 31%. Monsieur le Ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre afin de remédier à ces situations qui peuvent porter atteinte à la crédibilité de l'action publique. Tu. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le le sénateur à la main. Concernant le recours à la procédure accélérée que vous évoquez, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire son engagement était essentiellement motivé par la faculté qu'elle donne de convoquer une CMP dès la fin de la première lecture. Son impact reste modéré sur les délais d'examen fixées par l'article 45 de la Constitution et le gouvernement s'est efforcé de maîtriser. Depuis le début de la 16e législature à hauteur de 36 jours entre le dépôt DPJ elle et leur examen. pendant l'assemblée saisie en l'occurrence. Concernant la remise des rapports pour la session 2021, 2022 71 % des rapports d'application des lois et 43% des autres rapports ponctuels été remis. Sur l'ensemble de la XVe législature, le taux de remise et de 52% les ministères s'efforce de répondre au mieux à ces demandes et je sais que le Sénat partage la préoccupation de ne pas les multiplier, afin de ne pas saturer les services qui sont aussi chargés de concevoir et d'appliquer les politiques publiques. Concernant enfin l'inflation législative, je partage votre préoccupation. Le gouvernement s'est efforcé depuis le début de cette législature, de limiter le nombre d'articles des projet de loi présenté au Parlement, avec pour consigne lors des travaux interministériels de préparation de se concentrer sur des articles politiquement significatif et d'éviter toute empiètement sur le domaine réglementaire. Et si l'on s'en tient au sujet de l'application des lois. Je me permets de souligner que sans une estimation du FCG au cours de la XVe législature, le nombre de renvois des décrets d'application entre le projet de loi, déposée et la loi promulguée a été plus que multiplié par 2. On peut prendre comme exemple la loi 3DS par exemple dont le texte initial comprenait 38 renvoient à des décrets d'application contre 96 dans la loi promulguée ce qui a modifié sensiblement l'ampleur du travail d'application. Il s'agit donc d'une responsabilité partagée entre le gouvernement et le Parlement et qui appelle collectivement à une forme de sobriété normative. Monsieur Marc quelques secondes, non merci. La parole est maintenant monsieur Guy la roche pour le groupe écologiste. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, à ce moment du débat, effectivement c'est difficile d'être original, enfin j'je j'aurais du mal à l'être en tout cas donc pardonnez le manque d'originalité de mes questions. Je vais revenir sur 2 sujets le nord de passage en procédure accélérée. Bon je comprends bien vos raisons, vous en avez expliqué quelques-unes. Il est toujours aussi haut en fait la procédure accélérée n'est plus une procédure extraordinaire c'est la procédure normale. Et en fait c'est la procédure normale qui devient une procédure exceptionnelle. Il est doté d'ailleurs que ce ne sont pas les lois qui passe en procédure accélérée qui voient leur application arriver le plus rapidement. Or pour pourraient penser en toute l'eau logique en fait on passe par une loi procédure accélérée parce qu'il est urgent, c'est que donc on va avoir la même urgence à l'appliquer. Ce n'est pas du tout le cas puisque le la durée le taux enfin le le temps d'application d'une loi en procédure accélérée, est en fait plus lent en moyenne que le temps d'application d'une loi aux procédures normales. Ça baisse il à vous poser de question. Puisque ses textes en procédure accélérée de répondent pas une situation d'urgence. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'utilisez avec aussi peu de dissert de banc. À moins que ce soit pour. Restreindre le temps du débat au Sénat.

Malgré tout, j'ai entendu vos chiffre c'est pas ceux du SIDA il y a une augmentation du nombre de rapports que que tu es rendu par le gouvernement. Mais il me semble que il n'a que 36% de ceux qui de qui vous aurez été demandée par le Sénat qui aurait été reçus et qui ont été rendues publiques. Donc ma question c'est, est-ce que ces rapports de pas rendu et rendue publique parce qu'en fait vous avez pas le temps de les faire vous n'êtes pas pourvus suffisamment personnel que l'administration ne répond pas à vos demandes ou est-ce que c'est parce qu'en fait ils sont établis. Ses rapports avec vous ne souhaitez pas les Road'public. Monsieur le Ministre. Monsieur le président. Merci Monsieur le sénateur Bénin hanche qui certaines de vos observations rejoignent celles évoquées à l'instant avec le sénateur Marc et par le sénateur Mac. Concernant le recours à la procédure accélérée, j'ajouterai pour objectiver son impact sur les délais d'examen fixées par l'article 45 de la Constitution qu'en moyenne pour les projets de loi sur la période 2021 2023, 36 jours c'est par le dépôt du texte de son examen. Pour la première assemblée saisie 58 jours c'est pas la transmission du texte par la première assemblée et son examen par la seconde assemblée et 17 jours c'est pas la fin de la première lecture et la réunion de la CMP et je précise vraiment Monsieur le Sénateur, que ces données sont tirées à la baisse par la quinzaine de projets de loi liés à l'épidémie. De la Covid-19 dont le Parlement s'était saisi avec une très grande diligence et comme je l'ai évoqué tout à l'heure le le recours à des procédures accélérées permet de convoquer une CMP après les premières lectures, ce qui est évidemment fort utile concernant la remise des rapports. Outre les éléments que j'ai eu l'occasion d'apporter précédemment. Permettez-moi de préciser que l'absence de transmission pour les 21 21 demandes de, de rapports

et donc il y a pas de dissimulation de rapports. Parfois un certain de délai de de mise. À la concertation des projets de rapport de relecture et de validation est nécessaire, ce qui est aussi, explique le retard. Mais 21. Rapport non rendu cette problématique et je me dirigerai dès demain vers les ministres, pour leur faire savoir.

Dans une circulaire datée du 27 décembre 2022. La Première ministre Élisabeth Borne a réaffirmé la dimension capitale que représente l'application des lois dans notre pays, ainsi que les grands principes émanant cet impératif démocratique. C'est la première fois depuis 2008 qu'une telle impulsion est donnée par le gouvernement afin d'assurer que les textes votés par le Parlement et des effets concrets pour nos concitoyens dans les meilleurs délais et ce de manière conforme à l'intention du législateur. À cette occasion, la Première ministre a notamment demandé à renforcer le réseau des correspondants ministériel pour l'application des lois, ce réseau qui gagnerait à être davantage connu est un maillon bienvenue afin de faire en sorte que la période qui sépare la publication d'une loi de l'intervention des mesures réglementaires d'application sera plus brève possible une exigence de célérité et d'efficacité qui répond à une triple exigence de démocratie de sécurité juridique et de responsabilité politique. Ainsi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser comment fonctionne ce réseau et quels sont les résultats attendus de cette initiative. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le Sénateur, Buy. Comme je l'ai en effet indiqué dans mon intervention liminaire comme vous l'avez rappelé la Première ministre a souhaité donner une nouvelle impulsion au processus d'application des lois en rappelant ses grands principes, ainsi que ses modalités de mise en oeuvre en lien notamment avec les assemblées parlementaires. À cette occasion, la Première ministre a souhaité réaffirmer la position centrale des correspondants ministérielle de l'application des lois, créé en 2011 et vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur le Sénateur. Ce rôle essentiel a été mis en exergue à plusieurs reprises depuis l'année dernière. Les correspondants ont ainsi été étroitement associée au groupe de travail sur l'application des lois conduit par le SG. Qui aboutit à une refonte des méthodes de travail des guides de procédure Ferrand et des outils de suivi en septembre 2022 dans un 1er temps et à l'élaboration de la circulaire de décembre 2022 dans un second temps. Les correspondants se sont vus confortés comme les interlocuteurs uniques du et Gégé en matière d'application des lois et de suivi des ordonnances et des rapports, enfin dans l'optique de fluidifier les échanges, la plateforme osmose développé par la Dinu m'a été déployée en février 2023 au sein du réseau. Ainsi le SG met à disposition de ses. Davantage outils données détaillées Annuaire des correspondants, élément de calendrier afin d'anticiper au mieux les différents exercices. Plateforme de discussion également. Ces différentes actions visent à conforter le rôle des correspondants ministériel comme tour de contrôle de l'application des lois dans chaque ministère, afin d'assurer un suivi centralisé de l'ensemble des textes prix et de pouvoir répondre avec le souci d'un processus d'applications toujours plus rapide et cohérent en conformité aux demandes réitérées du président Patriat depuis de nombreuses années. La parole est maintenant Monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste. Merci monsieur le président, madame la présidente Gruny, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le débat annuel sur l'application des lois me donne l'occasion de formulé 3 observations Monsieur le Ministre, le 1er qui concerne le recours trop fréquent à la procédure accélérée. Cela a déjà été dit 45, loi sur 64 la procédure accélérée, suppose un caractère d'urgence. Or 21 de ses lois attendent leurs décrets d'application. Elles sont donc en souffrance, ce qui permet d'interroger où est passé l'urgence qui motiver le recours à cette procédure. Deuxième observation, Monsieur le Ministre, vous savez, ici au Sénat. Parmi les règles qui m'ont été inculquées. Depuis mon arrivée dans cette haute assemblée, c'est que nous sommes particulièrement parcimonieux pour ne pas dire chiche sur la commande des rapports qui sont faites. Or il y a un certain nombre de rapports 2 tiers d'entre eux en particulier que nous attendons désespérément pour éclairer nos travaux et nous permettre de mieux légiférer pour les projets de loi les propositions de loi que nous aurons à examiner dans les prochains mois. Comment comptez-vous y remédier. 3ème observation qui concerne cette fois-ci la loi 3DS. Vous le savez il rit existe aujourd'hui encore une cinquantaine de décrets et d'arrêtés qui n'ont pas été publiés qui concernent des sujets qui sont tout sauf mineur. Quelques exemples. Le décret qui concerne. Le classement en calamité naturelle exceptionnelle pour les territoires ultramarins avec les changements climatiques, malheureusement il est à craindre que ce genre de phénomène ne se produise 2ème décret qui en attente toujours, c'est celui qui est relatif à la dénomination des voix et des lieux-dits par les conseils municipaux. C'est tout sauf anecdotique parce qu'effectivement lorsque vous n'avez pas une voix qui est clairement dénommé à lui dit qu'est clairement. Mais vous ne pouvez pas recevoir votre courrier dans les délais normaux troisième type d'exemple c'est le décret d'application qui concerne le Cnfpt, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion et je prends ma casquette de délégué du Centre national de la fonction publique territoriale d'Occitanie. Nous attendons toujours ces décrets pour pouvoir accompagner du mieux possible les collectivités, les municipalités, les départements et les régions. Merci beaucoup monsieur le ministre, de vos réponses. Monsieur le Ministre. monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Vous évoquiez un certain nombre de sujets que nous avons déjà évoqué mais pour la procédure accélérée, c'est devenu la norme régulièrement depuis un certain nombre d'années, je pense que ça notamment une utilité en terme de volume de textes traité au Parlement dans son ensemble. Ça aussi. Un intérêt en terme en terme de normes qui sont En l'occurrence. Très présente et qui donc permet clairement à ses textes en procédure accélérée d'aller d'aller plus vite et donc de répondre plus rapidement aux besoins des administrés et puis ça permet d'avoir une CMP comme je l'évoquais à la fin de la première lecture. Sur les rapports. J'ai me suis déjà. Exprimé sur le sujet, je voudrais quand même vous rappeler que sur la loi 3DS plus spécifiquement au 31 mars. Nous avions un taux de d'application de 61% et au 31 mai, un taux de 71%. Alors il reste du travail à faire. Je vous répondrai très précisément par écrit parce que j'ai pas les réponses spécifiques au décret que vous avez évoquées, mais en ce qui concerne plus largement cette problématique de de ralentissement. De la sortie des décrets concernant la loi 3DS.

il y a aussi de nombreuses. Consultations obligatoires sur les mesures réglementaires à prendre et puis. Il y a eu, comme je l'aurais plaît tout à l'heure une forte inflation. Des, des mesures d'application entre le texte proposé par le gouvernement et le texte final. Je rappelle 36. 38 au départ 96 au moment de la promulgation du texte. Et puis encore une fois, je répondrai précisément. À vos questions sur les décrets que vous avez précisément cité. Merci la parole est maintenant madame la présidente, Éliane Assassi. Pour le groupe CRCE. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, mes chers collègues. 14 des 29 mesures de la loi dite de sécurité globale ont été rendue applicable, ce qui veut dire que moins de la moitié des dispositions ont cours les autres demeurant lettre mordent simple palabres, nous n'avons eu l'occasion de le dire depuis mai. Comment ne pas se réjouir que l'ex-article 24, devenu article 52 contesté dans une tribune publiée dans Le Monde par 3 prix Nobel de la paix par un homme extrêmement large de manifestantes et de manifestants de parlementaires. Et de militants politiques et associatifs fut censurée avec 4 autres mesures par le Conseil constitutionnel, marquant un camouflet pour ces dispositions que nous considérons contraire à la liberté d'informer et flou dans la applications. Nous sommes donc face à l'exemple typique d'un projet de loi qui clive la société dans toutes ses composantes. Pourtant, ce texte ne produira que peu d'effet en droit, d'une part pour des raisons inhérentes à son inconstitutionnalité et d'autre part, de la simple volonté du gouvernement de ne pas l'appliquer. Se pose alors une question simple, pourquoi agir contre les intérêts du plus grand nombre de négliger les principes constitutionnels. Outre qu'une seule habilitations à légiférer sur ordonnance sur quatre était utilisé par le gouvernement, le texte continue de produire des effets. Plus de deux années après sa promulgation, un arrêté du 8 janvier 2023. Pris à bas bruit introduit la connaissance des principes de la République au de formation obligatoire pour exercer dans la sécurité privée, prévue à l'article 23, ces dispositions auront pour conséquence de substituer 3h de formation initiale au nom de l'apprentissage des valeurs de la République au détriment d'enseignements fondamentaux sur les libertés publiques ou les remontées d'informations. Face à la gravité de telles dispositions. Je crains que le gouvernement des volontairement temporiser jouer la montre pour éviter de prendre ces mesures réglementaires en pleine ébullition. Face à ce projet de loi contestée. Je vous le disais il y a des cas où nous préférerions que le droit que vous produisez ne fusent pas appliqué. Monsieur le Ministre. Je sais pas s'il y a vraiment une question mais madame la présidente. Ah ça si je vais évoquer quelques points. Concernant l'application de la loi sécurité globale. Du 25 mai 2021 de la loi principes de la République du 24 août 2021. C'est de loi atteignent un taux d'application respectivement de 94% et de 100% pour la deuxième. Les 2 mesures restant à prendre pour la loi sécurité globale concerne les conditions dans lesquelles le port d'armes hors service par un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public, le texte étant en cours d'échanges inter-, services et d'autre part les missions et la composition des groupes locaux de traitement de la délinquance qu'un procureur de la République ou son représentant peut créer et présider lorsqu'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le décret étant en cours de finalisation. 2 ordonnances importantes ont par ailleurs été prise en application de la loi du 25 mai 2021 la première du 30 mars 2022 relatives aux modalités d'organisation de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de priver de sécurité créée en 2011 dans la contexte de préparation de la Coupe du monde de rugby des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette ordonnance permet au gouvernement de disposer ainsi d'un organe de régulation réel. Et au nord de marche afin de contribuer à la sécurité de ces rencontre sportive. Dans le cas du continuum de sécurité la seconde ordonnance du 16 mai 2023 et relatives à la formation aux activités prévues de sécurité et son objectif est de poursuivre la moralisation du secteur de la formation aux activités privées de sécurité et d'en améliorer la qualité. L'ordonnance a été élaboré sur la base de large concertation menée en 2022. Les principales mesures. Mesures de l'ordonnance sur la création d'un agrément de dirigeants d'organismes de formation et d'une carte professionnelle de formateur. L'encadrement des conditions de sous-traitance et l'encadrement des conditions d'organisation des examens pour en garantir la fiabilité. 2 ordonnances importantes ont ailleurs été prise en application donc de la loi 2021 mais je voulais déjà évoqué. Je le Ministre vous constatez que vous venez de répondent que sur ce texte de loi. Tout a été pris justement au moment où Madame la présidente disait justement sur ce texte de loi, elle n'en voulait pas, mais c'est gentil de lui avoir quand même répondu très bien allez dernières interventions celle de madame Amel Gacquerre. Pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la loi Egalim promulguée en 2018, prévoit plusieurs mesures très ambitieuses pour améliorer la qualité des repas servis par la restauration collective. L'article 24, par exemple, fixe un objectif de 50% de produits durables et de qualité dans l'offre alimentaire proposé par les institutions publiques. Cette priorité donnée aux produits de nos terroirs et notamment aux produits dont la qualité reconnue à l'image de nos AOP IGP ou du Label Rouge, constitue un signal fort envoyé aux agriculteurs et producteurs en effet cet objectif constitue un levier important pour soutenir la structuration de nos filières agricoles notamment agro- agro- écologique et pour le développement de la production locale. 3 ans plus tard en 2021, la loi climat et résilience a été plus loin, elle a rehaussé cet objectif ambitieux en le fixant à 60% de produits durables et de qualité pour les produits animaux et cela au plus tard au 1er janvier 2024. Pourtant, Monsieur le Ministre, au 1er janvier 2022, le compte n'y est pas. En effet, selon les chiffres de l'Observatoire national de la restauration collective bio et durable. Un tiers des cantines scolaires n'atteignent pas. Par exemple l'objectif intermédiaire de 20% des produits durables lors de l'année 2021. Monsieur le ministre, il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Il sont primordiaux pour la santé de nos concitoyens et pour soutenir nos agriculteurs. Qu'en est-il. Qu'est-il fait pardon aujourd'hui afin d'atteindre ses objectifs fixés par les loi Egalim et climat et résilience. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Le gouvernement est pleinement engagé pour la mise en neuf des objectifs fixés Parlement par le Parlement en la matière. D'une part des mesures d'accompagnement avec la mise en place en juin 2022 d'un groupe de travail économique du Conseil national de la restauration collective, à la demande des parties prenantes. D'autre part avec la création de la plateforme ma cantine dédié aux gestionnaires de cantines afin de les accompagner dans la mise en oeuvre de la loi. Et par des marges de manoeuvre actionnés sur le levier de la commande publique, notamment grâce aux adaptations adoptés dans la loi climat et résilience et d'autre part, à travers des mesures financières, avec une enveloppe de 50 millions d'euros de soutien aux cantines des petites communes pour financer l'achat d'équipements nécessaires à la cuisine et la transformation de produits frais et former les personnels. D'autre part avec une enveloppe de 85 millions d'euros pour les projets alimentaires territoriaux étroitement lié à la restauration collective et bien souvent évidemment en lien avec les agriculteurs, que vous évoquiez tout à l'heure et avec, enfin une politique de tarification sociale pour accompagner les collectivités locales avec 100.000 enfants ayant bénéficié de repas à un euro. euro. Voilà monsieur le président, si vous le permettez, je crois que c'est la dernière. Question auquel je dois répondre à laquelle je voudrais répondre. J'en profite donc pour remercier Madame le président ses équipes de la DLC. Le secrétaire général du gouvernement, mon équipe et bien sûr mais dans des des sénatrices et messieurs les sénateurs pour le travail réalisé. Madame Deckers. Il vous reste 20 secondes, non. Très bien, merci infiniment, Monsieur le Ministre, nous allons passer au débat suivant.

L'ordre du jour appelle le débat sur la gestion des déchets dans les outre-mer à la demande de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute. Madame la Ministre, vous pourrez donc. Si vous le souhaitez pendant près chaque orateur. Et naturellement. Vous interviendrez. À la fin du débat la parole et tout d'abord aux orateurs de la délégation qui a demandé ce débat. Et la parole est à madame Gisèle Jourda au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Si je devais résumer avec ma collègue Viviane Malet. Le principal enseignement de nos travaux sur les déchets dans les outre-mer je retiendrai assurément le mot urgence. Urgence à agir pour répondre à la double urgence sanitaire et environnemental. Dans la plupart de nos territoires ultramarins, la cote d'alerte est dépassée. Ce mot n'est pas galvaudé, je dois avouer que ce que nous avons appris et vu de nos yeux vu au cours de notre mission ma plusieurs fois choqué et bouleversé. À Mayotte, tout particulièrement, nous avons constaté l'existence de décharges sauvages à ciel ouvert, au coeur de bidonvilles au milieu desquelles des enfants jouent. Des tas de déchets il brûle. Continuellement lors de pluies violentes. Une grande partie de ces déchets finissent dans le lagon et la mangrove à Saint Pierre et Miquelon, où pourtant la collecte et le tri sont exemplaires des décharges littoral brûle à ciel ouvert à chaque tempête, une partie des déchets, fini à la mer. L'urgence environnementale est criante et cette pollution ne vient pas de l'autre bout du monde. Notre responsabilité est entière, alors même que les outre-mer concentrent 80% de la biodiversité française. Notre mission a aussi mis en évidence l'urgence sanitaire à laquelle doivent faire face ces territoires les maladies favorisées par cette situation sont notamment la dingue l'hépatite A, la typhoïde et la leptospirose la collecte déficiente dans des zones. Difficiles d'accès ainsi que dans les quartiers informels. Le fléau des dépôts sauvages et le poison lent des anciennes décharges illégales sont autant de dangers pour des territoires fragilisés. Cet état d'urgence Madame la Ministre et la conséquence directe du retard majeur des outre-mer. Quelques indicateurs rendent compte de ce décalage complet. Le taux d'enfouissement suffit à offrir un aperçu du rattrapage nécessaire au niveau national, 15% des déchets ménagers sont enfouis 85% étant valorisé en outre-mer le rapport est inversé. À l'exception de la Martinique qui a enfoui en 2020 40 % de ses déchets ménagers et de Saint-Barthélemy, tous les autres territoires affichent des taux d'un fouillis se de 60 à 80%. Pratiquement 5% à Mayotte en Guyane ou à Saint-Martin. Alors que faut-il faire en premier lieu, il faut souligner la forte prise de conscience sur tous les territoires, les militaires, les initiatives fourmillent pour inverser la tendance et trouver des solutions innovantes et adaptées. En second lieu, cette situation ne résulte pas d'un désengagement des autorités responsables au contraire les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que l'État sont mobilisés et fournissent des efforts financiers importants. Pourtant, ces efforts ne suffisent pas à rattraper un retard structurel et un nouvel élan est nécessaire. Plus qu'un élan cet homme plan Marshall qu'il faut voir un plan Marshall XXL pour Mayotte et la Guyane. Ma collègue co-rapportrice Viviane Malet dès qu'il aura dans un instant ce plan Marshall qui s'articule autour de 26 recommandations concrètes et précises. Je conclurai en évoquant l'aspect européenne les spécificités des régions ultrapériphériques n'y sont pas assez prises en compte les discussions en cours sur la révision du règlement européen relatif au transfert des déchets en témoigne dans le droit fil de notre rapport, nous avons déposé une proposition de les auditions qui sera examiné examiné par la commission des Affaires européennes où nous aurons à coeur bientôt avec ma collègue Marta de Cidrac d'en débattre pour continuer à tracer le sillon de ce rapport qui se veut, qui se veut un levier pour agir fort et pour argile vite je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Viviane Malet au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, nous 26 recommandations découle directement du diagnostic qui vient de vous être présenté par ma collègue Gilles elle Jourda une nouvelle stratégie doit être bâti notamment pour préserver la santé et bien sûr l'exceptionnelle biodiversité de nos outre-mer qui ne peuvent pas devenir des territoires dépotoir. Les outre-mer doivent donc et d'urgence relever 2 défis un premier à court terme, gérer l'urgence et et en retrouvant des moyens d'action et consolider les bases d'une gestion des déchets maîtrisé. Deuxièmement à long terme, s'engager résolument sur la voie de l'économie circulaire qui est un chemin plus long mais plus durable. Cette stratégie passe d'abord par l'adoption de plans de rattrapage exceptionnel cousu main. Pour chaque territoire ces plans devront être. Un des volets prioritaires des futurs contrats cadres ces plans ainsi que des adaptations ciblées de la réglementation, en particulier en matière de gouvernance et d'action Découvrez organisme. Permettront. De prendre le virage d'une économie circulaire réaliste et adapté aux contraintes de ces territoires. Le temps qui nous est accordée ne permet pas de présenter toutes nos recommandations a 26 bien sûr je me concentrer sur les principales, la première concerne les financements, nous estimons que des financements supplémentaires exceptionnelle de l'État à hauteur de 100, 250 millions d'euros sur 5 ans sont indispensables pour réaliser des équipements prioritaires et structurant. En plus des aides actuelles de l'état des déchetteries qui par exemple des centres de tri boire des formes de stockage, manquent presque partout. La 2ème proposition forte et l'exonération de la TGAP pendant 5 7 ou 10 ans selon les territoires. Depuis plusieurs années, du bricole on des rabais ponctuelles et partielles sans visibilité. Il faut une exonération claires prévisibles qui redonnera immédiatement des marges de manoeuvre au budget de fonctionnement des oeufs PDI et des syndicats mixtes. 3ème axe fort une contractualisation entre tous les acteurs avec des engagements sur les objectifs et les calendriers cette contractualisation inclura une mise en commun de l'ingénierie autour de plateformes de projets 4ème priorité responsabilisé des éco-organismes malgré les progrès de la loi geeks il ne rattrape. Que très lentement le retard accumulé depuis plus de 20 ans, malheureusement sans. Nous n'avancerons pas au rythme exiger. Aussi, à défaut de progrès spectaculaires à court terme, il ne faut expérimenter d'outre-mer un mécanisme incitatif de pénalités financières qui pèserait sur les échos Garnier qui n'atteignent pas leur objectif territorialisée 5ème propositions importantes toujours en lien avec l'accent mis sur les éco-organismes. Nous proposons d'abaisser à une tonne au lieu de 100, le seuil à partir duquel le coup de nettoiement d'un dépôt sauvage et pris en charge par les secours gagner il faut envoyer un signal fort le rattrapage doit être rapide et nette et non pas étalée sur 20 ans. Notre 6ème proposition porte sur la gouvernance. Ou qu'il convient d'aller vers un opérateur unique sur chaque territoire, en charge du traitement des déchets. Il manque encore une véritable instance de pilotage dans ce but, nous proposons que dans chaque région. La commission consultative d'élaboration et de suivi C. C. E S du plan régional de prévention des déchets devienne un vérité une véritable instance de coordination et de pilotage. Septièmement développer des dispositifs de gratification directe du tri pourront que j'ai les collectes sélectives dans des zones défavorisées ou isolées des projets locaux innovants ont déjà montré leur pertinence. Il faut aller plus loin, par exemple à Mayotte. Enfin, nous plaidons pour le développement de la valorisation énergétique des déchets dans les outre-mer avec un cadre pérenne pérenne et favorable au prix de rachat de l'électricité ainsi produite. Malgré tous les progrès possible en matière de recyclage de réemploi de prévention de déchets. Il nous paraît pas réaliste d'imaginer une gestion des déchets outre-mer sans un véritable essor de la valorisation énergétique. Je terminerai en remerciant ici la présidente du Groupe d'études sénatoriales sur l'économie circulaire Marta de Cidrac ainsi que ses collègues qui ont suivi et enrichi nos travaux ce travail de concert permettra de donner à nos travaux les législatives qu'ils appellent, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite du débat. La parole est à Madame Micheline Jacques pour 7 minutes pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues la gestion le traitement, la valorisation des déchets sont parmi les nombreux défis que les autres maires ont à relever. À cet égard le constat du rapport que nous ont présentés nos collègues et Gisèle Jourda et Viviane Malet est à la fois précis éclairants est alarmant, décrivant une scène glaçante à Mayotte nos collègues nous fournissent une photographie des conséquences du retard de la gestion des déchets sur les populations et l'environnement qui ne peut nous laisser ni insensible ni inactifs et même si l'image est pas rock sismique. Au-delà du constat, nos collègues nous oriente vers des pistes destinées à corriger les politiques publiques de gestion des déchets dans l'inadaptation semble être à bien des égards la source des situations sur lesquelles vous nous alerter. Au fil des pages, le caractère multidimensionnel de l'enjeu de la gestion des déchets apparaît nettement. De même que la nécessité d'aborder l'indispensable rattrapage avec des solutions pragmatiques et à partir d'un regard lucide à ces conditions, il est possible de résoudre l'épineuse question du traitement des déchets en s'appuyant sur les leviers de développement qu'elle renferme. Saint-Barthélemy a très tôt défini une politique de gestion et de traitement de ces déchets garantissant son autonomie. Cette organisation que l'on doit d'ailleurs à Michel Magras, reposait sur l'idée que la propreté de Lille conséquence visible de l'élimination de la gestion des déchets devait se situer au coeur de la politique économique de l'île compte tenu de sa dimension fortement touristique tout autant que de sa politique environnementale. C'est ainsi qu'elle est devenue une priorité de politique publique et partant d'engagement financier sa Barthélémy a donc fait le choix des 2002 du traitement par incinération couplée à une valorisation énergétique permettant d'alimenter l'usine de dessalement. Dès lors, totalement autonome. La gouvernance simplifiée et l'étroitesse du territoire ont certes favorisé le succès de cette politique mais qui n'aurait pu être totale sans l'adhésion de la population qui est primordial, l'économie de Saint-Barthélemy en fait un territoire importateurs et producteurs de déchets pour rester attractif le traitement et la gestion des déchets doivent continuer de constituer une dépense prioritaire pour la collectivité. C'est donc forte de cette expérience que je souscris d'emblée à l'ensemble des préconisations de nos collègues. Parler du traitement des déchets outre-mer est une nouvelle occasion d'éprouver le cadre normatif et son adaptation à ces territoires en effet comment réussir une politique publique, lorsque les normes qui s'y appliquent constitue un frein. Dans un contexte où le déficit d'ingénierie a régulièrement pointé la complexité des objectifs et le premier obstacle au bon développement d'une politique efficiente de gestion de déchets le panorama nous est qui nous est présenté, bien s'il en était besoin renforcé la conviction de la nécessité de former davantage en fonction des besoins. J'ai eu l'occasion ma qualité de rapporteur pour avis de la mission Outre-mer de préconiser la création d'au moins une école d'ingénieurs par bassin océanique notre République qui a raison d'être exigences ne cesse de durcir les objectifs et les contraintes qui pèsent sur la gestion de nos déchets souvent irréalistes au regard des situations ultramarines. L'exemple des cahiers des charges des éco-organismes inadapté aux outre-mer est éloquent, nos collègues relève que seul le cahier des charges de la filière emballages ménagers de ces organismes contient des dispositions propres aux outre-mer. Or, dans la construction de filières responsable élargie du producteur, ils sont des acteurs et des partenaires sans trop le rapport soulève également la complexité des données obstacle à une bonne planification du reste également pointée par la Cour des comptes cette impossibilité de collecter des d'autres n'vient s'ajouter une fragilité générale en cette matière dans les outre-mer une bonne politique de rattrapage pourrait être soutenu par la planification mais elle est difficile à mettre en oeuvre en l'absence de données entre outils la fiscalité applicable aux déchets devraient être un facteur d'encouragement. Si l'on prend l'exemple de la TGAP elle vient au contraire grever les Budgets de fonctionnement des personnes chargées du traitement des déchets alors que les besoins en investissements sont colossaux pour y faire face, une meilleure mobilisation des fonds structurels européens est donc essentiel. S'agissant de la TGAP toujours les les réfaction dont bénéficient les outre-mer sont un facteur d'incertitude, on ne sait à quel horizon. Elles seront supprimés. Alors que la visibilité favorise les investissements, l'affectation de cette taxe au budget de l'État ont par ailleurs de moins en moins compréhensibles dans le contexte ultra-marins. Les pistes d'amélioration suggérés par nos collègues mérite donc d'être explorées, à l'occasion de la prochaine session but budgétaire. Si cela n'a pas encore été fait dans le cadre Lucio. Les besoins en financement sont indéniablement très élevé, que ce soit pour les équipements structurants ou le fonctionnement en effet outre-mer le coût de gestion du service public des déchets est en moyenne 1,7 fois plus important qu'en métropole pour une ressource fiscale moindre en matière fiscale. Les éléments mis en évidence par nos collègues constitue en outre une invitation supplémentaire à l'échange de bonnes pratiques entre territoires ultramarins. Les solutions innovantes et incitatives mises en Oeuvres par Wallis et Futuna ou encore la Nouvelle-Calédonie peuvent utilement nourrir la réflexion sur la fiscalité de l'ensemble des territoires. La gestion des déchets outre-mer est aussi marquée par une culture moins développé des réflexes de tri, de même que la responsabilisation du consommateur. Les points de collecte volontaire et sont moins développés au profit du porte à porte comme je l'indiquais plus haut, une politique de gestion des déchets ne peut se concevoir sans l'adhésion des populations et leur implication. C'est pourquoi, comme le suggère nos collègues il y a lieu d'aborder la question de la gratification sans tabou. Le retard pris dans la structuration des politiques s'est répercuté sur les développements de la culture du tri. Elle doit être plus fortement encouragé outre-mer tout en renforçant l'effectivité des sanctions, cela va sans dire. Au moment où le poids de l'empreinte carbone est au coeur de toutes les politiques publiques. On ne saurait s'en affranchir dans la réflexion des déchets outre-mer qui sont dans ce domaine, marqué par une forte dépendance aux exportations. Dans cette optique, la valorisation et la prévention offrent des solutions pour réduire le coût écologique de la gestion des j'ai envisagé cette fois dans le cadre des échanges le tribut payé localement par l'environnement est déjà bien lourde du fait de l'enfouissement habiliter les collectivités à définir les matières dont elles autorisent l'entrée elle a encore une préconisation particulièrement pertinente. À côté, priorité doit être donnée au développement de filières de valorisation en particulier énergétique. Le rapport sur le logement social relevait déjà des difficultés résultant de l'absence de gestion locale de l'amiante qui pourrait peut être faire l'objet de réemploi j'en terminerai par cet aspect l'encouragement au réemploi dans une optique de développement d'économie circulaire est un autre outil de gestion de déchets qui doit être encouragée. Merci cher collègue. Réveiller l'hémicycle. La parole est maintenant monsieur Jean-Louis Lagourgue pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la Ministre naturellement vous me demandez à tout enfin à tout moment après chaque orateur si vous souhaitez sinon vous intervenez à la fin. Monsieur Lagourgue 5 minutes pour le groupe les indépendants. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Ensemble pour une ville plus propre ces slogans c'est le slogan de l'association propre réunion qui oeuvrent depuis 2017 grâce à ses bénévoles à nettoyer la réunion des dépôts d'ordures sauvages. Je souhaite ainsi commencer par saluer toutes les initiatives locales et bénévoles qui contribuent à la préservation de nos territoires. En effet, certains d'entre nous, on peut être déjà entendu quelqu'un revenir d'un voyage dans l'un de ces territoires ultramarins et dire. Et pour cause, c'était magnifique. Mais qu'est-ce que c'était sale. Dans certaines ces territoires, des paysages de cartes postales sont malheureusement parfois entachés d'ordures. Bien sûr, c'est aussi le cas de certains territoires hexagonaux. Mais comme souvent dans les outre-mer les problématiques sont exacerbé par l'insularité. Le climat, la densité de population et la taille des territoires. Malheureusement la problématique des déchets dans les Outre-mer ne se limite pas au dépôt sauvage et c'est souvent toute la chaîne de gestion qui est en difficulté. De la collecte, traitement et même si la situation demeure très inégale selon les Drôme comme la situation était ainsi beaucoup plus alarmante à Mayotte et en Guyane. qu'elle ne peut l'être à Saint-Barthélemy, où à la Réunion. À d'iode à titre d'exemple Mayotte et la Guyane enfouissent presque 100% de leurs déchets entre 15% au niveau national. Pourtant les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets sont nombreuses, risques sanitaires, tout d'abord avec une problématique prolifération de certaines maladies comme la dengue, la typhoïde ou la leptospirose risque économique ensuite pour certaines de ces régions, dont l'économie est axée sur le tourisme et dont la dégradation des paysages à cause des déchets risquerait de détourner. Les touristes de ces destinations enfin risques environnementaux dans les territoires qui à eux seuls n'abrite pas moins de 80% de la biodiversité française et de nombreuses espèces endémiques. Les nombreuses décharges illégales actuelle ou ancienne dans lesquelles des batteries sont abandonnés polluent les sols et les nappes phréatiques. Comme le souligne le rapport de la délégation sénatoriale sur le sujet ces situations résultent de causes diverses qui se cumulent parfois voire souvent sur le même territoire, problème de gouvernance avec une multiplicité d'acteurs qui ne parviennent pas à se coordonner financement insuffisant pour permettre une remise à niveau rapide éco-organismes est pour le moins discret. Dans le cas des filières responsabilité élargie du producteur ou encore des difficulté voire impossibilité d'exporter certains déchets. À ce titre, île de la Réunion et sa voisine mahoraises subissent depuis 2020 d'importantes difficultés dans l'exportation de leurs déchets dangereux. Les stocks se sont actuel se sont tellement accumulées, qu'il a été demandé aux producteurs de ces déchets, de les conserver et de déconnecter et des collègues des collègues qui ont été interrompues. Nous avons ainsi dû stocker l'équivalent de plus d'une année de déchets dangereux. Dont des batteries et des piles des boues chargées d'hydrocarbures en cause la saturation post-Covid du transport maritime conjugué à des compagnies particulièrement frileuse à transporter des déchets dangereux. À raison d'une réglementation complexe. Si la situation du moins pour ce qui est du surstockage a pu être établi en octobre dernier à coups de négociations et de procédures exceptionnelles. Elle pose évidemment la question de la dépendance, nos 2 régions de l'océan Indien aux liaisons maritimes vers l'Europe, situé à plus de 9000 et eurodéputés ont arrêté en janvier dernier leur position. Je suis un durcissement de la réglementation relative à l'exportation des déchets hors de l'Union européenne, qu'ils soient dangereux ou non. Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que la France usera de toute son influence lors des négociations à venir afin que les nouveaux textes tiennent compte des contraintes propres aux outre-mer comment comptez-vous soutenir les initiatives locales qui fleurissent pour le recyclage de déchets en matière de crédit messieurs tout en matière de gouvernance. En parallèle, comment comptez-vous appuyer le développement de la coopération régionale entre août outre-mer français d'une part, et entre les Outre-mer et d'autres États d'une même zone géographique. D'autre part, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Merci à la délégation aux outre-mer à Gisèle Jourda et à Viviane Malet pour leur considérable travail de y être plongé m'a convaincu que la problématique des déchets outre-mer hé bien moins une particularité exotique, une simple affaire de retard qu'une mise à l'épreuve en conditions compliquées et disparate de notre politique publique globale un révélateur de de ces carences de ces dérives, mais aussi des innovations prometteuses qui interpelle. Notre responsabilité politique et qui peuvent nous amener à des adaptations des avancées dont le bénéfice pourrait profiter autant aux Outre-mer qu'nos territoires de métropole aux outre-mer les difficultés, les freins joue sans doute plus qu'ailleurs, les coûts sont structurellement plus élevés. Reste que, comme partout ailleurs. L'équation est du même ordre que chacune des 3 parties, producteurs, consommateurs pouvoirs publics assume pleinement ses responsabilités, responsabilités des producteurs. Quant aux impacts et à la fin de vie de leurs produits. Or le système des REP est extrêmement peu contraignant Les Échos ne sont pas tenus à des objectifs par territoire pour les Outre-mer, c'est encore plus handicapant qu'ailleurs. La responsabilité des consommateurs pour des usages et des comportements vertueux rendue d'autant plus indispensable par les difficultés de collecte là par des apports volontaires, les contraintes de l'insularité et de la surexposition aux risques naturels. La responsabilité, enfin des acteurs publics, collectivités, État, Europe législateur pour que les normes les règles, les cahiers des charges, les moyens d'investir et de fonctionner durablement les contrôles, les sanctions et l'accompagnement soit à la hauteur des enjeux, des contraintes spécifiques et des trajectoires. Dingue paludisme saturnisme hépatite A ces maladies prolifèrent dans de nombreuses régions d'outre- mer parce qu'une partie des déchets se retrouvent dans des décharges ou tout simplement comme dépôt sauvage comme épave. Aussi de véhicules dans la nature, les outre-mer abrite 80% de la biodiversité française lorsqu'une mangrove hein lagon une forêt ou un cours d'eau se transforme en dépotoir. C'est un désastre écologique sanitaire social touristique aussi. La France est ambitieuse pour un traité international sur la pollution plastique cette ambition nécessite une application concrète dans nos Outre-mer impacté parmi les recommandations du rapport de la délégation aux outre-mer je retiens 2 idées-forces. D'abord la nécessité de. C'est l'exigence de notre système de responsabilité élargie des producteurs l'éco-organisme mandataire du metteur sur le marché doit être tenu par un objectif. Pourquoi. Sinon, on ferait-il des efforts en Guadeloupe ou en Guyane, si cela lui coûte plus cher qu'en métropole et qu'il ne risque pas qu'ne qu'ne risque pas de sanction, s'il n'atteint pas de résultats dans ces territoires où collecté, recyclé. Hé bien plus cher qu'à Strasbourg ou à Lyon, il s'agit donc d'habiliter les outre-mer à intervenir dans les cahiers des charges à adapter à adopter leurs propres normes de mise sur le marché de consigne de réemploi pour que nos outre-mer est un levier d'action déterminant il faudra abaisser de à une tonne le seuil à partir duquel le coup de nettoiement d'un dépôt sauvage et pris en charge par les éco-organismes 2ème idée-force de cette série de recommandations fournir à nos outre-mer les moyens de répondre au niveau nettement plus élevé des coûts pour leurs déchets, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas là de mauvaise gestion publique mais de spécificités qui font qu'en Outre-mer c'est largement sur les contribuables. Sur l'ensemble de la population. Que pèse le coût du traitement des déchets issus d'activités économiques ou que par exemple comme le dit à l'association Amorce. On ne monte pas un centre de tri outre-mer aussi aisément qu'on le fait en région parisienne, il apparaît évident que des plans de rattrapage exceptionnel s'impose. L'État doit mettre sur la table des moyens financiers, particulièrement en faveur des territoires de Mayotte et de la Guyane 250 millions sur 5 ans au minimum, permettant aux collectivités de mettre sur pied les infrastructures prioritaires les équipements structurants, donner les moyens, c'est aussi remédier aux effets plombant de la TGAP dont les paramètres déterminés pour la métropole vise notamment à éviter qu'ils reviennent moins cher de mettre des déchets en décharge que de les recycler ce bon principe devient contre-productif en outre-mer où l'enfouissement à une telle part que la TGAP fonctionne comme un frein plutôt qu'une incitation à agir car il prive de moyens de financer l'indispensable rattrapage la recommandation 12 d'exonérations TGAP adaptée pour les territoires d'outre- mer est donc capital de même pour l'aide au fret pour lever les entraves à la mutualisation et à la massification des flux de déchets à traiter entre territoires proches enfin la recommandation 23 largement développé dans le projet de résolution européenne de nos collègues vise opportunément à rendent plus adapté aux outre-mer les dispositifs et les aides européennes. Pour conclure, si tout ce débat toutes ces attentes. Ce rapport de la délégation cette résolution européenne à venir en rester là, qu'elle ne se traduisait pas en actions concrètes. Ce serait une immense déception je parlais à l'instant de responsabilité des acteurs publics Madame la Ministre celle de votre gouvernement est particulièrement attendu. Merci cher collègue. La parole est maintenant Monsieur Georges Patient pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président. Madame la Ministre. Monsieur le président de la délégation aux outre-mer. Mesdames les rapporteurs, chers collègues. En matière d'urgence, tout est question de perception et de référentiel. Il semblerait que la gestion des déchets en outre-mer mer passe sous les radars de l'État. C'est une urgence qui dure depuis de nombreuses années. Et qui semble être appelée à durer encore longtemps. L'excellent rapport de nos collègues Gisèle Jourda et Viviane Malet en dresse un tableau édifiant. Peut-être permettra-t-il de réveiller les consciences. Je tiens à les remercier et les féliciter pour leur travail précis et exhaustifs. Comme le rappelle ce rapport, la gestion des déchets et tout autant un enjeu de santé publique. Que de protection de l'environnement ou de développement économique de la même importance. Que l'assainissement, ou l'adduction en eau potable. L'urgence n'est donc pas seulement dans le respect d'une réglementation européenne ou dans l'application d'une loi. L'urgence se situe bien dans la protection de la santé des habitants de nos territoires. Et de la préservation du Cadre de vie. Avant même d'évoquer l'économie circulaire, comme précisé dans le rapport. Or les défaillances apparaissent à tous les niveaux du parcours. D'un déchet de sa production à son élimination. Nous en sommes encore à éviter qu'une majorité des déchets finissent dans la nature. C'est pourquoi les investissements doivent avant tout aller vers les équipements de base. Comme les centres d'enfouissement des déchets. Les incinérateurs les déchetteries ou les outils de collecte. Les taux de collectes sont insuffisants. Par exemple, sur mon territoire. La Guyane. Pour certaines cours communes complètement. Il en reste malheureusement quelques-unes. Les seuls moyens d'accès sont la pirogue ou l'avion. La collecte et l'acheminement des déchets verts, centre de tri ou de traitements. Il reste une gageure. Si la collecte est problématique le cri le traitement et la valorisation le sont tout autant. Avec 2 déchetterie et 2 installations de stockage de déchets non dangereux. La Guyane affiche un taux de valorisation extrêmement faible de 18%. La grande majorité de ce qui est collecté fini enfoui. Et c'est le cas pour tous les outre-mer avec un taux moyen de 67% contre 15% au niveau national. La collecte et la mère des batailles. Plus nous collectons plus nous protégeant la population et mieux nous pouvons gérer. Trier et valoriser avec des filières Savall rentable mais qui pour financer cette coulée. Le rapport cite le cas extrême de la commune de Camopi en Guyane. Qui ne touche aucune taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cas particulier de certaines communes de Guyane où le fasse où le foncier appartient intégralement à l'État. Hein. Foncier non imposables. Mais en moyenne en outre-mer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne couvre que 80% du coût du service public. Avec certaines communes à seulement 15%. Les EPCI de Guyane et de Mayotte sont les plus en difficulté avec des taux de couverture d'à peine 25%. Et de 50%. C'est intenable. C'est pourquoi il faut faire appel à la solidarité nationale et mettre en place une taxe. À l'image de ce qui existe pour l'électricité avec la taxe sur la consommation finale d'électricité, également appelée. Contribution au service public de l'électricité. Une taxe qui aidera à financer le service public de déchets dans les régions d'outre-mer. Les régions les plus défavorisés, mais où les coûts de ce service sont les plus élevés. Comment en Guyane et à Mayotte. Par exemple pour le PIB par habitant est respectivement de 42% et 26% de la moyenne nationale. La population peut-elle financer un système qui coûte une fois cette plus que dans l'Hexagone. Il y a là une terrible injustice. Par ailleurs, je ne peux que souscrire à la recommandation des rapporteurs. Confirmant une exonération de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette taxe. Transposition du principe pollueur-payeur séduisante sur le papier, sauf dans les Outre-mer 2 défauts majeurs. Il n'y a pas d'alternative au stockage, faute de rentabilité. La trajectoire à la hausse du coût de la tonne fait gonfler le montant de la taxe. Sans possibilité pour les collectivités de faire supporter son coût par l'air particulier ou de réorienter les déchets vers d'autres filières. Au final, cette taxe se révèle contreproductive car en aggravant les coûts de fonctionnement elle oblitère sérieusement les capacités d'investissement des collectivités donc de transition. Ainsi qu'il est nécessaire de suspendre l'application de la TGAP en outre-mer. Tant que n'existeront pas des alternatives au seul enfouissement. Il serait même bon d'envisager de flécher le produit de cette taxe vers le soutien au développement des filières alternatives. Dans les régions où la rentabilité n'est pas possible. Par ailleurs la tes TGAP génère des comportements d'évitement chez certains professionnels. Qui se débarrassent de leurs déchets dans des dépôts sauvages. C'est un mal qui touche tout le territoire national. Qui abîme les paysages et multiplie les sites pollués. Mais c'est une double peine pour les collectivités. Qui en plus de pays la TGAP doivent assumer les coûts d'enlèvement et de nettoyage. Il faut abaisser le seuil de 100 tonnes à partir duquel ce sont les filières REP qui prennent en charge ces coups comme le proposent les rapporteurs. Enfin on peut se poser la question de la pertinence du dogme de la valorisation par le recyclage comme unique solution. Le coût en sera-t-il supportable pour nos économies étroite est-il envisageable de multiplier ces coûts en regroupant la gestion d'une filière entre plusieurs territoires ultramarins. Mais surtout pourquoi exclure d'emblée. La valorisation énergétique des déchets. Pour conclure, j'aimerais que le gouvernement nous précise s'il entend profiter du prochain conseil interministériel de l'outre- mer le CIOM pour avancer sur ces sujets, je vous en remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Gisèle Jourda pour le groupe socialiste pour six minutes. Monsieur le président. Monsieur le Président de la dégradation Madame la Ministre. Je profite de ce second temps d'intervention pour mettre l'accent sur l'urgence sanitaire liée à cette gestion des déchets. L'insécurité sanitaire, ça n'est pas qu'un sentiment quelques données objectives permettent de mieux appréhender évaluer ce risque qui n'est pas propre aux outre-mer mais qui était exacerbé du fait du climat de la densité de population et de la pauvreté. Je tiens à insister sur les risques sanitaires associés à ces pollutions. Diffuses souvent à proximité immédiate des populations. La commission d'enquête sur les pollutions industrielles et minières des soldes dont j'avais été rapportrice en 2020 avait mis en lumière les risques majeurs de pollution souvent invisibles et dans la mémoire se perd rapidement fait peser, à court et long terme des risques importants sur des populations déjà en situation de Prague de précarité nos auditions et nos déplacements ont mis en évidence une dure réalité sur des territoires de la République qui ne peut être occulté ou édulcoré. Le cas paroxystique de Mayotte doit être une cause nationale. Les décharges sauvages sont à ciel ouvert, au coeur de bidonvilles au milieu desquels des enfants jouent des batteries de voitures, ils servent de Pierre de gué pour franchir des ruisseaux, des femmes lavent leur linge dans des bassins alimentés par ses taux et des tas de déchets il brûle continuellement en Guyane, la situation est assez similaire à la seule différence que l'espace disponible permet de diluer cette sensation de débordements. Alors quelles sont les conséquences de cette pollution. Lors de son audition. La direction générale de la Santé a souligné que l'abandon des déchets sur l'espace public ou privé, notamment les batteries les produits électroménagers ou les véhicules hors d'usage favorise la prolifération d'espèces nuisibles et de rongeurs qui sont vecteurs de maladies transmissibles, aux populations comme la dengue, le paludisme ou la leptospirose à la réunion des regroupements de cas de plombémie et de saturnisme infantile ont été observées autour de zones de précarité dans lesquels des batteries avait été abandonné des pollutions diffuses. À l'avenir. La tendance à une autre hausse quasi exponentielle et très inquiétante pour ne pas dire alarmantes les déchets abandonnés sont autant de shit de gîtes larvaires propices à la prolifération des moustiques, des épidémies régulière de Deng mais aussi 2 zika ou du chikungunya touche régulièrement une grande partie de la population dans les Antilles en Guyane, dans l'océan Indien et dans le Pacifique, elles entraînent des arrêts maladie de nombreuses hospitalisations et des décès. Les rongeurs et les reins en particulier favorise la transmission de la leptospirose qui est une maladie bactérienne grave pouvant conduire à l'insuffisance rénale, voire à la mode un cinq avait % des cas en Guyane. Une centaine de cas et comptabilisé chaque année, le taux est 70 fois supérieur à celui de la France hexagonale. D'autres maladies encore peuvent être favorisée par une mauvaise gestion des déchets comme la typhoïde ou l'hépatite A. Je reprends l'illustration de Mayotte qui cumulent tristement les maladies vectorielles. Les maladies zoonotique également les maladies diri que comme la typhoïde il y a eu 23 cas de paludisme sur les 8 premiers mois de 2022, 3. Suspicion de Deng et 152 cas de l'Epshom cirrhose. Sur les 8 premiers mois de 2022 à ce jour 100 cas de typhoïde ont déjà été des comme des documenté toujours en 2022, il est naturellement impossible d'isoler précisément les facteurs concourant à la transmission de ces maladies ou de l'imputer au seul déchet mais il est certain que les déchets créés à tout le moins, des conditions plus favorables de contamination. Et que dire de la qualité de l'air. Pour sûr, elle est également affectée notamment par l'incinération des déchets verts fréquents sous les climats tropicaux plus grave les indices des décharges dégage des fumées toxiques de tels incendies sont réguliers, par exemple à la décharge de sirop en Martinique en 2021 et je ne parle pas des déchets radioactifs en Polynésie française, notre collègue là Nath ni en parlera mieux que moi. Bien que la question des Sargasses soit en dehors du Champ de ce rapport, il faut aussi citer les émanations de gaz toxique en raison de leur décomposition des zones habitent à proximité des zones habitées, les conséquences à long terme sont encore mal connus. Enfin les déchets industriels et miniers existe aussi à l'outre-mer en Guyane française. Les activités d'orpaillage illégal sont à l'origine d'une double pollution mercuriels liés aux expositions professionnelles et à la contamination des poissons carnivores et puis Ivor la Nouvelle Calédonie et l'autre territoire marqué par une activité minière conséquente. Plusieurs initiatives ont été lancées pour évaluer l'impact sanitaire de ces déchets sur les populations locales. La priorité est de poser les bases réelles, madame la Ministre du nos politiques que des déchets des infrastructures essentielles. Comme Comme les déchetteries ou centres de tri, voire tout simplement de camions de collecte des centres de stockage des comités de Vallauris. Des comités de valorisation énergétique, il faut aller à l'essentiel dans les territoires les plus M. partez Mayotte et la Guyane. Sans ces bases le virage vers l'économie circulaire ne pourra être pris. Vous connaissez Madame la Ministre MAM mobilisation sur ce jeu de sujet notre territoire audois ayant été impactés par des pollutions minières historique des enfants y ont été exposés donc réitéré que nous ne pouvons. Abandonner nos territoires ultramarins, des mesures doivent voter être prise en urgence et elles doivent être Madame Lim, la ministre à la hauteur de ces enjeux. Merci cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Le débat actuel témoigne de l'importance de chaque politique publique au quotidien et aujourd'hui donc, celle de la gestion des déchets et plus particulièrement en outre-mer. Les conclusions du rapport d'information sur le sujet présenté en fin d'année dernière sont alarmantes. Cela a été dit. Il est urgent d'agir des territoires et des populations en dépendent. je remercie d'ailleurs ici. Toutes les personnes qui ont contribué à enrichir cette réflexion afin que l'on puisse débattre aujourd'hui. Les outre-mer souffrent d'un retard majeur concernant la politique de gestion des déchets, ce sont des territoires dans lesquels la sonnette d'alarme est tirée, concernant l'urgence sanitaire et environnemental. Qui sont donc les problématiques que nous avons ça. Ici. Les chiffres d'ailleurs évoque cette réalité, le taux d'enfouissement moyen des déchets ménagers de 67% contre 15% au niveau national, au niveau. Du territoire national. Le coût de gestion moyen des déchets ménagers et 1,7 fois plus élevé que dans l'Hexagone, la quantité moyenne d'emménager d'emballages ménagers collectés par habitant et par an, et du 14 kilos. Dans les territoires d'outre-mer quand elle est de un peu plus de 51 kilos pour la France entière. Les Outre-mer souffre donc d'un retard en terme d'équipements pour assurer pleinement les missions de service public auprès de ses habitants. Le nombre de déchetterie par habitant et de à neuf fois plus faible dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole. Dans un contexte de crise sociale à Mayotte comme en Guyane. C'est non action si l'on peut dire concernant la santé et l'environnement le permettent au climat de s'apaiser, au contraire ça devient aussi une source de profond mécontentement. Des plans de rattrapage exceptionnel pour la Guyane et Mayotte sont évoqués dans ce rapport. Il nous semble pertinent et je dirai même indispensables pour rattraper ce retard accru. Il n'y a ni recyclage ni filière Didier pour faire mettre en place une économie circulaire réalistes et adaptées qui répondent aux besoins local. D'Éric correspondent aux réalités locales, D'importants gisements de déchets, dont ceux des quartiers informels des dépôts sauvages et des des et, des décharges illégales échappe à la collecte 41% de la population de Mamoudzou chef- lieu de Mayotte n'en bénéficient pas. L'urgence sanitaire et environnemental est déclaré. Il est donc urgent d'agir. Ces dépôts ont des conséquences sur ces territoires fragilisés puisque beaucoup de population n'ont pas accès à l'eau potable. Ainsi, certaines maladies sont favorisés par cette non politiques surtout en Mayotte et en Guyane, la dingue ni l'hépatite A la typhoïde autant de pathologies qui ont été rappelés ici évidemment. Les coûts environnementaux sont énormes, les sols sont pollués. Ils ne permettent plus à la faune et à la fleur d'outre-mer de s'épanouir dans un milieu sain et propice à ceux-là, sachant que les outre-mer abrite quand même 80% de la biodiversité française. Madame la Ministre vous l'aurez compris. Les financements sont insuffisants en tout cas pas à la hauteur des enjeux. Les propositions d'ailleurs du projet de loi de finances 2023 était encore faible face aux enjeux que j'ai essayé de rappeler rapidement ici. Et les taxes ne peuvent pas être la solution à tous les maux. Il nous faut donc du concret pour accompagner les élus, la santé des habitants en dépend. La prévention et la pédagogie autour de ces sujets sont inexistantes. Il faut donner les moyens humains et financiers afin d'agir pour montrer d'importance au quotidien de ces petites actions, pour un meilleur cadre de vie. Tout le monde doit prendre ses responsabilités bien entendu. Une réelle gouvernance sur le sujet semble indispensable des moyens à la hauteur des besoins sont nécessaires des pénalités pour celles et ceux qui ne respectent pas cela et je pense surtout aux éco-organismes. Ce qui me paraît assez primordial. Dans un contexte de réchauffement climatique et de crises environnementales. Nos priorités sont donc clairs, nos actions doivent répondre aux enjeux de développement durable pour nous et surtout pour les générations futures. Des Outre-mer donc accuse un retard majeur en matière de gestion des déchets. La cote d'alerte est souvent dépassé dans certains territoires, il y a donc un effort particulier à accomplir pour que l'égalité républicaine devienne une réalité là. Où on en a le plus besoin. Merci de votre attention. Merci cher collègue. La parole est maintenant madame Lana Teto toi nuit pour le groupe Union centriste pour huit minutes.

Monsieur le Président Madame. La Ministre Monsieur. Président à la délégation des outre-. Mes chers collègues. Après plus de six mois de travaux engagés par la délégation sénatoriale aux outre-mer le constat général est hélas alarmant. Et plus particulièrement dans des départements qu'il convient de placer en situation d'urgence sanitaire et environnemental mais d'une manière générale les Outre-mer accusent des lacunes et des retards majeurs on maintien de gestion des déchets ou plus de 67% de ces derniers sont enfuis et seulement 15% valoriser ces indicateurs sont différents selon chaque territoire d'outre-, mer. Mais ces ratios dans interpellé en comparaison aux données de l'Hexagone, où seulement 15% des déchets sont enfouis. Certes. Certaines collectivités ultramarines sont bien plus avancés lié à la dynamique des politiques Zambie dans nos mental. Localement, avec des moyens conséquents déployés en matière de sensibilisation au tri et augmenter d'investissements structurants pour geler la filière Ultramarins on connaît parfaitement nos défis liés à l'insularité, à l'absence de foncier à l'éloignement au coût du transport et à la nécessité de préserver notre biodiversité qui le président de la richesse de nos îles sur laquelle nos activités principales économique de développement repose. Mais ces défis nécessitent chaque jour de nouveaux moyens budgétaires car la vague de déchets ne cesse d'augmenter et les ambitions les incitations à la voir l'organisation de nos déchets comme le développement d'une économie circulaire sont encore à déployer plus qu'ailleurs pour la pour inventions de notre environnement. Une véritable. Une véritable politique de conduite de changement de nos comportements éteint insuffler dans nos îles et à produire autrement, d'une manière générale car. Dans les outre-mers le danger sanitaire et environnemental. Hé bien omniprésent avec le constat de décharges illégales et de dépôt sauvage qui échappe à la collecte. Le rapport de noms de collègues sénatrice Madame Gisèle Jourda et Madame Viviane Malet que le groupe centriste. Tiens à saluer pour cet énorme travail non mais face à la réalité de ce constat inquiétant. De la collecte et du traitement des déchets dans nos territoires ultramarins qui contribue aux crises sanitaires et environnementales qu'ils connaissent. Lorsqu'on prend connaissance des cas de leptospirose transmise par l'Iran en outre-mer est con Guyane et à Mayotte. Il est notamment 70 fois supérieur au taux national, il y a bien urgence de rattrapage massif et de mise en place de politiques volontaristes et durable pour ces territoires, les enjeux de santé publique sont énormes. Et outre cet aspect sanitaire le flux croissant des déchets défigure les paysages et détruit la biodiversité et que dire de l'état de nos océans, qui sont aujourd'hui de véritables poubelles de la pollution plastique à à l'aube du sommet des membres de l'ONU à Paris. Il est du genre de travailler tous ensemble pour générer une économie moins polluantes. On ne doit pas négliger la préservation de notre environnement. Sans oublier que nos Outre-mer constituent 80% de la biodiversité française aussi selon le prendre les différents constats de mes collègues sur la gestion des déchets dans les différents territoires je souscris entièrement aux préconisations du rapport sénatorial et à la proposition de résolution européenne déposée par mes deux collègues sur le sujet. Un appel à la solidarité nationale pour les financements d'investissements structurants et durables pour faire face à cette situation d'urgence la nécessité de mobiliser les aides européennes d'adapter la politique européenne en matière de gestion des déchets aux spécificités des rues et des. et de simplification de procédure européenne notamment en matière d'export des déchets. Permettent de développer la conclusion d'accord les journaux dans la zone relevant de chaque territoire d'outre-, mer. En dernier lieu, permettez-moi de parler de ma collectivité ou la charge de la collecte des du traitement des ordures ménagères et des déchets végétaux revient aux communes depuis 2004 un éminent sénateur avait déposé un amendement. À cette époque-là, je ne citerai pas de noms. Et communes qui ne sont, et qui ne seront pas en mesure, faute de moyens de financement et d'ingénierie de respecter le délai imparti que leur incombe pour assumer complètement cette charge au 31 décembre 2024. Une demande récurrente d'évaluation des charges à sans cesse été sollicité pour la mise en oeuvre de ces nouvelles compétences environnementales mais qui n'a pas abouti à ce jour-là, puis de l'État à la réalisation d'une étude globale en la matière est primordiale est fortement attendu pour conclu. Plaidant pour une économie moins polluante à l'échelon international et espérons que toutes de nos décharges à ciel ouvert sont définitivement condamné. Dans l'ensemble des outre-mer pour la préservation de notre biodiversité et de notre santé publique avec l'aide de l'État et de Merci de votre attention. Monsieur le. Le président, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je me félicite que le Sénat organise ce débat sur la gestion des déchets en outre-mer faisant suite au au rapport de nos collègues Gisèle Jourda et Viviane Malet que je tiens sincèrement à saluer pour leur engagement dans ce dossier et que j'ai mesuré en particulier. Sur le terrain lors de leurs déplacements à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment la gestion des déchets, comme la gestion de l'eau et l'assainissement est un mensonge, c'est un marqueur fort. Pour nos concitoyens de la réussite ou l'échec de nos politiques publiques ce dossier nous oblige tous. Collectivement, il serait évidemment aisés, voire caricaturale de s'en tenir au constat rappelé par les précédents orateurs. La situation de nos territoires et ça a été dit connaît des stades d'avancer différentes. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon ce soir que je vais vous parler car l'enjeu de notre débat c'est aussi d'ouvrir des perspectives de progrès avant tout les deux communes gèrent la collecte et le traitement des déchets ménagers mais également de tous les autres déchets, compte tenu de la la fête implantation des éco-organismes sur mon territoire et de l'absence notamment d'opérateurs privés susceptibles de traiter les déchets des entreprises de tous les secteurs, y compris ceux du BTP. Cette situation n'est pas une nouvelle évidemment, mais il n'est pas durablement tenable. D'autant que la partie non valorisés et ça a été dit par Gisèle Jourda et brûlés à ciel ouvert. Nous rapporteurs ont mesuré je pense pouvoir le dire le désarroi des maire de la commune de Saint Pierre et demi quand Langlade comme s'ils étaient arrivés au bout de leur capacité à tout absorbé finalement sur les sites des décharges la collecte des déchets ménagers et parfaitement assumée et obtient des résultats remarquables en matière de prévention et de tri pour les biodéchets des particuliers alors que l'obligation nationale entrera en vigueur en 2024, l'archipel a déjà franchi le pas dès 2018 et je pense qu'il faut le saluer. Des alternatives à la situation actuelle existe mais elle nécessite l'engagement de tous les acteurs. Je salue l'approche pragmatique du ministre-Carenco qui a pu mesurer l'ampleur de nos défis lors de sa visite début je souhaite mettre en évidence quelques pistes qui mérite me semble-t-il d'être creusé pour l'archipel en 1er lieu il existe un plan national de résorption des décharges littoral présentant des risques de relargage de déchets en mer. Alors si certaines communes ultramarines ont été retenus et je m'en félicite. J'avoue ne pas comprendre pourquoi les décharges de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas été intégré dans ce dispositif, car c'est justement parce que la décharge de Saint-Pierre Pierre déborde sur le domaine public maritime avec des rejets en mer à par forte tempête comme l'a rappelé Gisèle Jourda que le maire de Saint-Pierre Pierre se retrouve aujourd'hui sous le coup d'une enquête judiciaire après le signalement de l'OFEV. Je demande donc à l'État au-delà d'obstacle juridique peut être sera levé sur ce dossier que les décharges littoral de l'archipel face d'abord l'objet d'un diagnostic du BRGM pour qu'ensuite un accompagnement des mairies au titre du plan national puisse être mis en place. On second lieu nous décharge ayant toute accepté par la force des choses, elle se retrouve ceinturés comme dans beaucoup d'endroits de véhicules hors d'usage d'accumulateurs de pneus et me faisons ici le relais des 2 mairies et la volonté affichée par le ministre délégué, nous souhaitons qu'une opération d'enlèvement de ce stock historique puisse être coordonné avec le soutien de l'État. Au-delà du constat partagé, il est urgent d'accompagner nos élus sur cette opération. En 3ème lieu, ça a été dit précédemment, l'intervention des éco-organismes doit être plus active depuis la création des filières REP. Si la loi s'applique en outre-mer il faut quand même constater que les filières ont beaucoup délaissé les Outre-mer est loin de stigmatiser qui que ce soit. Je le gouvernement a a réuni les éco-organismes pour les mettre face à leurs responsabilités et a demandé une feuille de route territorialisée peut être Madame la Ministre que vous auriez des éléments sur cet aspect des choses à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a un consensus sur la nécessité de mettre en place progressivement une plateforme inter-rep avec un représentant local désigné et dédié à ces opérations. Le déplacement des éco-organismes sur place en septembre prochain et la structuration de nouvelles filières REP devra permettre d'accélérer les réponses. Il faudra sans doute un cahier des charges propre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et des mécanismes de pénalités. Ça a été dit d'ailleurs pour les autres Outre-mer lorsque les objectifs des éco-organismes ne sont pas atteints. Il est nécessaire que l'État accompagne. Et la forme reste à déterminer évidemment la mairie de Saint-Pierre pour qu'elle se dote d'un incinérateur de petite capacité pour que cesse le brûlage à ciel ouvert en mutualisant évidemment le flux des deux îles puisque la mairie ne peut pas porter seule cette ambition, je tiens à rappeler qu'en 2014. Par Karine Claireaux. La commune de Saint Pierre a obtenu le Label 0 déchet 0 gaspillage entre 2015 et 2020, il faut le dire. La quantité de déchets ménagers non valorisables mis en décharge a été divisé par 5 Saint-Pierre-et-Miquelon et Miquelon est sans doute l'un des territoires ultramarins sur lequel les efforts de prévention et de communication et de réduction ont été le plus fort au coeur de la stratégie de gestion des déchets, le maire actuel il Yannick Cambray, poursuit ce travail avec ses équipes et s'investit pour tendre vers une gestion conforme de nos déchets ménagers ont lien avec la municipalité de migrants non lad qui disposent de capacités réduites. Les autres acteurs et je le dis solennellement devront également prendre leurs responsabilités sur leurs propres déchets sans doute cela nécessitera-t-il un accompagnement Madame la Ministre comme les élus de l'archipel. J'en appelle à l'accompagnement et un suivi étroit de l'État dans la mise en oeuvre d'une gestion des déchets vertueuse assumée par tous les acteurs responsables au regard de la loi. Très bien monsieur le président. La parole est enfin dernière oratrice dans la discussion générale à mardi. Marta de Cidrac pour le groupe Les Républicains. Pour sept minutes. Je Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Dans une France riche de la diversité de ses territoires nos outre-mer ont toujours eu une place à part leur spécificité souvent entendu mais parfois incomprise donne à cette c'est space une singularité à nul autre pareil. Dans de nombreux domaines cela de fortes conséquences sur les politiques à conduire éloignement géographique différences climatiques spécificité insulaire nos outre-mer demandent aux décideurs publics et aux législateurs que nous sommes un effort permanent de contextualisation de différenciation et d'attention aux problématiques de ces territoires. Ce débat est une excellente opportunité d'en prendre conscience, au moment où s'ouvre à Paris le 2ème la 2ème phase de négociations internationales contre la pollution plastique mais surtout à travers le prisme environnementale du traitement des déchets. À ce titre je remercie la délégation aux outre-mer du Sénat de l'avoir impulsé et salue au passage le rapport d'information qui a été déjà cité sur la gestion des déchets en outre-mer de nos collègues Gisèle Jourda et Viviane Malet. Un bref rappel géographique à des milliers de kilomètres, au milieu d'immenses océans. Il s'agit de territoires souvent de faible superficie mais qui confère à notre pays par leur implantation dans tous les océans, le 2ème domaine maritime Avec pareil à tous nous incombe aussi une responsabilité mondiale en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Par ailleurs, nous l'oublions pas, il s'agit aussi de l'Union européenne à travers leur statut de région ultrapériphérique les Outre-mer française permet à l'Union européenne d'être présente en dehors du continent européen, et dans tous les océans, là encore c'est un atout pour l'Union européenne mais qui demande en retour de prendre en compte la spécificité ultramarine française. Ce cadre français européen est essentielle pour comprendre la politique de traitement des déchets ultramarins un domaine. Ou les atouts de l'outre-mer s'accompagne de responsabilités et de contrainte spécifique dans le cadre de l'évaluation de la loi j'ai que j'ai rencontré les différentes parties prenantes du traitement des déchets ultramarins qu'il s'agisse des élus locaux ou de professionnels du secteur. Tous m'ont fait part de problématiques ultramarines bien spécifiques, parfois très différentes de celles rencontrées dans l'Hexagone 2ème espace maritime mondial. La France concentre à elle seule dans ces ou 10 pour % des récifs coralliens 20% des atolls de de la planète et près de 10% de la diversité mondiale des espèces marines, notre responsabilité à l'échelle mondiale et donc de laisser à nos enfants des espaces maritimes non pollué vierge de déchets qui mettrait en péril des écosystèmes déjà fragilisé. En effet, à l'exception de la Guyane outre-mer sont des écosystèmes insulaires. Ils sont donc plus sensibles à la pollution et se régénère beaucoup moins rapidement. Les risques encourus ne sont pas que sanitaires. Ils sont aussi sociaux et économiques lorsque des Terres arables deviennent impropres à la culture ou que la qualité de l'eau se dégrade. Ce sont des ressources qui disparaissent ou qui demande à être importe. Un exemple concret de pollution dont s'alarment les acteurs locaux, cela a déjà été rappelé à maintes reprises à l'occasion de différents échanges l'accumulation de déchets issus de l'industrie automobile. vous serez tous frappés mais je pense que vous le savez, chers collègues, les nombreuses carcasses de voitures qui parsèment parfois nos il faute d'installations capable de pouvoir les traiter. Dans l'Hexagone mais donc plus encore dans nos outre-, un mauvais traitement des déchets, on porte de grandes conséquences. Il faudra être capable de l'anticiper, face aux défis de demain. Quid de l'augmentation du nombre de véhicules électriques en outre-mer et du traitement de leur batterie. Alors même que le traitement des véhicules thermiques fait défaut. Quid des modes de consommation de nos concitoyens qui évolue vers le toujours plus face choc par exemple pour ne citer que ceux-là au ou objet technologique à fort potentiel polluant tout cela au risque de voir les déchets saturée et polluer nos territoires ultramarins faute d'exutoire et de traitements performants. Au niveau local des pistes d'améliorations claires ont été identifiées par mes collègues de la délégation aux outre-mer les sous que les solutions nationales ne sont pas les seuls attendu de nombreux acteurs locaux considèrent être entravée par la réglementation européenne qui s'imposent à eux en tant que En effet, le règlement européen sur les transferts de déchets dits RTD pose de réelles difficultés dans nos départements et territoires d'outre-mer qui ne peuvent exporter leurs déchets dangereux vers les ports des pays tiers à proximité géographique. Selon le RTD ses exportations devrait se faire exclusivement vers l'Union européenne, mais cette solution ne paraît ni raisonnable ni viable, d'un point de vue environnemental et économique. À contrario, certains ports de pays tiers disposerait pourtant d'infrastructures qui permettrait de les traiter, ou à défaut de leur permettre simplement de transiter ce que le RTD ne facilite pas non plus Madame la Ministre. En principe ce règlement met en oeuvre dans le droit de l'Union européenne, les dispositions de la Convention de Bâle et de la décision de l'OCDE en matière de transfert de déchets dangereux dans les faits, il est bien plus strict que le droit international. Je sais Madame la Ministre que ce règlement est en cours d'examen et de révision à Bruxelles nos territoires ultramarins compte sur votre voix afin que leurs spécificités soient prises en compte dans ce futur texte. Il y a de ça quelques mois j'interrogé le ministre des Outre-mer d'ailleurs qui reconnaissait l'importance des enjeux que cela pose. La France est le seul pays de l'Union européenne à compter autant de rue aussi éloigné du continent européen, c'est un atout national et communautaire à valoriser et non à pénaliser. Le droit européen devra assurément évoluer vers une plus grande souplesse, si nous ne voulons pas aujourd'hui préparé les bombes à retardement écologique de demain. Au niveau national. Les travaux de notre délégation sénatoriale ont identifié des axes de progression clair simplifier la gouvernance améliorer le financement de la gestion des déchets insiste inciter les filières REP à une obligation de résultat aller chercher de nouveaux gisements de déchets et développer l'économie circulaire, ces dispositions sont déjà à l'oeuvre dans l'Hexagone et figure dans la loi Hajek déployons les beaucoup plus amplement dans les outre-mer de manière à ce que nous arrivions à des résultats efficient leur application doit aller de Pair avec une négociation sur la question des rues qui respectent nos concitoyens ultramarins ainsi que la définition d'une véritable stratégie maritime qui protège les écosystèmes de nos territoires ultramarins. Je vous remercie. Merci cher collègue magnifique. La parole est maintenant Madame Dominique Faure Ministre délégué chargé des collectivités territoriales la ruralité pour cinq minutes si vous faites six. On ne dira rien. Merci Monsieur le Président pour votre bienveillance. Monsieur le président. Mesdames. Les le rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs. Vous comprenez bien que je tiens tout d'abord à. Remercier la délégation aux outre-mer d'avoir organisé ce débat qui permet de faire un point sur les avancées en matière de gestion des déchets en outre-mer je souhaite remercier les sénatrices Gisèle Jourda et Viviane Malet pour leur rapport qui, je le souhaite inspirera les actions du gouvernement en la matière Après vous avoir chaleureusement remercié de façon sincère, je tiens à excuser l'absence du ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco qui actuellement en Nouvelle-Calédonie avec le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Il a fait de la gestion des déchets, l'une de ses priorités et il aurait aimé être à mes côtés. Voir ici à ma place pour pouvoir intervenir. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. La situation des déchets d'outre-mer n'est pas satisfaisante. Oui le constat, madame la sénatrice est alarmant. Mais le but, monsieur le président. Comme vous l'avez dit, c'est d'ouvrir des perspectives de progrès et des perspectives concrètes. Alors la situation des déchets ses 67% des déchets ménagers. Certains d'entre vous l'ont dit qu'ils sont enfouis, contre 15% à l'échelle nationale, c'est la gestion des déchets ménagers qui coûte en moyenne 1,7 1,7 fois plus cher et pour illustrer avec les déchets d'emballages trois à quatre fois moins de ces déchets qui sont collectés par le bac jaune. Votre rapport de décembre dernier a dressé un état des lieux exhaustif des difficultés elles sont multiples, des coûts plus élevés, l'absence de marché des exportations compliqué. Par ailleurs, le nombre de déchetterie est insuffisant et Les Échos organismes des filières REP reste trop peu mobilisés sur ces territoires. Cette gestion des conséquences sanitaires et environnementales, sociales, économiques néfastes. Vous l'avez tous dit pour nos compatriotes ultramarins et pour la biodiversité. En effet les dépôts sauvages polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques. Favorise la prolifération de rongeurs ou de moustiques transmettant la dengue et le paludisme. La loi de 2020 et la loi climat et résilience de 2021 ont fixé des objectifs ambitieux qu'il convient de mettre en oeuvre dans tous les territoires, les retards pris dans les Outre-mer nécessite de redoubler d'efforts et d'apporter une réponse à nos compatriotes ultramarins qui ont pu avoir un sentiment d'abandon. Le gouvernement, on est donc non seulement pleinement conscient mais surtout entièrement mobilisé, le gouvernement prépare ainsi un plan d'actions concret et territorialisée. Avec une feuille de route interministérielle. Avec une feuille de route interministérielle de progrès pour la gestion des déchets outre-mer ce projet de feuille de route repart des recommandations de votre excellent rapport de décembre dernier tient compte des retours d'expérience des préfets et de l'Ademe sur les territoires d'outre-mer vous l'évoquiez dans votre rapport, le premier à l'amélioration et la gouvernance. Un gros travail de rationalisation va être fait par les collectivités, les collectivités sont en effet compétente en matière de planification et d'organisation de la gestion des déchets, l'État se tient à leurs côtés comme nous le faisons actuellement avec le SMT VD en Martinique. À ce jour, la Réunion, Saint Martin Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon doivent encore adopter leurs plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Le prochain comité interministériel outre-mer le CIOM que vous avez cité. Nombre d'entre vous qui est programmé le 12 juin à 15h, sera l'occasion d'aller plus loin et de reprendre directement certaines mesures de votre rapport pour mieux organiser encore cette gestion. J'en cite au moins deux pour être concrète l'autorité unique comme la gratification du geste de tri mais vous travaillerez le 12 juin sur beaucoup d'autres en matière de financement. L'État est au rendez-vous il est via les contrats de convergence et de transformation les CCT dont la nouvelle génération est en cours de négociation pour rappel sur la période 2019 2022, le ministère des Outre-mer à contractualiser avec l'Adem. Un montant total de 41 millions d'euros pour accompagner les collectivités. Malheureusement ces montants comme souvent en outre-mer ne sont pas assez consommer. Aussi, rien ne sert de voter des Budgets mirobolants. S'ils ne sont pas dépensés. Le gouvernement travaille dans le cadre du siom à mettre à disposition des collectivités territoriales de l'expertise en ingénierie pour que les crédits proposés par le gouvernement et voté par le Parlement parviennent réellement à financer des projets. En complément, le fonds exceptionnel d'investissement peut apporter une aide ponctuelle pour certains projets ciblés le FEI depuis 2010, le ministère des Outre-mer à financer des projets de gestion et de valorisation des déchets à hauteur de 31,2 millions d'euros, soit environ 2, 6 millions d'euros par an pour 2023. Mon collègue Jean-François Carenco, a décidé de doubler cette enveloppe et de le conserver, centré sur la Guyane, qui en a fait sa priorité. Le Fonds Vert lui-même est également un outil dont les collectivités ultramarines doivent se saisir la collectivité de biodéchets représentent déjà 10% des dossiers déposés lors du premier appel à projets ainsi 870.000 euros seront alloués à la Martinique pour des travaux de mise en oeuvre du captage de biogaz. Des études seront également financées pour la mise en oeuvre du tri à la source des biodéchets à Marie-Galante et pour l'élimination des déchets métalliques du lagon à la Réunion. Enfin, les fonds européens sont des atouts précieux pour les collectivités pour la période 2014 2020, c'est 155 millions d'euros qui ont été engagées en faveur de la gestion d'été des déchets en outre- mer. J'en profite pour vous dire la commissaire que je connais bien Élisa Ferreira qui, qui est la commissaire sur les fonds européens. La politique de cohésion, elle. J'interpelle. J'ai mon collègue Jean-François Carenco, et elle m'interpelle régulièrement sur ces sujets et elle est triste de voir à quel point on n'arrive pas à consommer. Ces millions d'euros qui nous viennent de l'Europe 155 millions d'euros engagés en faveur de la gestion des déchets en outre-mer comme je l'évoquais précédemment les collectivités régionales doivent encore mieux se saisir de ces aux pertes unités de financement améliorer la consommation des fonds. Un autre constat que le gouvernement partage c'est que les éco-organismes des filières REP ne sont pas au rendez-vous en outre-mer ce n'est pas normal que les ultramarins ne puissent pas bénéficier d'un service de collecte performant pour les déchets relevant de ces filières REP la loi Hajek a justement prévu de remobiliser ses éco-organismes pour rattraper d'ici 3 ans, les retards en matière de collecte et de traitement des déchets en outre-mer.

Et c'est pas un droit acquis. Ça je le sais, vous avez raison. Je conclus brièvement je souhaiterais aborder un dernier point dans votre rapport, s'est largement fait l'écho, c'est le transfert de déchets, soit des Outre-mer vers l'Hexagone, soit entre les différences d'outre-mer les autorités françaises sont pleinement mobilisées dans le cas de la révision actuelle du règlement européen sur le sujet pour que les conditions de transit vers l'Union européenne soit facilité lors de la récente conférence de coopération régionale Antilles Guyane la problématique des déchets a fait l'objet de débats spécifique et une réflexion est en cours pour mutualiser optimisée et mieux coopérer sur la question. Je tiens encore une fois à vous remercier pour la qualité de vos travaux et la richesse de vos propositions. avec Jean-François Carenco avec Bérangère Couillard ce le prochain comité interministériel outre-mer pour améliorer encore la gestion des déchets outre-mer notre ambition commune et que ces déchets ne soient plus des encombrants enfouir mais bien des ressources à exploiter en outre-mer comme dans l'Hexagone. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Mes chers collègues, vous allez comprendre ma générosité qui n'a en rien naturel c'est que, en accord avec l'ensemble des groupes politiques et le gouvernement. Je vous propose de prendre l'examen de la proposition de résolution proposant au gouvernement de renforcer l'accès au service public. À 19h 15 à l'issue de ce débat et comme le Ministre des la à 19h 15 j'avais un petit peu de marge pour le gouvernement, donc Madame la Ministre vous avez profité de ce décalage par rapport à monsieur Guérini. Je donne la parole tout de suite au président de la délégation monsieur Artano. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Je serais presque tenté. Monsieur le Président de demander également un rab de nature républicaine. Je tiens tout d'abord vous remercier Madame la Ministre pour votre participation à ce débat en séance avec l'absence signalée du Ministre délégué une qu'on la comprenons parfaitement. C'est un sujet évidemment fondamental mais complexe en raison des réalités de chacun de nos territoires. Vous l'aurez compris, nos délégations. Attendent des réponses claires et vous avez apporté un certain nombre d'éléments 26 recommandations dans ce rapport sont sur la table et et le gouvernement doit son sévir mais pas que son Dans tous les cas sont les assurés sur le fait que notre délégation on fera un suivi évidemment précis et exigeant au cours des prochains mois sans aucun esprit partisan, c'est ce qui nous caractérise. En effet, ce débat intervient à un moment clé, puisque vous l'avez indiqué le siom se tiendra le 12 juin prochain avec, nous l'espérons évidemment un volet. Déchets qui nous paraît incontournable et prioritaire vos propos ainsi que certaines déclarations récentes du gouvernement, ce sont des premiers signaux positifs, il faut désormais évidemment concrétisée par des actes s'agissant notamment de l'action des éco- éco-organismes que vous avez rappelé notre délégation a noté attentivement que vos collègues Bérangère Couillard et en pensant qu'un coup avait réuni comme je l'ai dit tout à l'heure conjointement le 6 avril dernier, les éco-organismes pour leur demander, je cite, de se mettre à niveau avant la fin de l'été. Dans un communiqué conjoint, les 2 ministres, s'appuyer sur le rapport de la délégation. Espérons que cette délégation cette déclaration occurrence. Sera un électrochoc à défaut je vous invite évidemment à engager le mécanisme de pénalités suggérés par nos rapporteurs dans le rapport et à abaisser les seuils de responsabilités, conformément aux recommandations. Agir vite et fort pour reprendre les mots de Gisèle Jourda est un impératif. Car le sujet des déchets est symptomatique des défis à relever pour nos outre-mer. Ont je environnementale enjeu sanitaire la gestion des déchets revêt un enjeu économique ça été rappelé par de Cidrac. Le développement touristique et donc la création de richesse ne peut réussir si les plages évidemment sont. Les routes bordées d'épaves et le paysage abîmer les déchets peuvent aussi être une opportunité pour rapatrier de la valeur ajoutée sur le territoire en développement des filières locales de recyclage quand cela est possible. Mais surtout pour les Outre-mer, les déchets sont l'autre services publics de base au coeur du quotidien de chacun au même titre que l'eau potable, l'assainissement, ou encore l'électricité sans lequel il n'y peut y avoir de développement harmonieux. Et digne. La crise de confiance qui s'est exprimé lors des dernières élections électorales. Échéances électorales dans les Outre-mer est notamment la conséquence des difficultés à fournir à nos concitoyens si servi que pour ces services pourtant essentiel du quotidien. Le récent rapport de la délégation sénatoriale sur l'avenir institutionnel outre-mer souligne d'ailleurs que la pertinence d'éventuelles évolutions institutionnelles doit être évaluée à l'aune de leur capacité à déployer des politiques publiques plus efficaces. La défiance et la crise démocratique ne seront surmontés que lorsque les résultats tangibles nous serons obtenus par ses services publics fondamentaux, un autre aspect transversal et celui de l'ingénierie, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, c'est-à-dire la capacité à transformer une idée en réalité. C'est le point faible des Outre-mer sur toutes les politiques publiques, là encore, le rapport fait quelques propositions, elles sont essentielles. Autant que celles relatives à l'effort financier qui n'est pas la seule donnée de cette équation ont enfin s'achèverait mon mon propos on pointant longe de la différenciation et la territorialisation notre délégation porte cette exigence sur tous les sujets ultramarins celui des déchets n'y échappe pas, vient de mal elle a évoqué notamment en mettant en avant la nécessité de développer la valorisation énergétique plus globalement il faut sans doute réinterroger sur nos petits territoires insulaires ou isolées, la hiérarchie des modes de traitement. Est-il par exemple toujours pertinent d'expédier à l'autre bout du monde. Des déchets plastiques ou de les recycler ou ne vaudrait pas mieux les valoriser localement pour produire de l'énergie. La valorisation matière doit être envisagée de manière pragmatique et réaliste. Et c'est au niveau de chaque territoire que la stratégie la plus fine sans idée préconçue doit être défini contractualiser j'ai bien noté Madame la Ministre que vous a appelé a volé appeler à une feuille de route territoriale. Et ça fait partie un peu de la méthode de gens a un coût, donc je me permets de le dire puisqu'il est absent mais ils ne m'ont. Vous ne m'en voudra guère. Je suis assez partisan pour que le gouvernement qui n'est pas seule responsable dans cette affaire, je le dis également les collectivités ont la responsabilité, les acteurs qui ne sont pas investis dans la gestion des déchets sont également. Responsables et le souhait c'est effectivement une contractualisation par territoire où tout le monde signera au bas de la page et tout le monde prendra ses responsabilités et je pense que c'est un cercle vertueux. Que j'appelle de mes voeux, à titre personnel mais je pense que beaucoup d'élus ici me rejoindront pour faire en sorte que. Nous soyons tous au rendez-vous de cette gestion vertueuse et pas seulement le gouvernement ou les éco-organismes ou les élus. C'est une responsabilité collective partagée et que nous devons impérativement contractualiser moi je suis partisan de cette contractualisation pour responsabiliser l'ensemble des acteurs, je vous remercie. Merci monsieur le président. Merci madame la ministre. Je vais suspendre cinq minutes, le temps de l'arrivée. De monsieur Guérini pour le texte suivant merci en tout cas, ce débat est terminé. Mais ils ne partaient pas tous

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution proposant au gouvernement de renforcer l'accès au service public. Présenté en application de l'article 34 à tirer 1 de la Constitution par monsieur Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues demande du groupe RDSE. Dans la discussion générale. La parole est au président requis et auteur de la proposition pour 10 minutes, monsieur le président. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre quotidien l'essor des plateformes téléphoniques a ses bons et ses mauvais côtés. Quand tout va bien peu les sièges public plutôt que patienter dans une interminable file d'attente est un une de temps surtout si on les géographiquement éloignés du du service Lequel entre nous n'a jamais connu, tapez 1. Tapez 2 tapez 3 avec au bout du compte de plus tôt au bout de la ligne un bip soit personne. Cette réalité a dit documenté par une récente enquête du magazine 70 millions de consommateurs. Réalisée en collaboration avec la défenseure des droits. Elle révèle les obstacles que rencontrent les usagers pour jouer nos services publics par téléphone. Les caisses, on lui par les enquêteurs ont montré que 42% des appels n'aboutissaient pas. Quand Russie c'est la durée d'attente ligne représente 9 minutes à moyen. moyen. Face à un manque de conseiller l'assurance maladie et le service plus critiqué. Pour la Caisse d'allocations familiales, près de la moitié des appels restent sans réponse car le conseiller en injoignable. Il rediriger l'usager vers Internet. Elles incertain qu'. On encore. Dans un monde n'pas fait la dématérialisation des démarches pour être la meilleure des solutions il six mois toutefois de conditions à avoir un minimum de compétences informatiques et un beau réseau malheureusement. Près de 14 millions de nos concitoyens sont frappés d'y être isthme comme vous l'avez souligné, notre ancien collègue du Gers Raymond Grall. Dans son rapport d'information illectronisme et inclusion numérique.

Il faudra faire davantage. Pour réduire le fossé entre les connecter et les non collecter. Proposition de résolution. Appelle notamment au développement d'une stratégie numérique inclusive. Tout au long du parcours scolaire de façon. Précoce. L'accès aux services publics dématérialisés c'est aussi bien entendu les question de réseau sur ce volet, nous sommes bien placés en particulier de l'été entre ruraux pour constater encore les difficultés de son déploiement dans certaines zones. Pourtant, mes chers collègues, c'est parce que les moyens pour se déplacer et communiquer sont mieux sous distincts en milieu rural que la téléphonie mobile et avec elle a Internet. Ils sont plus utiles qu'ailleurs, l'ancien sénateur de la Lozère Alain Bertrand la maîtresse justement. Relevé dans son rapport sur ce qu'il. L'hyper-ruralité. Garantir l'accès au numérique étonne de voir que nous rappelle aussi la déclaration européenne 10 26 janvier 2022 sur les droits et principes de Amérique en effet un de ses articles précise je cite que toute personne devrait avoir accès à des technologies qui vise à une alors à diviser la transformation numérique devrait contribuer. À l'équité sociale et économique dans l'Union. Certes l'étage, les opérateurs s'efforce de mieux prendre en compte la couverture des territoires ruraux à travers différents plans d'action mais ce mythe entre collègue chargé de la transition numérique. Elle était. Télécommunications Télécommunications Annick dernier devant la commission des affaires économiques du Sénat, il fallait trouver un accord entre l'État, les opérateurs et les collectivités pour relever les défis restant du grand chantier de la fibre et répartir l'effort financier de manière équitable et juste, on est bien d'accord. D'autant plus, comme l'a rappelé en décembre dernier notre collègue et rigole lors des questions d'actualité au gouvernement. Qu'il y a le défi qualitatif comme dit quantitative du déploiement du réseau, mais aussi celui de la qualité, le Renault Clio pour. Abandonné pose problème car il est mal entretenu, y compris dans les territoires qui n'ont pourtant pas la fibre et où les délais de dépendance sur le long. Attendant rideau actuel du nord du débit devrait être inférieure à celle fixée par l'Union européenne à l'horizon 2025. Aussi la numérisation ça public à marche forcée comme l'a qualifié le Secours populaire en 2021. À Robert et non des moindres, certains usagers renoncent à leur droit. Je citerai l'exemple souligné pour Assemblée des départements de France, qui a identifié cet hiver la sous-consommation du chèque carburant comme la conséquence de la fracture numérique face à tout cela. Il est donc fondamental que le contact humain reste possible. Là aussi, j'ai dit j'ai été pourraient être relativisée. Si dans le même temps l'État s'était pas déchargé du maintien de service publics de proximité. La dégradation continue des comptes publics. Depuis la fin des années sont Nice comme il y a une démographie défavorable dans certains communes ont en effet conduit à des réformes rationalisant Alexis le maillage territorial des services publics, comme vous le savez, sa collègue. C'est un vent toucher aussi bien les administrations de Sécurité sociale que les Henri et la Poste tout le territoire a été concernés y compris le tamarin pourtant mal lotis. Bien que dans son rapport sur l'accès aux services publics dans les territoires ruraux. La Cour des comptes, considère qu'il n'y a pas eu d'abandon. Les territoires ruraux par les grands réseaux nationaux de service public. Elle relève toutefois que le niveau d'implantation varie selon les réseaux considéré c'est vrai les schémas départementaux dans le Libération de la visibilité des services publics ont permis d'améliorer la situation ou de la contenir. Et bien sûr grâce à la mobilisation des collectivités locales, très impliquée dans le développement d'une offre de services publics mutualiser le pire a été évité. Je pense au réseau mais on fera le service et qui permet à l'effet de maintenir un accompagnement adapté aux besoins locaux. J'ajoute toutefois que moins d'un quart des services publics de des services de mes des maison France service pardon sont accessibles par le transport en commun et que, implantation et leur fonctionnement repose sur la bonne volonté et les moyens financiers des collectivités locales. Mon groupe souhaiterez, je le répète un partenariat plus équitable avec entre l'État et les collectivités locales car public demeure une composante essentielle de l'aménagement et l'attractivité des territoires. Même s'il faut le dire, quelques fois dans les communes des des des commerces fermés et les derniers qui reste c'est quelquefois service public. Mais j'ai un collègue le principe d'égalité des droits est au coeur du pacte républicain. Il est pas besoin de démontrer combien de nos concitoyens, ils sont sensibles. La disparition programmée du timbre rouge il distribuait ses sentiments. Alors que les Français sera de moins en moins dans les bureaux de poste ou pour y envoyer un courrier. Il supporte mal leur réagit à lire leurs. Organisation ce paradoxe s'explique simplement. La Poste bénéficie tout simplement de l'image mais très populaire du facteur non nos agit souvent connu de tous, ils représentent le principal ambassadeur du lien social. Ainsi que le gardien de la présence, le public de proximité si nécessaire à la cohésion.

Si. Merci monsieur le président. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à Monsieur Daniel Chassain pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'accession au service public est un combat que mène la République depuis sa naissance et la création des départements, chaque citoyen devait pouvoir rejoindre la préfecture est retourné chez lui en moins d'une journée à cheval. ce combat ne sera jamais définitivement achevé au contraire il doit sans cet être mené à mesure que les services publics se spécialise afin qu'il soit accessible à tous nos concitoyens. La proposition de résolution du président. Ruquier qui est un homme de grande expérience a été maire, conseiller départemental sénateur depuis longtemps va dans le bon sens. Souhaité par nos concitoyens l'accès numérique est certes un déficit de notre siècle. Il ne se substitue pas pour autant totalement à l'accès et à l'échange humain en face ou par téléphone comme ça vient d'être dit. Mais nous avons besoin d'autres services au public dans tous les milieux urbains péri-urbains et ruraux plus profond se pose les mêmes questions. La mobilité ferroviaire routière des services d'accès à la CAF, l'assurance maladie, les services de l'enfant du maintien des écoles de l'éducation inclusive. N'insuffisante de de. Avoir accès à la culture, au sport le téléphonie mobile, la formation, la sécurité, c'est ce que souhaitent nos concitoyens avec aussi l'accès aux services de santé plus de soignants en pas plus de soignants n'est pas aux médecins et aux infirmiers, très important pour le maintien à domicile avec l'Etihad. Les pharmacies qu'il faut. Valoriser le maintien des services hospitaliers en particulier les Les agents. De France service apport partout où ils existent un soutien très efficace pour aider les usagers il faut. Les développer cet investissement national est un renfort indispensable. À l'ensemble des actions mises en oeuvre par les élus locaux pour maintenir la population. L'accès aisé au service public est nécessaire. Par tous les modes possibles afin de correspondre aux besoins de nos concitoyens qui seront ainsi reconnue par la République apportant la confiance et l'adhésion pacte républicain. L'accès aisé aux services publics constituent également la condition essentielle de l'éviter des terrines attractivité des territoires. Et la stimulation de cercle vertueux qui amènera entreprises et population à s'installer. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, n'oublions pas le message des gilets jaunes qui était majoritairement issus des territoires victime de diverses désertification dont celle des services publics, travaillant à l'inverse à une répartition favorable aussi aux territoires ruraux des activités économiques et sociales qui doit pouvoir trouver aussi aisément que possible dans les services publics des partenaires pour leur réussite. C'est aussi je crois, le sens de cette résolution. J'y souscris. La création des espaces France-Serbie sous la désignation de sous-préfet à la relance, sont des mesures qui s'inscrivent dans cette vision, nous devons aussi réfléchir à la création de sous-préfets développeurs à la coordination de soutien nationaux, régionaux intercommunaux pour le financement d'atelier relais pour les TPE. À l'avenir de zones de revitalisation rurale, les femmes ZRR qui, contrairement à ce qui est dit sont peu coûteuses et efficaces. Monsieur le ministre, il faut les conserver mais aussi un aménagement fixe spécifique du Dusan pour les communes rurales qui ont peu construit la nécessité aussi de développer des services au public polyvalent et polymorphe afin de correspondre aux habitudes et aux spécificités locales aux côtés des buralistes historiquement les premiers préposé détaché de l'administration, les restaurants ruraux les épicerie multiservices sont des exemples qui peuvent devenir des lieux ressources aux côtés des services publics plus casse-, plus classique. Monsieur le Ministre donc. au président Roquier et au groupe RDSE, mes chers collègues, continuant à être imaginatifs et ambitieux pour que l'ensemble des services publics puissent accéder au service. Pour que l'ensemble des publics français puissent accéder aux services publics qu'mérite nous voterons bien sûr cette résolution. Merci cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Paul Toussaint Parigi pour le groupe écologiste pour cinq minutes.

Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues. La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui a le mérite de vouloir sanctifié et rappelé le rôle essentiel. Que jouent les services publics. Rappeler qui sont une condition indispensable de l'accès de tous. À leurs droits fondamentaux. Droit à la santé, au logement, à l'éducation à la justice à l'hébergement d'urgence. Qui sont l'expression concrète des principes que l'esprit républicain a progressivement pour ai affiné et légaliser. Pour étayer et garantir des droits et libertés. Qui sont le terreau de l'économie, le maillage des solidarités. Les ferments de notre citoyenneté tenu de garantir l'égalité des usagers d'assurer une continuité d'action et de l'adapter aux besoins de ceux-ci. Que face à ces impératifs. Nous avons tous le devoir vigilant d'analyser avec lucidité leurs forces, leurs faiblesses, et en conséquence leur impérieuse améliorations sont. Encore trop souvent les villes, les petites et moyennes villes ainsi que les métropoles domine les choix et représentations qui sont faits. Au cours de ces dernières années. Les vagues de réforme de l'action publique se sont traduites par la fermeture de nombreux services de proximité. Ce courant a laissé des pans entiers de territoires éloignés des grandes infrastructures numériques et de transport et aux habitants le sentiment d'être marginalisé abandonné élu d'un territoire majoritairement rural je sais combien l'égalité d'accès à ces derniers est encore loin d'être acquise et même bien des fois en décroissance je sais comme les réponses apportées ne tiennent pas compte des spécificités locales en Corse. Les communes rurales concentre la moitié de la population régionale, l'éloignement des pôles urbains se conjugue avec le relief montagneux de l'île à des temps de transport plus élevé que la métropole. Couplé à aux impacts encore très prégnantes de la fracture numérique qui jalonnent nos territoires de nombreuses zones blanches. Oui. L'Administration dématérialisée a hélas trop souvent été accompagnée de la fermeture de guichets de proximité et donc de la suppression de tout contact humain. Même si elle a constitué des avancées que l'on ne peut nier et elle a également été synonyme d'exclusion. Exclusive pour ceux à qui elle apparaît comme un obstacle parfois à surmontables les personnes âgées, les personnes handicapées celles en situation de précarité sociale alors que bien souvent, ce sont ces mêmes populations pour qui l'accès aux droits sociaux garantis par les services publics revêt un caractère vital. Notre vision du progrès n'est pas conciliable avec l'éloignement des usagers de leurs droits, avec le renforcement de la fracture territoriale. L'épisode de 2018 nous la rappeler haut et fort. Si le rapport du CEC et la mise en place de l'agenda rural remplace le le devant de la scène des problématiques du monde rural. Si à cor et à cri ces derniers commencent à mieux être pris en compte. Il y a pas encore aujourd'hui la coupe aux lèvres. Les territoires ruraux qui recouvre des réalités très différentes continuent de souffrir de réponse mal adaptés à leurs spécificités. Alors qu'un accès égalitaire reste un rouage essentiel du pacte républicain. Si l'augmentation des maison France Service doit se conjuguer à une montée en gamme de leur qualité. Il faut davantage associer les élus locaux qui connaissent parfaitement les territoires et leurs besoins. Ce dont il est question ici, c'est de la justice territoriale pour éviter les exclusions. Il nous faut construire un capital collectif accessible à Toulouse. Nous pensons qu'il repose sur une couverture numérique pleine et entière et sur la recherche d'un meilleur équilibre entre l'accompagnement plus attentif des personnes à l'accès à l'accès mais des matérialisé mais aussi sur la mise en place des réels services de proximité. Améliorer leur fonctionnement simplifié leurs procédures sont des nécessités d'autant plus impérieuse que le service ne sont pas des simples acteurs économiques ou sociaux, ils sont les garants de la cohésion sociale et les symboles de l'action publique. Je voulais remercier mon collègue. Le président Jean-Claude Requier pour cette proposition de résolution en espérant que le plan France ruralité dévoilé il y a peu permettent de tenir ce pari de taille. Les attentes sont fortes et le moment crucial. Il ne faudrait pas que les nouvelles coupes budgétaires ne Vienne contrarier l'espoir de notre territoire. Je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président requiers. En saluant et en vous remerciant pour votre initiative. Mes chers collègues. Si vous souhaitez accéder à l'hôpital public taper hein si vous souhaitez effectuer un dépôt de plainte auprès d'un fonctionnaire de police taper enfin si vous souhaitez obtenir un rendez vous pour demander un nouveau passeport ou une nouvelle carte d'identité nationale d'identité tapé Troie mais si vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller. Tapez dièse. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec l'État votre temps d'attente est estimé à. 35 heures. Trêve de plaisanterie, mes chers collègues du pourrions en rire mais bien qu'exagérée. Une telle introduction reflète parfois le 1er contact aride quand la plupart de nos concitoyens avec les multiples une plateforme d'accueil de nos services publics. L'accès de nos compatriotes au service public et pourtant essentielle essentielle pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans l'action publique essentiel aussi car aux yeux de beaucoup de Français, un service public de qualité requiert de la facilité en termes d'accès de l'efficacité en matière de solutions et de la rapidité s'agissant des délais de traitement. Le principe d'égalité d'accès aux services publics signifie que tous les usagers doivent être traités de manière équivalente. Je crois que le réseau des maison France services dont il faut saluer les résultats est une étape importante permettant d'atteindre ses objectifs et de retrouver une certaine proximité là où les Françaises et les Français les plus éloignés, se sentaient délaissés. Ce réseau qui compte désormais plus de 2500 structures labellisé répartis sur l'ensemble du territoire est un bel outil au service d'une proximité retrouvée mais il ne peut à lui seul résoudre la problématique pour laquelle nous sommes réunis. Force est de constater que l'accès au service public rencontre encore certains obstacles qui rendent la vie compliquée à tout le monde. Parmi ces freins figurent notamment l'accès au numérique et la et la complexité bureaucratique si singulière à notre pays en ce qui concerne l'accès au numérique. Il est essentiel de garantir un accueil équitable pour tous, la création des conseillers numériques et la pérennisation de leur financement est une avancée majeure et je salue Monsieur le Ministre, votre engagement particulier à ce sujet. Mais le service public ne ne doivent pas être limité à un nombre restreint de personnes ils doivent être ouvert à l'ensemble de la population. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures visant à réduire la fracture numérique il à fournir les outils les ressources nécessaires à tous les citoyens pour accéder aux services publics en ligne. Par ailleurs, la bureaucratie présente aujourd'hui un un problème structurel majeur au fil des décennies à la prospérer sans limite, devenant ainsi un obstacle au bon fonctionnement des services publics, les procédures administratives se sont alourdit considérablement les 100 lettre morte la nécessaire et attendu simplification Jérôme Fourquet disait récemment dans un numéro de L'Express. Ce que je disais, il faut qu'il y a au moins 15 cases à remplir sinon l'administration c'est un malaise cette caricature très juste nous invite à nous remettre en question. Il est essentiel de revoir en profondeur cette bureaucratie excessive et simplifier les procédures administratives de plus, il convient de souligner que l'inflation législative constitue un frein majeur à la simplification que nous appelons toutes et tous de nos voeux à l'occasion de nos diverses prises de parole à la tribune où je me trouve autant du point de vue des élus locaux que de nos concitoyens. Il est donc nécessaire d'entreprendre une réflexion approfondie sur cette inflation législative et d'adopter des mesures permettant de simplifier le cadre législatif et réglementaire pour faciliter le quotidien des usagers et des élus somme toute sans nous attaquer aux obstacles liés à l'accès au numérique à la bureaucratie excessive et à l'inflation législative, nous continuerons, nous continuerons d'aller dans le mur. Cela nécessite des efforts de simplification, de modernisation et d'adaptation aux besoins des citoyens afin de de rendre les services publics plus accessible, plus efficace et plus proche des attentes des Français bien évidemment notre groupe RDPI salue cette. Proposition de résolution et la vôtre. Je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il allait très loin le temps où le maillage des services publics dans notre pays était le moteur d'un développement équilibré du territoire faisant de la ruralité française, un modèle unique en Europe. Ce temps a été broyé par la succession d'objectifs d'économie sous couvert de modernisation de l'État qui ont favorisé un processus de concentration des services dans les épaule intermédiaire ou les grandes villes. Le souci de rationalisation de l'offre de réduction des coûts et la perte de proximité sont devenus la norme. L'exemple de la SNCF qui s'est concentrée au seul développement de la mobilité de métropole, la métropole en délaissant les autres lignes qualifiés de secondaires l'illustre parfaitement. On n'entretient plus une ligne le temps de parcours augmente les gens prennent la voiture enfin on ferme la vie faute de rentabilité. L'État n'a cessé de poursuivre cette logique de fermer une multitude de services, lui, que ce soit du côté des écoles, des hôpitaux, des maternités, des gares, des services de trésorerie des tribunaux de gendarmerie, j'en passe. J'en veux pour preuve dans la Nièvre, le département que je connais bien la grande faucheuse statistique fait sont neufs. Tous les jours sur notre territoire et apporte son lot d'annonces de fermetures de services. Ici la fermeture de classe ce postes en moins pour la rentrée 2023 2024 dans nos villages là des voies de chemin de fer mal entretenu, la multiplication des trains en retard, des gares et des guichets que l'on ferme là encore la fermeture des maternités de Clamecy de conne d'autant les suspensions des services d'urgence de Clamecy Decize le transfert du Centre U15 de Nevers à Dijon là aussi la fermeture de 11 trésoreries et si le sentiment d'abandon qui alimentent la colère de nos concitoyens provenaient en grande partie de la dépasse, disparition de nombreux services publics de proximité ou là de leur suppression annoncée à court terme. Face à la multiplication des déserts, que l'on connaît que connaît notre pays. Quelles réponses peut-on apporter dans tous ces territoires à faible densité habité par des publics souvent fragiles, précaires ou âgés qui reste en retrait des zones les mieux équipés en service. Comment continuer à fermer les yeux et laisser à l'écart de la société des individus peu con dictée victime de l'illectronisme vivant dans des territoires où la distance se calcule en temps de parcours et où la mobilité est rendue plus difficile. Comment ne pas comprendre alors ce sentiment d'abandon et allemand ressenti dès lors que la dimension sociale du service public disparaît. Élus, habitants, commerçants se rendent compte de la mort des directions départementales des services de l'État et de leur maillage local, ils se rendent compte que l'on les dessaisis de leur richesse l'que sont nos services publics nos habitants des villages ruraux sont non seulement attachés au lieu où il réside. Mais plus globalement ils ont à l'attachement affectif aux gens qui vivent à une identité. La défense des services publics et dans un tel contexte, le symbole d'une lutte pour le maintien d'une vie face à un déclin qui semblait inéluctable et qui in fine et induit lorsqu'ils disparaissent un triple choc psychologique économique, démographique. C'est pour quoi il est plus que nécessaire de s'interroger sur ce que coûte l'absence de ses services publics et sur ce qu'ils peuvent apporter en termes de cohésion sociale, d'accès au droit d'emploi, de lutte contre le réchauffement climatique mais également de développement économique de plus nos territoires sont désormais recherchés car oui, chers collègues, les différents recensements de population montre que nos territoires sont redevenus attractifs. Cela suppose aussi de requestionner. Le financement de nos services publics la filme ce glissement de l'impôt sur les re-plus riches a rendu à la fois. a perdu à la fois le sens de la contribution injuste et a appauvrit l'État donc les services publics. Or l'impôt est acceptée par tous, lorsqu'ils financent les services publics qui sont le Patrimoine de ceux qui n'en ont pas parce qu'ils permettent à chacun et chacune, quelles que soient ses moyens d'accéder aux services et réseaux indispensable à la vie humaine. Il est impératif de les financer à hauteur des besoins, c'est cette ambition d'un service public offrant des garanties collectives qui doit être au club, au coeur de la construction d'alternatives de progrès, l'innovation, l'appel aux bonnes volontés sont souvent insuffisants pour connecter ces individus et ces territoires on l'observe aisément aujourd'hui avec l'horizon des maison France Service qui constitue certes une avancée mais qui ne compense que partiellement un manque mais avec des différences constatées dans l'éventail des services accessibles et dans la densité de leur maillage territorial selon les départements, l'articulation avec nos collectivités locales, reste à renforcer, car je vous le rappelle nos mairies sont le premier niveau d'entrer dans nos institutions publiques et la première voie d'accès au service public. Pour conclure je crois profondément que la présence des services publics doit être pensé comme un investissement d'avenir. Ah, pardi. Sur les un Paris sur les générations à venir est un enjeu fort pour le devenir des territoires ruraux. C'est la raison pour laquelle nous voterons m'l'ensemble de mon groupe pour cette proposition de résolution dont je salue l'initiative de nos collègues du RDSE et en particulier de son président Jean-Claude Ruquier. Je vous remercie. Merci cher collègue. Là. La parole est maintenant madame Michelle Gréaume pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Qui pourrait s'opposer au renforcement de l'accès au services public. Et pourtant. L'examen des différents votes lors des précédents projets de loi de finances ici dans cet hémicycle comme à l'Assemblée Monde que la réponse ne va pas nécessairement D'où quelques interrogations sur les raisons réelles qui ont conduit au dépôt de cette proposition de résolution. Cependant, l'enjeu est certain en matière de cohésion sociale, d'accès au droit d'égalité territoriale et entre nous, concitoyens, notamment. Cette proposition de résolution le rappelle bien d'ailleurs. C'est la particularité de notre République depuis l'année de naissance de notre constitution d'avoir développé des services publics fort utiles à l'intérêt général à l'accès garanti pour chaque citoyen en tout point du territoire. Mais aujourd'hui, les temps sont durs, les enseignants désertent un Champ de ruines. Les hôpitaux ferme des lits à tour de bras les collectivités sont bien en peine à mettre en oeuvre des politiques publiques pourtant nécessaire finalement tous les secteurs public semblent concerner les gouvernements successifs ont veillé à saper un modèle que beaucoup nous envier pour céder l'école, l'hôpital, les transports et j'en passe au privé. Jusqu'à notre énergie, notre eau et peut être bien notre ère qu'ici. Oui il y a un enjeu à renforcer les services publics. Et améliorer leur accessibilité par des recrutements en nombre en renforçant l'attractivité des métiers de la fonction publique, par une meilleure rémunération et par la formation. 500.000 emplois sont nécessaires pour tenir nos objectifs sociaux nos objectifs sanitaires éducatif écologique et économique. Il y a tant à faire. Alors certes, cette résolution aborde le problème mais n'apporte pas de solutions véritables. D'abord parce qu'elle ne présume pas des efforts qui seront mis au budget 2024 et ce n'est bien entendu pas dans la portée d'une résolution. Ensuite parce qu'elle s'intéresse principalement à la question du numérique à son déploiement et à son utilisation. Il me semble d'ailleurs qu'en matière de déploiement, la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize que nous avons voté favorise la déjà l'accès au très haut débit. Alors pourquoi déposer une telle proposition de résolution. Il faut évidemment qu'Internet soit accessible à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. Techniquement, comment en matière de compétences, parce qu'Internet peut faciliter les communications. Et c'est d'ailleurs ce rôle 1er. Il ne doit pas en revanche servir de prétexte pour dégrader nos services publics, pour qu'un enseignant soit face à des milliers d'élèves isolés derrière un ordinateur pour qu'un médecin ausculte sans pouvoir intervenir pour qu'un formulaire soit remplie sans accompagnement. Ni pour que les collectivités se sentent laissées à l'abandon. 84% des démarches administratives. Prioritaire serait déjà accessible en ligne cela et pratique pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Le vrai problème étant que ces mêmes démarches sont de plus en plus difficile d'accès physiquement l'électronique et la précarité numérique concerne un quart de nos concitoyens. Pensons à eux aussi et je dirais même, pensons à eux d'abord puisque ce sont souvent les plus précaires qui sont les plus confrontés au numérique pour leur démarche et parfois découragés. Notre devoir est aussi de lutter contre le non recours. C'est pour toutes ces insuffisances. Malgré ses intentions positives que nous nous abstiendrons donc sur cette résolution, qui n'apporte rien de plus à la PPL Si nous voulons de véritables services publics ce n'est pas avec un clic droit que cela se réglera mais dans les lignes budgétaires du projet de loi de finances, merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Jean Marie Mison pour le groupe Union centriste pour 4 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de résolution de nos collègues du RDSE. Réclame au gouvernement un renforcement de l'accès au service public. À quatre mois des sénatoriales c'est bienvenu. Et le texte de la proposition a bien raison de souligner que le numérique. N'est souvent qu'un cautère sur une jambe de bois, de les territoires ruraux notamment. Prétendre remplacer les services publics par des formulaires en ligne. C'est tout simplement ne pas tout comprendre aux besoins de nos concitoyens. Quand on parle de service public dans nos campagnes aux particuliers. Ce n'est pas à sa dès. À sa déclaration d'impôts en ligne que l'on pense mais en 1er lieu à la santé. Monsieur le Ministre rendez-vous compte une étude récente. De l'Association des maires ruraux de France montre que l'espérance de vie des ruraux. Et des urbains étaient identiques en 1990 mais que l'écart au détriment des ruraux est désormais de 2 ans pour les hommes et près d'un an pour les femmes. Ah. Résultat grandement imputable. À la dégradation de l'accès aux services de soin en zone rurale. C'est dire si le phénomène est allé loin et quand on parle de dégradation de l'accès aux services de soin, c'est autant à l'hôpital dans les structures. Sont supprimés ou débordés que la médecine de ville. Compense, médecine de ville qui. Ne prend plus de nouveaux patients ou alors après des temps d'attente qui se chiffrent en mois pour avoir un rendez vous avec un spécialiste. C'est cela la réalité actuelle de l'accès au service public le plus essentiel qu'qui soit dans les territoires. Face à ce phénomène. Les solutions sont connues, mais elles ne sont pas mises en oeuvre. D'abord pour répondre à la pénurie de médecins. Ma collègue daphné Ract-Madoux vous interrogé hier dans un autre débat sur la revalorisation du statut des professionnels des Des professions paramédicales, pardon. Lorsqu'il n'y a plus de médecin, ce sont les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, les pharmaciens qui interviennent. Ce faisant, ils mettent en jeu leur responsabilité quand allons-nous les protéger leur donnant un vrai statut. Quand allons-nous véritablement faire de la délégation d'actes. Ces questions sont essentielles pour répondre à l'urgence de la situation. Mais. À plus long terme et de manière structurelle la solution est ailleurs. Elle est aussi. Elle aussi est bien connu. Il faut en finir avec. Le pseudo exercice libéral de la médecine. Les médecins ne sont certes pas des fonctionnaires mais ils sont rémunérés par les tarifs de la Sécurité sociale et bénéficie de la liberté d'installation comme une profession libérale. Des rapports du Sénat l'ont réclamée de longue date, dont celui de notre collègue Hervé Maurey. Dans un rapport intitulé déserts médicaux agir vraiment il y a déjà 10 ans. Toutes les professions médicales ou paramédicales sont soumises à des impératifs d'installation territoriales. Il n'y a que les médecins qui peuvent continuer de s'installer là où il le souhaite, cela ne peut plus durer. D'autant moins que les nouvelles générations de médecins, en particulier les femmes sont beaucoup plus ouverte à cette idée que les anciennes générations. Alors à quand le changement. Monsieur le ministre, c'est continuera plus d'écriteaux le cabinet n'acceptent pas de nouveaux patients que l'on pourra vraiment parler de restauration de l'accès de tous au service public. Merci de votre attention.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer l'initiative de notre président Jean-Claude Requier auteur de cette proposition de résolution qui pointe un sujet certes bien connu depuis de nombreuses années mais hélas toujours aussi actuel. Parler de crise du service public, c'est faire renaître une vieille marotte du discours sur l'administration française. Nous pourrions croire qu'il s'agit d'un phénomène né de l'émergence de ce que certains qualifient de néolibéralisme. Et qui a pu conduire à une forme de porosité dans la frontière entre les sphères du public et du privé, il y a du vrai. Il semble que le modèle de l'État providence ne soit plus privilégié depuis longtemps par nos institutions. Les politiques publiques. Désormais des interventions d'acteurs privés tendant à restreindre l'état dans ses seules missions régaliennes. J'ai aussi le sentiment que le service public est né en crise et qu'il a toujours subi des vagues d'attaques et de remise en cause aussi, le Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales, doit tout mettre en oeuvre pour défendre cette Pierre angulaire de la solidarité sociale et de la cohésion territoriale. Le service public et le moyen d'assurer l'égalité dans notre pays. L'égalité de l'accès aux soins de l'accès aux transports, à l'école au service des impôts, de la sécurité d'ailleurs sur ce thème nous traiterons aussi dans quelques jours, des moyens budgétaires de la justice. Il devrait continuer d'augmenter d'être conséquent dans les années à venir cette tendance doit s'élargir aux autres administrations. Ce n'est pas la première fois que notre groupe s'inquiète de l'état des services publics dans notre pays. Le président là requis a rappelé tout à l'heure, que ce soit à l'occasion des travaux de Raymond Vall sur 10 l'acte Ronis ou se Alain Bertrand. Sur l'hyper-, ruralité, l'un comme l'autre souligner à quel point nos territoires se situer dans une forme de précarité administrative que le numérique était bien incapables de combler. Depuis 2 ans nous avons consacré dans la loi le principe de différenciation territoriale. Je crois qu'il faut qu'il s'associe au service public. Le cas de la ruralité, l'illustre parfaitement derrière ce mot nous trouvons des territoires aux caractéristiques souvent très différentes. La ruralité rassemble comme dans les zones urbaines, des populations hétérogènes, qui ont des modes de vie très différemment. Cette diversité est source de difficultés pour l'emploi l'implantation des services administratifs. Pardon, parce qu'il est nécessaire d'adapter les politiques publiques au plus près des besoins de chaque territoire. Certes il existe un socle commun de service indispensable mais il est nécessaire d'adapter les dispositifs nationaux aux populations des zones rurales. Cela doit passer par un accompagnement des projets locaux, le groupe RDSE est à l'origine de l'initiative parlementaire qui a permis la mise en place de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Le bilan de son action et peut être encore insuffisant mais cette insuffisance ne tient qu'à l'étendue des défis auxquels elle est confrontée. D'une autre manière non saluant la mise en place du réseau France ce service créé en 2019 et l'établissement de maisons de service au public, même si le maillage territorial reste à parfaire et les services qui sont apportées à renforcer nous identifiant néanmoins des progrès à faire et de ce point de vue le manque de moyens, les mains que de moyens se font largement sentir et nous appelons de nos voeux la pérennisation des moyens. Voire un accompagnement supplémentaire aux collectivités qui ont relevé relever le défi de créer des espaces un service. Oui la question des moyens et fondamental. Nous pourrons établir tous les plans et schémas possibles, je pense au schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public ou encore le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires toute programmation sera vaine, si elle ne s'accompagne pas de son pendant budgétaire. Les réponses apportées à ces problématiques et ne se trouveront pas dans le réflexe hélas trop courant de la dématérialisation, certes il permet d'éviter des files d'attente aux guichets ou des déplacements chronophage et de ce point de vue il faut y voir incontestablement une facilité pour de très nombreux citoyens. Faut-il encore que l'administrer soit à même de recourir à cet outil Je crois qu'il est possible de trouver d'autres solutions, le numérique n'a pas le monopole de la simplification au contraire si simplifie parfois il peut aussi privé certains usagers de toute autonomie. J'entends qu'il faille poursuivre de développer ses services. Mais il faut aussi les adapter pour nos concitoyens qui souffrent de ne pas savoir s'en servir et surtout il est impératif que la digitalisation se fasse en parallèle et non un lieu et place du développement des guichets physiques pour qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée tout ce ces remarques vont donc dans le bon sens et dans le sens de la proposition débattue et nous voterons bien entendu unanimement en faveur de son adoption, je vous remercie. Merci cher collègue. Là. Parole et maintenant Monsieur Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, chers collègues. Et s'il y a bien une prérogative à laquelle les Français n'ont cessé d'exprimer leur attachement, c'est celle de l'accès à leurs services publics. Le service public est constitutif de notre identité française par la multitude de secteurs auxquels il apporte son concours le haut niveau d'intervention qui est attendu de l'État doit s'accompagner d'un haut niveau d'efficience et de performance. C'est pour ces raisons que le désengagement progressif de l'État dans certains territoires paraît d'autant plus déconcertants pour nos concitoyens. Le sentiment d'abandon gagne du terrain. Le lien de confiance entre administrés et administration s'étiole. Il concerne plus particulièrement les territoires ruraux, qui rappelons-le rassemble encore 88% de nos communes et plus d'un Français sur 3 dans une logique de renforcement de la performance publique de l'État, illustré en matière financière par la LOLF. Les services publics ont opéré un vaste mouvement de transformation au détriment parfois. De leur accessibilité au grand public. Fermeture de bureaux de poste de trésorerie de guichets, Pôle emploi ou la sécurité sociale mais aussi des classements des petites lignes ferroviaires du réseau d'intérêt local. Fermeture de lits d'hôpitaux et quasi systématiquement sur la compensation suffisante pour assurer leur bonne performance les moyens n'ont pas d'ailleurs toujours été accompagner adéquatement. La hausse de fréquentation de certains services par exemple le guichet de paiement des amendes de Seine-Saint-Denis qui bien qu'il recouvre une population de plus d'1,6 millions d'habitants ne propose que 9h d'ouverture hebdomadaire au public. Voilà un témoignage parlant de dysfonctionnements sérieux d'un service public pourtant indispensable à la vie quotidienne de milliers d'individus. La dématérialisation des procédures administratives si elle témoigne un investissement déterminant de l'État dans le numérique. C'était la fête à marche forcée pour beaucoup de nos concitoyens. Il convient de rappeler que plus de 14 millions de Français éprouvent encore des difficultés avec la compréhension et l'utilisation des plateformes digitales des services publics dans mon département de laine, l'État a mis sur pied en mars 2021 un vaste plan quadriennal de lutte contre l'illettrisme et l'électronicien décomposé en 4 axes et 20. Dédié à l'amélioration de l'offre de formation à destination des personnes en difficulté. De telles démarches doivent être encouragées et approfondie partout dans le pays. Les zones blanches téléphonique reste une autre préoccupation majeure des territoires concernés, autant que l'absence de très haut débit, il est indispensable que l'État a fermé son rôle de contraintes auprès des opérateurs. Parmi les solutions déjà dégagé pour résorber le problème le recrutement de conseiller numérique ou le fléchage de 250 millions d'euros dans le cadre du plan France relance, sont des éléments encourageants mais qui demeure encore bien insuffisant face à l'ampleur de la fracture numérique. Afin d'approfondir ces solutions. Le débat sera peut être appelé à terme à porter sur une réflexion élargie sur le rôle des territoires pour notre République et sur le niveau de la confiance que le gouvernement sera disposé à leur accorder. Il ne paraît en somme pas acceptable d'imposer sur le long terme une vision purement comptable et financière, sur des services régissant la vie quotidienne de nos concitoyens. Le maintien d'un interlocuteur physique en dernier recours et l'une des préconisations mise en valeur par la proposition de résolution, il doit rester la règle et non l'exception. Un accent doit aussi être porté sur le renforcement de l'attractivité des métiers de la fonction publique en relation avec l'usager. Un tel objectif passera nécessairement par une revalorisation des carrières et des grilles indiciaires. Dans les territoires, la constitution de pôles centralisé mutualiser et facile d'accès doit se pour Les progrès permis par le déploiement des 2378 maison France Service compter en janvier 2022 doivent être salué des améliorations peuvent toutefois être sur la accessibilité car moins de 25% d'entre elles étaient à l'heure actuelle accessible en transports en commun. Il faut rappeler en outre le rôle que les acteurs locaux peuvent jouer sinon substitution du moins en complémentarité avec les administrations publiques, les missions locales ont par exemple trouvé à cet effet. Leur valeur ajoutée pour renforcer l'action de Pôle Emploi dans les politiques d'insertion et d'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. En somme, le véritable enjeu de l'accès au service public et celui de l'accès à la démocratie, la démocratie fonctionne. Du moment qu'elle est intelligible aux concitoyens les services publics doivent inscrire leur action au service de cette intelligibilité notre groupe salue donc l'ambition et la portée de la proposition de résolution nos collègues du groupe RDSE qu'elle votera tout en rappelant avec force les travaux rendus par le Sénat, de manière constante depuis plus d'une dizaine d'années et qui n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la désaffectation des services publics dans les territoires. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant Madame Martine Filleul pour le groupe socialiste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur Jean-Claude Requier auteur de la proposition de résolution, chers collègues. Les services publics jouent ce rôle fondamental de servir l'intérêt général en soustrayant certaines activités à la logique du marché et à la recherche du profit, il nous appartient de protéger cet héritage menacé par un délitement progressif qui remettent en cause la base de notre contrat social. Aujourd'hui l'administration dématérialisée provoque un sentiment d'abandon et cristallise les tensions. Tensions chez les Français tout d'abord chez ses 13 millions de personnes en situation d'illectronisme, véritable illettrisme du XXIe siècle. Il touche toutes les classes sociales et toutes les générations, contrairement à aux idées aux aux idées habituellement reçues, il est davantage présent parmi nos concitoyens les plus précaires, ceux pour qui l'accès à l'information et l'utilisation de leurs droits sont plus que primordiaux. Au-delà, même pour ceux qui utilisent aisément les outils numériques, la complexité des procédures le jargon employé les erreurs de dossier reste un obstacle à la jouissance des droits. Chers collègues, rappelez-vous, autrefois on remplit comme on pouvait le formulaire Cerfa et une fois au guichet, on le compléter avec un agent du service public. Aujourd'hui, ce même formulaire Cerfa dématérialisé. Il n'est plus possible de s'entretenir avec un agent par souci d'économie, l'usager est devenu un agent du service public. Tensions également chez les élus locaux cette dématérialisation à marche forcée des services publics a été encore plus douloureusement vécue dans le monde rural. Je le constate chaque semaine lors des rencontres avec les maires de mon département les secrétaires de mairie sont sur-sollicités par les administrés pour les assister dans leurs démarches. À tel point que la collectivité souvent obligés de soutenir complémentaire ment des associations pour les pour les aider une nouvelle fois l'État se décharge sur les communes alors oui le dispositif des conseillers numérique est une première étape dans le processus de monter en compétences numériques des citoyens et par conséquent d'être fortement renforcés compte au maison France Service. Elles offrent un service très inégale selon les endroits. Si cette certaines apporte toutes celles qui s'factions. D'autres sont par contre de réels coquille vide mais, contrairement aux déclarations pour encore beaucoup de Français aucune alternative ou téléphonique n'est proposé. La défenseure des droits la rappeler encore très récemment. Il est aujourd'hui plus que nécessaire et urgent de mettre en place une véritable politique publique d'inclusion numérique cohérentes complètes et digne de ce nom. Celle-ci doit s'attaquer au problème par toutes les cibles et partout les angles et nécessite un financement à la hauteur de l'enjeu pour traiter ce mal à la source, à l'école par un apprentissage plus approfondie des outils numériques et par et par ailleurs le développement indispensable de l'aller vers qui est absolument incontournable. Ainsi la question de l'accès au service public hé bien celle de l'accès au droit d'un accès au droit, rendu aujourd'hui difficile et qui pour les naufragés du numérique vire parfois à la détresse humaine et sociale, la nécessité de renforcer tous les modes d'accès au service public est un impératif auquel nous souscrivons. C'est pourquoi, comme l'a déjà dit mon collègue Patrice Joly. Le groupe socialiste votera pour cette proposition de résolution, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant ma de madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il n'y aura pas de république sans services publics sur notre territoire. Ce slogan pourrait résumer l'ambition de la présente proposition de résolution. Nous ne pouvons qu'y souscrire. Il faut immédiatement ajouté que le numérique ne pourra pas totalement se substituer au service public traditionnel. Une problématique essentielle à laquelle le texte de la proposition de résolution consacre à juste titre l'essentiel de ses développements. Les limites du numérique sont connues. Je pense tout d'abord à la persistance de l'illectronisme, fléau à l'origine de multiples fractures. Une fracture générationnelle puisque les seniors sont souvent moins à l'aise avec l'informatique que les jeunes une fracture sociale car les classes populaires sont plus facilement perdus par le numérique que les classes aisées. Enfin une fracture territoriale entre urbains et ruraux en effet loin d'aider les zones rurales. Dématérialisée les services publics ne fait que les enclaves. Un peu plus. Anne. Outre les territoires ruraux se heurte à un problème d'accès matériel au numérique. C'est tout le problème du déploiement de la fibre et de la couverture des zones blanches hélas la fibre est trop fréquemment déployée à la hussarde, c'est pour faire cesser ces pratiques que le Sénat a voté la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Nous espérons qu'elle prospère aura l'examen de la présente proposition de résolution est une bonne occasion, Monsieur le Ministre, de vous interroger à nouveau sur vos intentions vis-à-vis de ce texte. La seconde grande limite du numérique pour renforcer l'accès de tous au service public tient au fait que tous les services publics ne sont pas numérisables. Il en va ainsi de l'école. Certes les effectifs scolarisés au sein du 1er degré de l'enseignement public ont amorcé une décrue au cours des dernières années. Mais cela ne doit pas impliquer de supprimer des postes à due proportion. Ces suppressions n'ont pas le même même pas de selon elle se situe en zone rurale ou les classes restantes seront surchargés ou en zone urbaine ou la redistribution des effectifs sur les classes ou établissements de proximité et plus aisée. C'est pourquoi une véritable approche prospective territoriale doit être effectué au cas par cas, en prenant en compte l'urbanisation à venir dans les territoires et non les zones les effectifs à l'instant T. Par ailleurs, des effectifs moins élevé dans les classes ou permettront des enseignements de meilleure qualité, notre classement Pisa devrait s'en trouver amélioré. Mais l'école est loin d'être le seul service public non numérisables en régression je tiens ainsi a évoqué le cas du service postal. Face à la récente réévaluation très conséquente de la mission d'aménagement du territoire, confie à la Poste portant son montant Net à 325 millions d'euros. Il apparaît paradoxal que des décisions de fermeture de bureaux ou des diminutions d'horaires non concertée au niveau des bassins de vie et remettant en cause l'aménagement du territoire en zone rurale, soit encore reprise dans les départements. Pour toutes ces raisons, je ne peux que remercier les membres du groupe RDSE d'avoir déposé la présente proposition de résolution que mon groupe de l'Union centriste votera évidemment je vous remercie. La parole est maintenant Madame Martine Berthet pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette proposition de résolution et le débat d'hier pointe toute l'importance des services publics dans l'attractivité et le dynamisme de nos territoires, tant en matière de droits sociaux d'emploi, de santé ou d'éducation que de mobilité ou d'économie d'état civil ou de justice domaines essentiels à la vie quotidienne de nos concitoyens. Si des politiques publiques palliatives ont été mises en oeuvre au fil du temps la notion même d'accessibilité aux services publics, qu'elles soient physiques par les transports ou intellectuelle face à l'île électroniquement a été trop souvent oubliées. Parmi les mesures récentes il est à noter le déploiement des 2006 des 2600 maison France Service qui apporte certes un 1er niveau de satisfaction. Mais au moment de lancer pour le gouvernement du nouveau dispositif France ruralité. Monsieur le Ministre, beaucoup reste à faire. Si chacun a une maison France Service à 30 minutes de chez lui comme cela nous a été dit hier par votre collègue 30 minutes c'est loin ça coûte du carburant qui est cher et comment s'y rendre quand on n'a pas de voiture. L'engagement de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales est indispensable en termes de visibilité du financement pour pérenniser le dispositif et sa participation doit être portée à 50.000 euros pour un engagement à la hauteur des besoins. Il est par ailleurs nécessaire que les opérateurs jouent pleinement leur rôle du second niveau en étant réactifs aux questions des agents d'accueil des France service on observe trop souvent des inégalités de réponse des opérateurs selon les départements et d'un opérateur à un autre, ils doivent respecter les critères les maison France services ont été audités pour être labellisée les opérateurs non. Ils se doivent aussi d'assurer la formation continue des agents France service de façon régulière et pertinente. Il est à noter que malgré des engagements pris par la haine, c'était les fiches de postes de ses agents n'ont toujours pas été réalisé. Pour terminer sur les France service leur déploiement doit s'adapter au contexte locaux. Je pense par exemple aux territoires de montagne et touristique. Pénalisé par une lecture stricte des critères concernant l'ouverture et le nombre de personnes d'accueil en période creuse comme des espaces saisonniers de mon département de la Savoie qui n'ont pu tous être labellisé. Le maillage de ces espaces doit aussi c'est s'effectuer en milieu urbain, car ce sont à présent les villes qui souffrent de la fermeture des accueille des opérateurs. Il est nécessaire d'articuler les acteurs et les démarches au niveau des différentes échelles territoriales. Il y a avec les communes pour une bonne information une bonne orientation des administrés schémas de service au niveau territorial SIDA qui a montré toute son utilité, pour le dialogue entre les collectivités, les opérateurs France service l'État et le département. L'animation départemental des France service est importante car les conditions de fonctionnement d'encadrement et d'implication sont très différentes des unes aux autres. Le 4 mai dernier, en réponse à ma question écrite du 29 septembre 2022. Concernant la pro, la prolongation des oeufs d'Aspe. Vous m'avez répondu, Monsieur le Ministre qu'une mission relative aux modalités d'accès aux services publics étaient en cours. Pouvez-vous nous en dire plus. Je ne terminerai pas sans parler de la question du numérique, une simplification des portails des opérateurs nationaux des formulaires et du vocabulaire et plus que souhaité comme pointée par le défenseur des droits et la Cour des comptes, une amplification des politiques d'inclusion numérique à destination des différents publics et la définition d'un chef de file de l'inclusion numérique afin de garantir la coordination et l'égalité territoriale sont nécessaires. La présence du très haut débit qui paraît être en 2023, une condition sine qua none à la vie dans nos territoires pour l'accès à l'ensemble des services que sont aussi la télémédecine et le télétravail ne va pas assez vite. En conclusion, Monsieur le Ministre, le déploiement du numérique pour un meilleur accès au service public ne doit pas oblitérer l'intérêt de la proximité physique des locaux. Du maintien des réseaux thématiques de proximité dont l'accueil social de proximité, de l'accès, conservé aux opérateurs de la nécessité d'un interlocuteur identifié et opérationnel pour l'ensemble de nos aussi concitoyens porté par cette proposition de résolution. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Monsieur Guillaume Chevrollier. Pour le groupe Les Républicains pour. Cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de résolution proposant au gouvernement de renforcer l'accès au service public. Mais je pense aussi à l'accès à la santé si préoccupant dans nos territoires ruraux. Ce texte insiste sur la nécessité de renforcer tous les modes d'accès au service public et de prévoir dans le même temps un partenariat plus équitable entre l'État et les collectivités locales. Il revient sur le besoin de proximité très largement exprimés par nos concitoyens des territoires ruraux en matière d'accès au service public. En effet, ces dernières années les communes rurales ont été particulièrement affectées par le regroupement et la disparition des services publics. Cela s'est accompagné d'une dématérialisation croissante des démarches administratives. Or en creux ce phénomène pose la question de l'égalité d'accès des citoyens devant leurs droits. Aujourd'hui 13 millions de Français sont touchés par l'île électronique. La population concernée et souvent âgées précaires. La numérisation croissante des services publics. Peut potentiellement produire pour elle des effets délétères. Entraînant finalement une certaine forme d'abandon de la part de l'État. Certes, plusieurs dispositifs ont été déployés depuis néanmoins des angles morts non négligeables demeure. Dans ce contexte, il me semble que nous pouvons définir trois axes d'actions pour améliorer l'accès aux services publics dans le territoire en prenant en compte le paramètre numérique. Dans un 1er temps, l'accès aux services publics dématérialisés nécessite le renforcement. De notre De notre infrastructure technique partout sur le territoire. Or encore aujourd'hui des différences substantielles de débit dans les connexions internet entre les zones urbaines et rurales subsiste la connexion Internet de certains territoires repose toujours largement sur le réseau cuivre voué à disparaître en 2030 faute d'un déploiement complet de la fibre aujourd'hui. La diminution des Budgets d'entretien la sensibilité du réseau et sa vulnérabilité en cas de coupure d'électricité, suscite de nombreuses inquiétudes notamment sur les capacités de communication avec les services publics de secours des réponses adaptées doivent être apportées. Enfin, si nous voulons garantir l'accès de tous au service public, il faut renforcer les dispositifs d'assistance et d'accompagnement numérique des populations en situation d'l'électronicien. En effet, alors que les démarches administratives numérique ne nécessite plus l'intermédiaire d'un nageur expérimenté ou de moins en moins, certains usagers se retrouvent livrés à eux-mêmes et finissent par renoncer à leurs droits. Les conseillers numériques ont été déployés. Mais leur contrat sont temporaires, avec une part de financement de l'État dégressive. Même si des mesures de pérennisation ont été annoncées les modalités de financement et de professionnalisation de ses employes reste. S'agissant de la lutte contre lui l'électronicien. Les personnes concernées sont très souvent isolées précaires ou âgés, elles n'ont pas toujours les moyens de s'équiper en matériel informatique ou la possibilité de se déplacer poursuivent des ateliers de formation. Ces populations se concentrent très souvent dans des zones de revitalisation rurale, il convient donc de cibler ces publics plus vulnérables et de mieux former les acteurs des services publics qui peuvent les accompagner dans leurs démarches. Il est également essentiel de garantir des moyens d'accès alternatif au service public. Nous ne pouvons envisager pour le moment un accès exclusif par voie numérique, et Monsieur le Ministre, nos concitoyens demandent vraiment des relations humaines et ça me semble justifié. Enfin je rappellerai que. Comme au début de mon intervention, l'État a fourni quelques efforts pour accompagner la numérisation des services publics via les structures labellisée France services et des schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services publics. Toutefois, ces dispositifs manque de lisibilité clarté ils viennent se superposer à l'action les municipalités de l'Agence nationale la cohésion des territoires ou des préfets. Il s'agit donc de gagner en cohérence en structurant les différentes échelles d'action. Aujourd'hui les collectivités. Des collectivités concours à la réalisation de services publics qui ne dépendent pas toujours d'elle et qui mobilise pourtant leurs propres moyens. Le financement actuel de ces coûts par l'État génère des des restes à charge importants. Le gouvernement a annoncé le déblocage de fonds supplémentaires mais il serait souhaitable de mettre en place un système de financement pérenne et équitable, le maillage territorial des maison France Service gagnera également à être affiné et complété par d'autres moyens, le cas échéant en 1000 moyens itinérant afin de rendre plus facile l'accès au dernier kilomètre pour les personnes qui ne se. Que difficilement. Monsieur le Ministre, la question de la mobilité reste un enjeu majeur notamment dans nos territoires ruraux ainsi cette proposition de résolution pourra servir de base à une réflexion autour d'une stratégie claire et de long terme permettant de rétablir la proximité et l'accessibilité des services publics partout et pour tous en lien avec nos communes et avec nos élus. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains votera pour son adoption. Je vous remercie. Merci cher collègue remarquables. La parole est maintenant monsieur Stanislas Guerini Ministre de la Transformation et de la fonction publique. Monsieur le président. Monsieur le Président, Ruquier, mesdames messieurs les les sénateurs. Oui, le principe d'égalité des droits. Vous l'avez rappelé monsieur le président, est au coeur de notre pacte républicain. Oui, l'accès au service public partout et pour tous. C'est le fondement de, de notre cohésion sociale. Oui. La dématérialisation de démarches administratives et souvent utile, mais elle doit s'accompagner d'une couverture numérique de qualité pour tous nos territoires et de l'accompagnement de ceux qui en sont le plus éloignés. Et oui nous. Agissons en même temps. De manière résolue afin que la numérisation de nos usages ne rime jamais avec la déshumanisation de nos services publics, vous l'avez dit en déployant moins de 3 ans 2600 Space France, service des milliers de conseillers numérique France service également. Vous le voyez, Monsieur le Président, Ruquier. Le gouvernement partage le constat que vous dressez. Et c'est tout l'objet de nos actions pour renforcer l'accès et la qualité de nos services publics. C'est précisément pour cela que la Première ministre a fait le choix de rassembler de réunir l'ensemble du gouvernement le 9 mai dernier à l'occasion d'un comité interministériel de la transformation publique pour mobiliser l'ensemble de l'action gouvernementale pour renforcer la qualité de nos services publics. je voudrais, à l'occasion de cette résolution de je voudrais vous remercier revenir ici sur 3 priorités que je porte pour rendre service public plus accessible, plus attractif, qualitatif. D'abord assurer ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de nos services publics ensuite mettre en place un accompagnement privilégié particulier pour celles et ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Et puis enfin. Prendre soin porté une attention particulière aux agents publics, je crois que c'est une condition pour réussir et relevé l'objectif de renforcer l'accès à nos services publics. Je le disais, la première priorité c'est les fondamentaux de nos services publics. Les Français ont des attentes simples vis-à-vis de nos services. Je suis, vous avez très bien exprimé, je dirais au nombre de 3. D'abord la question des délais. C'est le principal sujet sur lequel il nous sollicitent quotidiennement et c'est vrai de tous nos services publics 2ème attente c'est de pouvoir parler à quelqu'un, tout simplement. Quand on est très éloigné du numérique, mais aussi tout simplement quand on est bloqué sur une démarche administrative qu'on ne comprend pas ou qui ne fonctionne pas en ligne ou qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un au téléphone puis la 3ème demande légitime, c'est de ne pas être baladé d'une administration à une autre. Vous savez que quand on donne une information, une fois elle soit réputé donner définitivement pour l'ensemble des administrations auxquelles nous sommes confrontés. Alors pour répondre à ces deux attends je partage de conviction de méthode. La première c'est de ne jamais opposé numériques et physiques, c'est que je crois que notre point de vigilance et d'avoir une attention portée sur tous les canaux d'accès à nos services publics je vais est revenu 2ème conviction de méthode, c'est de ne pas simplifier pour simplifier. Simplifier en partant de la ville, les gens en partant des moments dans la vie de nos concitoyens où ils ont besoin d'avoir accès à nos services publics. Je crois profondément à cette méthode là et c'est fort de ses convictions que nous avons pris des décisions fortes à l'occasion du comité inter-. La transformation publique pour améliorer tous les canaux d'accès. À nos services publics je commence. D'un mot, par le téléphone. Je crois que vous l'avez dit les uns et les autres caractère insupportable de devoir attends de n'avoir personne en ligne de faire du numéro 1 à 12 pour se contacter tel ou tel service c'est quelque chose que nous avons tous les uns et les autres vécu et donc nous devons avoir une mobilisation accrue sur la qualité de l'accueil téléphonique. Nous avons lancé un nouveau plan pour renforcer la qualité de l'accueil téléphonique, avec des objectifs très clairs, un taux de décrocher supérieure à 9 fois sur 10 dans l'année qui est devant nous établir un outil de mesure de la satisfaction des usagers qui ont contacté ou essayer de contacter une administration au téléphone et développer aussi, c'est un engagement très concret, la possibilité de prendre rendez-vous d'être rappelé par une administration quand on en formule la demande. Je veux aussi dire notre mobilisation pour renforcer la qualité du numérique que vous nous devons apporter je pas tenir ici. Un discours qui est parfois une facilité, on parle du numérique que de façon négative, au fond, il faut faire du bon numérique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de démarches que nous devons pouvoir numériser parce que ça correspond aux attentes de nos concitoyens parce qu'aujourd'hui déjà plus de 9 fois sur 10 les interactions de nos concitoyens se font via le numérique, mais faire du bon numérique c'est d'abord faire du numérique qui soit accessible à tous, vous l'avez rappelé, les uns et les autres sur les démarches est censé les 250 démarche qui sont utilisés par plus de 200.000 Français chaque année, nous avons un taux de numérisation de ces démarches qui est désormais acceptable. Plus de 94% et pour autant, je prends un sujet très concrets. L'accès. Numérique aux personnes qui sont en situation de handicap. Nous sommes en retard sur ces questions là faire du monde numérique c'est faire par exemple du numérique, accessible à nos concitoyens qui sont en situation de handicap et dès lors nous renforcerons ce 1er niveau d'accessibilité c'est faire du numérique où on répond à la promesse, dites-le nous une fois c'est-à-dire que les informations, je le disais, sont partagés entre les administrations et puis je le disais, d'un mot sur la méthode, nous devons simplifier le quotidien des Français sur les principaux moments de leur vie quotidienne. C'est pour ça que nous avons choisi de travailler par moments de la vie de nos concitoyens pour poursuivent des objectifs cruciaux. Répondre à ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans ces moments particuliers appliquer le droit à l'erreur. Faire le dites-le nous une fois améliorer l'ensemble du parcours usagers je cite des cinq moments de vie que nous avons choisi de traiter de façon Le fait de devenir étudiant, on sait que c'est un moment très particulier où il y a beaucoup de complexité parfois pour l'accès au logement, c'est un engagement très clair le fait de renouveler évidemment son identité. Nous manquons de ton de temps ici pour aborder ce sujet en détail mais les objectifs sont très clairs de diviser par deux les délais c'était encore à l'occasion des questions au gouvernement. Une question posée à très juste titre, le fait de partir à l'étranger pour expérimenter la dématérialisation du renouvellement des titres pour les Français de l'étranger qui pour le coup est appelé de leurs voeux. Le fait de rénover son logement. On sait parfois la complexité de l'accès aux aides sur cette politique publique et donc de mobiliser notamment le réseau France service sur cette dimension particulière et enfin le fait de perdre un proche, ce sont des moments d'une grande brutalité vécue par 8 à 10% de nos concitoyens chaque année et donc nous devons être plus proactif dans le versement notamment de la pension de réversion, ou l'accompagnement volontaire des veuves et des veufs dans leurs démarches. Ça ce sont des moments fondamentaux je dirais qui concerne l'ensemble de nos concitoyens et puis vous l'avez dit à juste titre. Il faut avoir une concentration accrue sur ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux de nos concitoyens qui sont. Soit intrinsèquement éloignés du numérique. Vous avez mentionné des exemples de personnes parfois âgés sont parfois aussi des jeunes qui sont à l'aise sur un téléphone portable mais beaucoup moins à l'aise quand il s'agit de remplir une démarche en ligne sont parfois des gens frappés de l'illectronisme elle et de cette frontière que vous avez à juste titre, rappeler et pour cela oui. Nous devons avoir un service public particulièrement accessible et de façon physique, il faut des voies et c'est pour ça que, notamment, mais l'investissement que nous mettons dans le réseau France service et indépendant. De la réponse que nous devons apporter France service ça fonctionne aujourd'hui ce sont 2600 espace à moins de 30 minutes pour 98% de nos concitoyens à moins de 20 minutes aujourd'hui pour en 92% d'entre eux ça marche aussi parce que il y a des démarches sont qualitative. Je rappelle souvent mais 8 fois sur 10, quelqu'un qui sort d'un espace France service il a eu sa démarche administrative traités et les retours sont bons aujourd'hui sur cette question là. Alors est-ce qu'on nous devons nous arrêter. Absolument pas, nous devons au contraire poursuivre, poursuivre l'investissement dans. Le réseau des espaces France service le faire à partir des territoires. J'ai annoncé que nous finançons et nous avons sanctuarisé ce budget pour financer la l'ouverture de 150 espace France service supplémentaires dès l'année 2023, nous allons renforcer le financement apporté à chacun des rend service dans un n'esprit une démarche partenariale avec les collectivités territoriales qui prennent une part très fort dans le financement d'espace rend service tu sais les 12 millions et demi d'euros mobilisé et voté au Sénat c'était un amendement du sénateur Delcros supplémentaires pour passer dès cette année, le ticket de financement de 30.000 à 35.000 euros pour chacun d'espaces française et nous devons poursuivre cette trajectoire en mobilisant les opérateurs nous allons le faire, nous devons aussi renforcer la formation j'ai annoncé que nous allons doubler le temps de formation des agents France service en mobilisant là aussi les opérateurs élargir le bouquet de services qui a apporté à nos concitoyens. Je pense aux expérimentations que nous menons avec les Crous avec la Banque de France avec aussi ma prime Rénov'pour intégrer cette politique publique dans le réseau France service et donc nous allons monter en puissance sur cette politique publique essentielle. Je veux aujourd'hui dans le temps qui m'est consacré aussi conclure peut-être par un élément qui a été moins évoqué mais qui est la tension que nous devons porter aux agents de service public. Si nous voulons relever ces défis que je crois que nous partageons. Alors il nous faut relever le défi de l'attractivité de la fonction publique, c'est souvent l'occasion de nos échanges et je veux le dire en rendant un hommage particulier à celles et ceux qui rend le service public. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, ces derniers jours encore, ont donné leur vie en faisant leur métier, c'est-à-dire de rendre le service au public. Nous leur devons beaucoup. Nous devons mieux les protéger leur permettre d'avoir des parcours de carrière plus diversifié des rémunérations aussi plus attractive. C'est l'objet du dialogue social intense qui est menée sur ces questions là, mais nous devons aussi améliorer leurs conditions de travail. Le première employeur du pays doit penser les questions de transformations du rapport au travail doit s'engager sur des promesses employeurs sur l'amélioration de l'organisation des services. La question de temps de travail. Les transformations des espaces de travail, la question de la santé au travail ou encore celle de l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous a rassemblés il y a quelques jours encore sur les bancs du Sénat par ce que si nos services publics fonctionnent et si je crois que notre ambition partagée pour l'amélioration de nos services publics. Doit être relevé. c'est grâce aux hommes et aux femmes qui rendent le service au quotidien, que nous pourrons réussir et donc je conclus Monsieur le Président, Ruquier et l'ensemble de votre groupe d'avoir porté cette résolution. Je veux dire mon avis favorable sur ce texte. d'ambition partagée et vous pouvez compter sur ma détermination pour agir à vos côtés mesdames et messieurs les sénateurs, pour renforcer l'accès à nos services publics. Merci, monsieur le Ministre. Chers collègues, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution, la conférence des présidents, a décidé que les interventions des orateurs. Explications de vote, je mais aux voix, la proposition de résolution qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition est adoptée. chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance jeudi 1er juin à 10h 30 pour l'examen d'une demande de création d'une commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique puis pour les questions orales. La séance est levée.